informé le Sénat que les candidatures ont été publiés pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance actuellement en cours d'examen ces candidatures seront ratifiés si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations est parvenu à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la désignation des 27 membres de la mission d'information sur la réinsertion des mineurs enfermés, créée à l'initiative du groupe, la République en marche, en application du droit de tirage prévu par l'article 6 bis de notre règlement, en application de l'article 8 alinéa 3 à 11 et l'article 110 de notre règlement, la liste des candidats établie par les groupes a été publié, elle sera donc ratifier si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure. Monsieur le ministre, mais chers collègues aussi heureux de saluer la présence. Dans tribunes des auditrices et des auditeurs de la 3ème promotion de l'institut du Sénat, le bureau du Sénat avait décidé en 2015, à l'initiative de notre ancien collègue Jean-Léonce Dupont, de mettre en oeuvre ce programme de formation en vue de mieux faire connaître les modalités de fonctionnement et les enjeux de notre démocratie parlementaire des personnalités diverses, les 20 auditeurs de cette 3ème promotion qui viennent départements différents, sont issus de tous les secteurs socio-professionnels, ils sont étudiants, fonctionnaires, responsables syndicaux, dirigeants d'entreprise notaire chirurgien exploitants agricoles ou encore journalistes tout au long de leurs travaux, qui ont commencé hier et s'achèveront fin juin il rencontreront dans le cadre d'ateliers organisés à leur intention, plusieurs de nos collègues sénateurs et les fonctionnaires du Sénat en votre nom à tous, je leur souhaite une excellente session au Sénat et je suis certain qu'à l'issue, c'est 3 mois, ils pourront être les témoins privilégiés de la place essentielle de notre institution au sein de la Ve République et de la qualité du travail parlementaire. Mais, chers collègues, l'ordre du jour, appelle à la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée pour un État au un État au service d'une société de confiance dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 146 au sein de l'article. 15 ans et c'est Monsieur Collombat qui le présente. Merci monsieur le président et chers collègues cette cette article est très représentatif de la nature de ce texte. Moi foi la proposition qui est faite, c'est-à-dire de mettre à disposition un numéro téléphonique qui ne soit pas surtaxé pour les usagers des administrations.

Pour pouvoir le dire, hé bien nous avions pensé déposer un amendement de suppression me pouvoir supprimer une aussi belle réalisation, on va le retirer. Dont acte cher collègue, l'amendement est retiré et nous en venons à l'amendement numéro 76 kilos présente Madame Lepage. Merci monsieur le président, mes chers collègues, tout d'abord je tiens à exprimer mon vif regret que cette mise à moment se soit vu opposer l'article 41 de la Constitution alors même que, de par leur objet, leur disposition il s'inscrivait pleinement dans l'esprit du texte ma déception est partagée par mes collègues représentant les Français établis hors de France et sera partagé également par les 3 millions de Français résidant hors de France, j'en viens à l'objet de mon amendement qui lui n'a pas été retoqué pour les Français établis hors de France, tout comme pour les compatriotes de passage à l'étranger pour des raisons touristiques ou professionnels, il peut être très difficile de joindre une administration par téléphone car le numéro mis à la disposition du public n'est parfois tout simplement pas accessible depuis l'étranger, cet amendement vise donc à s'assurer que toutes les administrations mettent à la disposition du public un numéro téléphonique non non surtaxé mais également accessible depuis l'étranger. Merci monsieur le président. Alors l'objet de l'amendement est, semble-t-il, de permettre aux Français établis hors de France de joints des administrations de l'État depuis l'étranger, mais le dispositif de l'amendement modifie le texte adopté en commission, sans que cet ajustement correspondent aux intentions de leurs auteurs, au demeurant, je précise que si les numéros courts ou certains numéros en 08 ne sont pas joignables depuis l'étranger, la plupart des services publics mettent à disposition un numéro de téléphone joignable depuis l'international, en plus du numéro du numéro court joignable en France, c'est par exemple le cas de l'assurance-maladie, de l'assurance vieillesse de Pôle emploi donc pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable pour les mêmes raisons que la commission, j'ajoute que l'article que nous discutons, a une portée générale, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux Français, en métropole comme en France à l'étranger, ce qui implique, pour le gouvernement de veiller à ce que les numéros sont accessibles comme Madame Lepage le demande au nom des Français de l'étranger.

notre avis Colomba sincèrement. Mais où est-ce qu'on est. C'est le sénat de la République et le sénat de la République en est à débattre de savoir si on veut créer un numéro de téléphone et si ce numéro de téléphone doit être ou pas habilité à être joint pas joint tout et la prochaine fois, faites-nous faire les circulaire même pas le même pas les décrets et les circulaires franchement l'abaissement du Parlement à ce point, il y a des limites, je voterai ce qu'on voudra, mais où est-ce qu'on eu quoi, enfin je demande vraiment au président du Sénat. De dire clairement qu'il y a un article 41 articles, 41 et un article 45 et puis il y a la constitution de la République qui fait la différence entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire et si on en met là-bas, ne vous étonnez pas qu'on se pose le problème de savoir à quoi sert le Parlement franchement. Bon alors, après avoir. Sur et Roger Karoutchi sur le fait que nous sommes bien au Sénat et que je préside la séance de l'homme, la parole à Jérôme Durand. Oui, nous allons évidemment monsieur le Président voter l'amendement déposé par notre collègue Claudine pages et j'en profite pour faire une explication de vote sur l'article 7 article aussi je relève avec d'autres mots, avait beaucoup moins de talent les, les, les propos de monsieur Karoutchi nous sommes à peu près à mi-chemin sur l'étude de ce texte et finalement les remarques qu'a formulées tout à l'heure, Claudine pas aimerais révèle bien notre nos difficultés avec cette société de confiance c'est emphatique, société de confiance, alors il y a du réglementaire, il y a du législatif, il y a l'organisationnel Claude ne pas s'interroger sur de nombreuses article 41 qui ont été opposés à des amendements et sur ce texte, voilà, on est toujours entre quelque chose qui s'annonçait très triomphant révolutionnaire et qui est est un petit peu décevant, il faut prendre ce qui a de bon, nous allons le faire et que les numéros des administrations ne soit pas surtaxé c'est une excellente chose, mais pour le reste, on a un petit peu déçu, on va essayer de mettre du rythme, cet après-midi pour qu'il y a de l'enthousiasme, mais malgré tout il faut chercher au fin fond de nos, de nos tripes notre motivation pour soutenir ce travail parlementaire, qui est un peu décevant parfois. Alors, Madame Lepage le gouvernement vous a. Proposé le retrait, vous maintenez l'amendement je mais on voit que faites-vous. que il y avait un article qui parlait de mettre à la disposition du public un numéro d'appel en France je me suis permis de faire la fin de de de l'extension pour les Français de l'étranger, voilà, donc je ne retire pas. S'il n'y a plus d'demande explication de vote, je n'en vois pas donc je mets aux voit cet amendement avec un avis défavorable de la commission également favorable du gouvernement qui vote pour. Celui qui vote contre. Il n'est pas adoptée, nous avons ensuite 2 à commandement faisant l'objet d'une discussion commune le 1er le numéro 48 ou du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, il s'agit simplement levé le gage sur cet article. Et le numéro 70 monsieur du Rhin.

Merci monsieur le président je me permettent de répondre à mon cher collègue, Roger Karoutchi, cet article ne vient pas du Sénat n'est-ce pas donc je voulais le le préciser, je remets les choses à leur place

payer très cher leurs attentes, Telefonica, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à cet article et bien sûr je suis nous sommes favorables aussi à l'amendement qui lève le gaz merci. Alors il me faut demander l'du gouvernement sur l'amendement numéro 70. Monsieur le Président, c'est une demande de retrait de l'amendement Monsieur Durand qui est gage l'Artic sur une augmentation de la taxe transactions financières qui a déjà été augmenté de 50 pourcent dans le PLF l'amendement du gouvernement et avec traditionnel, donc c'est une demande de retrait au profit de l'amendement du gouvernement. Il est retiré, alors il me reste à mettre au voile amendement numéro 48 du gouvernement qui vote pour. Merci qui vote contre.

Oui, Monsieur le ministre, je profite de votre présence dans l'hémicycle pour vous sensibiliser, ou en tous les cas vous alerter, même sur un sujet sur lequel plusieurs dans notre Nous on est et vous interpelle par mon intermédiaire, les expérimentations mises en oeuvre par Les collectivités territoriales en matière de tarification sociale de l'eau, la loi Brottes de d'avril 2013 a permis aux collectivités organisatrices des services d'eau et d'assainissement qui le souhaite en tous les cas d'expérimenter pour une durée de 5 ans, avril 2013, la mise en place d'une tarification sociale de l'eau par le biais, par exemple, de l'attribution d'aides au paiement, pour les petits, facture d'eau pour les personnes en difficulté, vous l'avez compris la fin du quinquennat. Arrivé. Aujourd'hui il n'y a pas de mesures qui sont mises en place, certes le Sénat doit étudier à l'initiative du groupe socialiste et républicain début avril une proposition de loi mais nous connaissons la vocation des propositions de loi, c'est-à-dire que ça peut prendre du temps, or les expérimentations et on est au coeur du sujet servait aussi à des évaluations, donc ma question, elle est finalement à votre endroit, à l'endroit du gouvernement, les doubles quelle est aujourd'hui l'intention du gouvernement par rapport à cette période quinquennale d'expérimentation fera-t-il droit très rapidement après l'examen de la proposition de loi au Sénat pour qu'elle soit également porté à l'Assemblée, ou alors une initiative ou gouvernementale est-elle prévue, vous le savez, c'est important, nous avons eu l'occasion déjà hier d'évoquer dans les débats, l'accessibilité aux services, le respect de la parole de l'État, et là, j'ajoute que ça concerne des Français qui sont parfois éloignés ou anti-cas en difficulté à la fois d'accès et même en l'occurrence sur la tarification sociale de paiement des services de l'eau. monsieur le président, Monsieur le Président, la commission spéciale je je ne reviens pas sur la loi du 15 avril 2013, que vous avez rappelé la possibilité qu'elles ouvrent aux collectivités de mener à bien des expérimentations, il est vrai que, compte tenu du délai nécessaire à la mise en place de cette expérimentation les premiers résultats obtenus par les collectivités sont intéressants mais trop récent pour permettre au niveau national, de déterminer s'il est opportun de généraliser certaines des solutions mises en oeuvre à l'ensemble du territoire, il le comité national de l'eau a émis une recommandation pour prolonger cette expérimentation, une proposition de loi a été déposée devant le Sénat le 7 février dernier par Madame Lubin messieurs qui rouge Caneira ainsi que plusieurs de leurs collègues pour prolonger l'expérimentation de 3 ans, comme l'autorise la loi, elle est inscrite et vous l'avez dit alors du jour de la séance, le 4 avril et le simple fait de déposer cette proposition de loi entraîne automatiquement une prolonge une prolongation d'un an maximum de l'expérimentation, le temps que le texte soit adopté, tels que le précise l'article LO on stresse 6 du code général des collectivités territoriales, en tout état de cause, le gouvernement oeuvrera pour cette proposition de loi soit adopté au plus tôt si votre assemblée l'adoptent, bien évidemment, afin de sécuriser les expérimentations en cours et d'en tirer les meilleurs enseignements avant toute décision, donc le fait que cette proposition soit déposée. Examiné par le Sénat et le cas échéant s'était adopté ouvre une prolongation automatique de un an et permettra l'adoption dans les meilleurs délais de cette proposition de loi qui permet de prolonger l'expérimentation. nous pouvons maintenant en venir à l'examen de l'amendement 147 qui sera défendu par monsieur Bocquet. Oui, monsieur le président Monsieur mini-chers collègues si notre groupe partage évidemment l'objectif de rendre les relations avec les administrations, plus simple, plus fluide, nous ne pensons pas que le référent unique en soi le garant en effet beaucoup de collectivités locales d'administrations ont déjà mis en place des guichets uniques. L'expérimentation qui est ici proposé concerne la mise en place d'un référent unique, je cite le texte à même de faire traiter les demandes qui lui sont adressées pour l'ensemble des services concernés. évidemment plusieurs problèmes nous apparaissent tout d'abord ce référent unique apparaît comme un pis-aller face à la baisse des moyens qui sont alloués depuis quelques années aux administrations qui expliquent grandement les difficultés de nos concitoyens à avoir leur demande traitée avec la plus grande sévérité une baisse des moyens dévolus aux services déconcentrés, qui va de Pair pour le coup avec la complexification de certaines démarches de plus penser qu'un référent unique puisse maîtriser la diversité des métiers des procédures administratives et les qualifications nécessaires pour traiter les demandes nous paraît tout à fait irréaliste le fonctionnaire omniscient, capable de trouver une réponse à la préoccupation des administrés, je ne suis pas certain que cela existe, et l'on peut même se demander si c'est tout à fait souhaitable en se référant deviendrait une sorte de numéros surtaxés d'informations à visage humain en quelque sorte plus concrètement doit encore, on peut raisonnablement penser que la participation des collectivités locales au dispositif ne traduisent une fine et la véritable intention dissimulés, selon nous, d'ailleurs, se référent unique : celle de permettre la poursuite sans difficulté majeure du processus de réduction de la présence territoriale des services de l'État, par transfert de charge en direction des collectivités processus à l'oeuvre depuis de nombreuses années, ainsi donc, si l'on peut dire, l'administration de conseil, de service ne serait plus une administration de guichet négligent de fête son flanc de Sophie comme on parle dans les milieux d'affaires autorisé au profit d'un Back office en lente mais sûre des errances

Lors des auditions que que nous avons menées les différentes parties prenantes ont salué ce dispositif auquel j'adhère également puisqu'il a pour objet la simplification des démarches administratives des usagers, je précise, un autre que l'article 15 n'a pas pour objet de constituer un réseau de maison de service au public, comme il fait référence, l'objet de l'amendement est un que nous avons à une commission spéciale supprimer l'article 15 bis qui prévoyait par ailleurs la mise en place ne référez unique dans les maisons de service au public, il vous est donc proposé un avis défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. monsieur le président, le gouvernement est attaché au dispositif proposé par le présent projet de loi, donc évidemment c'est un avis défavorable à la suppression de l'article que telle que proposée par le groupe. 2 avis défavorables, vous maintenez l'amendement il est maintenu, les demandes d'explications de vote, je n'en vois pas je le mais au voile 147 2 avis défavorables qui vote pour. Merci qui vote contre. Il n'est pas adopté l'amendement 200 rectifier monsieur Gremillet. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, à l'inverse, effectivement, cet amendement n'est pas de supprimer, mais de donner une capacité décisionnelle à l'intérieur, l'interlocuteur unique si on veut être efficace donnions les moyens à cette personne de pouvoir décider de répondre effectivement concrètement du maire efficace aux interlocuteurs et d'ailleurs il y a un avis du Conseil d'État du 23 novembre 2017 qui va dans ce sens, qui préconise notamment de donner un pouvoir de décision à l'interlocuteur référent unique tels que c'est proposé à l'article 15. Merci, quel est l'avis de la commission s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. En fait il il est demandé une demande de retrait, où on a vidé proposer un avis défavorable à cet amendement, présenté comme rédactionnel modifie un fait, le rôle du référent unique l'expérimentation prévoit que le référent unique facilite la vie des usagers un cordon là leur démarche, leur démarche pour une procédure donner et, d'autre part, fruit traiter les demandes par les services concernés, à ce stade, le référent unique n'a pas vocation à traiter lui-même les demandes ni à prendre des décisions et à ce sujet, nous avons été alertés par notamment l'association des élus, et notamment l'Association des maires de France, c'est certain, la conduirait la suppression du verbe faire, proposé par cet amendement, la commission spéciale n'a pas souhaité conférer des pouvoirs de décision référent unique, d'où le demande de retrait sinon un avis défavorable. C'est ma vie, Monsieur le Président, le gouvernement considère plus sage de procéder par étapes, 2 d'abord dans les démarches de facilitation et, le cas échéant si l'expérimentation est concluante, la question pourrait être abordée, mais en en en l'état et à ce stade, c'est un avis défavorable, une demande de retrait. Alors, de demandes de retrait que souhaitez-vous faire cher collègue. On veut gagner, d'efficacité, on veut simplifier on veut rendre effectivement concrets : l'action de ce référent unique et en donne pas la capacité décisionnelle, ça veut dire qu'il y va être l'animateur d'attente de de de réponse des uns et des autres, sincèrement, je pensais qu'on avait bien plus d'ambition dans ce texte de volonté décisionnel, je suis au regret mais je,

Alors l'amendement est retiré, nous allons pouvoir passer au vote sur l'article 15 je vous en prie, chers collègues, vous avez la parole. Explications de vote, nous nous voterons cet article, l'idée est bonne d'un référent unique, on va bien d'où ça vient, ce rapprochement et cette simplification de nos concitoyens au service, mais les questions qui sont posées sont des vrais Christian avec quels moyens quelles formations, quels profils de se référant formation initiale mais aussi formation continue pour être efficace, donc nous voterons mais nous demandons aussi d'avoir les preuves de l'exercice de la mise en place de ce référent unique. Merci à d'autres demandes d'explications de vote, je n'en vois pas mais au moins, l'article 15 qui vote pour. Qui vote contre qui s'abstient être. Adopté l'article 15 bis et supprimer l'article 15 ter, dans le cadre de la législation en commission et réservé. Après l'article 15 je suis l'amendement 211 rectifier du gouvernement Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, il s'agit par cet amendement d'instituer un dispositif d'indicateurs de qualité et de résultats, mesurant la satisfaction des usagers, ce dispositif devrait être mis en oeuvre par les administrations en contact avec le public et les indicateurs feront l'objet d'une publication, l'objectif de cette disposition et d'assurer l'information à destination d'une part des administrations qui pourront ainsi prendre conscience des progrès effectués et, d'autre part des usagers, qui seront renseignés sur les performances de l'administration avec laquelle ils sont en contact, cet amendement traduit ainsi au travers dispositions contraignantes l'objectif qu'il vous a été proposé d'insérer dans la stratégie nationale dans inondations pour l'action publique, à savoir l'accès pour toute personne une information transparente sur l'efficacité et la qualité des services publics en relation avec les usagers. Merci, monsieur le rapporteur, quel élu de la commission, pardon madame. Un duo que Un duo que je fasse attention. Facile à présent amendements ont été déposés tardivement, monsieur le ministre et donc prévoit dans la loi la publication d'indicateurs de résultats et du qualité de service des administrations de l'État recevant du public, public, je ne peut être que favorable à cette démarche : pourquoi la tente de l'inscrire dans la loi pour le faire, nul besoin d'une disposition législative me semble pour mettre en 9 ce type de dispositif qui existe déjà dans certains plus de service public et même parmi ceux des collectivités territoriales et en août, le second paragraphe de votre amendement renvoie l'entrée en vigueur de la disposition à une date inconnue fixé par décret et au plus tard au 31 décembre 2020, ce qui a plutôt tendance à tempérer l'urgence d'introduire cette disposition dans la loi alors c'est plutôt un avis défavorable, il n'y suis désolé ça je je reviens à ce que j'ai dit hier à ma collègue. Alors, explication de vote Monsieur Bocquet la parole. Oui, très brièvement, nous allons bien sûr voter contre cet article non pas par dogmatisme et parce que il nous pose de vraies questions, d'abord sur l'évaluation, à ma connaissance, il y a déjà la LOLF qui permet certaines pratiques d'évaluation, deuxièmement, quels seront les critères d'évaluation de l'efficience de l'administration et j'ai l'impression que de plus en plus, on va faire beaucoup d'administrations et de statistiques, au lieu de s'occuper des gens. Halem polluantes. Oui, c'est toute la dimension finalement qui renvoie à ce qu'on appelle la quand ouf on est tout le temps en train de quantifier, c'est de transformer des réalités et de les faire rentrer à toute force dans les tableaux Excel. Bon, évidemment, c'est bien de mesurer la satisfaction est souvent, on s'en arrête là et puis on s'en arrête à avoir plus 1 plus 2 pourcent se regarder d'où on part et on dirait que ça va mieux, donc je crois qu'on rentre effectivement dans une dans une sphère où l'administration génère beaucoup d'chiffres. Ils sont pas forcément toujours très analyser ni regarder bon n'est pas contre évaluer, bien entendu, mais encore faut-il avoir les garanties que ces évaluations soient vraiment de nature à avoir aussi une évaluation qualitative des services publics et puis que n'en reste pas uniquement remplir ses tableaux sans qu'il soit jamais lu. Pas d'autres demandes d'explications de vote, donc je vous rappelle que nous sommes sur le 211 rectifier avec un avis défavorable de la commission du métro et cet amendement du gouvernement qui vote pour.

Merci monsieur le président, moi je juste que c'est important que le Sénat débattent de sujets de vie quotidienne, ça me choque pas qu'on parle de droit au contrôle de droit à l'erreur de numéros surtaxés de référent unique voilà ce concerne quand même la vie des citoyens et des entreprises, l'article 16 ans, mais aussi une bonne illustration puisque c'est d'expérimentation, l'expérimentation pour une la limitation de la durée des contrats sera-t-il pour les PME dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée cumulée des contrôles réalisés sur un même établissement au sein d'une petite ou moyenne entreprise sera limitée à 9 mois sur une période consécutifs de 3 ans, ce sont près d'un 1000000 de de PME qui sont concernés par l'expérimentation l'objectif avec cette mesure et de passer du contrôle sanction à un contrôle plutôt de type conseil dans le cas d'une politique partenariale avec les entreprises désireuses de se conformer à leurs obligations, elle permet aussi de diminuer les charges liées au contrôle, il faut avoir en tête quand même parfois la succession que représentent les contrôles, Urssaf, répression des fraudes, contrôle de Hama salariale et puis aussi la succession de la matière vérifier il y a un chiffre d'affaires, les conditions de travail des équipements techniques etc donc tout ça est consommateur de temps notamment pour pour les dirigeants qui sont parfois qu'confronté à la complexité du droit à l'incertitude que prend le compte que prendra durée du contrôle et puis aussi les contrôles qui sont effectués par intermittence, sans qu'on sache quand est-ce qui commence, quant à ceux qui finissent là aussi, c'est le même principe que pour droit l'horaire, c'est ce qui compte, c'est la bonne foi, l'idée c'est bien de d'inciter, de conseiller des entreprises qui veulent se conformer à leurs obligations et donc en les accompagnant l'article a d'ailleurs été je crois largement améliorée, notamment par Stanislas Guérini à l'Assemblée nationale, voilà pour notamment préciser un certain nombre de un certain nombre de points qui était une demande forte des des entreprises, voilà un article qui me paraît utile et il me paraît utile que nous en débattions. Alors nous avons maintenant l'examen l'amendement 148. Monsieur Bocquet non je vous en prie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc nous proposons et nous souhaitons supprimer cet article, outre que cela limite le droit au contrôle la fixation est assez formelle puisque, dans la pratique, et pour donner un exemple précis, l'objectif de l'inspecteur vérificateur de la DGF Ipsos situe à une procédure achevée par mois cette segmentation du contrôle fiscal consacré par l'article la DGE se préoccupant des dossiers, des entreprises et groupes ayant plus de de 250 millions de chiffre d'affaires et s'acquittant de plus ou moins 50 pourcent de l'cet article donc nuit à Sun efficacité les groupes qui constitue en effet le portefeuille d'entreprises contrôlables par les services de la DGE dispose aussi d'une forme de réseau de filiales et sous-filiales, dont les services déconcentrés peuvent avoir une connaissance plus fine complémentaire de ce que peut faire la direction spécialisée pour le reste, monsieur Mini ce contenu de ce que j'ai de ces exceptions c'est article est bel et bien un article d'affichage, c'est la raison pour laquelle nous demandons sa suppression. quel est l'avis de la Commission, que notre commission a au contraire souhaité renforcer et ceci en modulant à la baisse cette durée pour les très petites entreprises, j'avoue par ailleurs avoir de du mal à suivre l'argumentation des auteurs qui semble nous expliquer à la fois que ce plafonnement entraverait et la capacité de contrôle de l'administration et qui ne sert à rien, ou presque, en raison de ses trop nombreuses exceptions, en fait, je rappelle que nous sommes visés ici que les PME et que le plafond envisagée aura surtout pour effet d'obliger les administrations à coordonner leur programme de contrôles pour éviter de concentrer la charge sur les même entreprise, donc c'est un avis défavorable. Moi je lui l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, là, l'avis est défavorable de la même manière, puisque le gouvernement avait introduit dans le texte initial des dispositions visant à limiter la durée de contrôle sur 3 ans, le gouvernement ne partage pas tout à fait la la rédaction issu de la commission spéciale et j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, mais en tout cas, défavorables à la suppression de l'article. 2 avis défavorables et demandes d'explications de vote, je n'en vois pas je mais on voit cet amendement 248 qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée, nous avons ensuite 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune, on commence par le numéro 49 du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, je disais à l'instant que le gouvernement ne partageait pas totalement la rédaction issue des travaux de la commission spéciale qui vise à réduire à 6 mois le délai cumulé de contrôle pour les entreprises de moins de salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros, nous ne sommes pas fait pas favorable à cette distinction opérée qui crée de régime juridique au sein de la même expérimentation et selon la taille des entreprises une telle distinction rend plus complexe la mise en oeuvre par les administrations concernées de cette mesure expérimentale et nous considérons que la limitation à 9 mois la durée cumulée est déjà une avancée importante, donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons par cet amendement, revenir à une lecture unique, quelle que soit la taille des entreprises dans le plafond des 250 salariés des PME. Merci, nous avons l'amendement 180 rectifier Madame Delattre qui le présente. Oui, merci Monsieur le Président, mais écoutez monsieur ministre nous nous allons même au-delà ou en-deçà des 9 mois c'est vrai que cet article 16 instaure à titre expérimental une limitation de la durée des contrôles administratifs sur les PME Il était temps, mais pour nous la durée retenue, fixé à 9 mois nous paraît encore excessive puisque cela revient à 3 mois de contrôle, en moyenne, soit le quart du temps passé en contrôle dans une entreprise sur une année et c'est pour ça que nous proposons de ramener la durée du contrôle à 6 mois sur 3 ans pour les entreprises de moins de 150 camps de salariés, moins de 50 millions d'euros. oui tout à fait puisque si celui-ci n'ait pas retenu ici le sens 80 n'est pas retenu pour les petites entreprises de moins 10 salariés nous préconisons de passer de 6 à 4 mois de de contrôle parce que là aussi beaucoup de temps, de mobiliser pour des petites entreprises qui ont autre chose à faire, et très peu de pièces en fait a montré à l'administration. Merci, nous allons maintenant entendent l'avis de la Commission sur ces 3 amendements. Alors merci Monsieur le Président, d'abord sur le l'amendement déposé par le gouvernement. Cet amendement entend revenir sur la modulation du plafond, le monde introduite par par votre commission sur la taille de l'entreprise, soit je rappelle le 9 mois sur la période de 3 ans pour les PME et 6 mois sur la même période, pour les très petites entreprises, très petites entreprises, moins de 10 salariés, chiffre d'affaires annuel inférieur, rappelons-le, à 2 millions d'euros, or aucun des arguments présentés par le gouvernement à l'appui, donne-t-elle amendements ne me semble recevable à en termes de complexité, d'abord, les administrations sont tout à fait capable comme elles le font déjà dans le cadre de nombreux dispositifs de gérer 2 plafonds différents selon la taille de l'entreprise, qui plus est, dans le cadre du président dispositif dans la complexité tiendra bien plus aux enjeux de coordination entre administrations ou au mode de calcul de la durée des contrôles qu'à la gestion de 2 plafonds, en en fait, le gouvernement avance ensuite que la limitation à 9 mois aurait, je cite l'assentiment des entreprises, or ce n'est pas du tout ce que nous ont dit leur représentant, que nous avons auditionnés et qui revendiquait même d'aller bien plus loin que les 6 mois que nous proposons pour les TPE, dernier point renvoyé au bilan de l'expérimentation pour affiner le cas échéant, cette durée selon la taille des entreprises est une réponse très zen, ça satisfaisante car l'homme pourrait alors objecté qu'on ne peut généraliser une mesure qui n'a pas été testés, or l'expérimentation a précisément pour but de tester le plafonnement dans plusieurs configurations avant sa généralisation éventuelle tester de plafonds différents permettra dès lors d'un Tir tous les hein saignement j'ajoute que le gouvernement ne peut pas nous expliquer, je suis désolé, monsieur le ministre, ne pas nous expliquer en même temps que l'administration doit s'adapter à son public et revendiqué de traiter une entreprise de 5 salariés comme un groupe de 200 collaborateurs. Donc, il vous est proposé sur cet amendement déposé par le gouvernement, donc je disais un avis défavorable sur les 2 autres amendements. Proposé par nos collègues. Ceux-ci vise en effet à réduire de 9 à 6 mois la durée cumulée des contrôles administratifs pour les PME de 10 salariés plus concernés par l'expérimentation et de 6 à 4 mois pour les TPE de moins de 10 salariés, je rappelle que cette modulation, a été ajouté par notre commission quant aux de délai à retenir, c'est certainement un éternel débat, mais il me semble que la position de Nantes commission est assez équilibré, elles tiennent compte à la fois de la charge plus importante que ces contrôles peuvent représenter pour le TPE et à la fois de la nécessité de maintenir une certaine capacité de contrôle de l'administration, j'ajoute que, comme vous l'avez constaté lors de l'examen de l'amendement 49, le gouvernement n'est déjà opposé à une limitation à 6 mois pour les soldes TPE et je le ferais, je le serai donc, a fortiori si nous abaisser encore les plafonds à 6 et 4 mois essayons déjà de préserver les acquis du texte, la commission dans la perspective des discussions à venir avec nos collègues députés, là aussi, il est demandé une demande de retrait ou un avis défavorable, voilà Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, les le gouvernement sur les 180 182 rectifier. Merci Monsieur le Président, en cohérence avec l'amendement que j'ai défendu au nom du gouvernement, la vie ne peut être que défavorable sur les 2 amendements proposés par Madame De Lattre, pour ce qui concerne l'amendement du gouvernement, je vais, je répète : nous sommes dans une phase d'expérimentation sur des territoires qui sont ciblées sur les entreprises qui relèvent de la catégorie des PME, nous sommes convaincus que cette expérimentation nécessite de la lisibilité et que nous aurions plus de complexité à introduire des seuils de différenciation au sein d'une même expérimentation s', raison pour laquelle le gouvernement maintient son amendement, considérant qu'il sera plus utile d'avoir une expérimentation qui porte sur l'ensemble des entreprises de moins de 150 salariés avec les mêmes critères. Merci, alors je mettre voilà Mandement numéro 49 pas de demandes d'explications de vote, je n'en vois pas, je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, qui vote pour. Eh bien écoutez, qui vote contre. Il n'est pas adoptée, sur les 180 rectifier 182 rectifier : demande de retrait de la commission défavorable du gouvernement, vous maintenez, cher collègue, ils sont maintenus, le sang 80 rectifier qui vote pour. Qui vote contre. Il n'est pas adopté même votent pour le 182 rectifier j'imagine même vote nous en venons à l'amendement numéro 168 qui est présentée par. Merci, monsieur Merci, monsieur le Ministre Mesdames, messieurs, mes chers collègues. L'article 16 propose tisser expérimentale de limiter la durée des contrôles pour les PME, la commission spéciale du Sénat propose à juste titre de moduler cette limitation de durée à la taille de l'entreprise, soit 9 mois pour les PME, soit 3 mois pour les TPE, article 16 prévoit toutefois que cette limitation de durée n'est pas opposable lorsqu'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire, or l'objet de contrôles, précisément, de repérer les éventuels manquements aux obligations en vigueur, il importe donc que la limitation de sa durée reste opposable, même quand les indices laissent supposer de tels manquements, l'amendement vise donc à prévoir que la durée de tout contrôle soit effectivement limité pour les PME, cela incitera l'administration de contrôle à cibler ces derniers en mettant fin, d'une part l'intermittence de la présence des contrôleurs, d'autre part à l'ignorance de ce qu'ils cherchent justement dénoncées dans le rapport de l'Assemblée nationale numéro 575 du 18 janvier 2018 afin de préserver la bonne marche des entreprises, il n'est plus acceptable de rencontrer des situations assez décrites pour le Fisc et les Urssaf, notamment les contrôles revienne un jour par semaine et vont revenir après un 1er passage un mois plutôt rare pour une séance de 2 heures et on et sont susceptibles de se manifester périodiquement quelques jours de nouveau ces séances intermittente dans les entreprises ne connaissent pas la faire apparaître du fait de leur rythme décousu perturbant notamment pour les PME, merci. Cet amendement vise à supprimer l'exception plafonnement de la durée des contrôles académie ce précis et concordants de Man comment a une obligation légale au réglementaire si je peux souscrire à certaines considérations exprimée dans son objet, mais qui n'ont pas de lien avec son dispositif en particulier lorsqu'il est question de la difficulté pour les entreprises à gérer les contrôle, contrôle perlé, avec une présence très intermittente des contrôleurs sur site, je ne peut en revanche être d'accord avec le fait, je cite, qu'il importe que la limitation de durée reste opposables même comme des indices laissent supposer des dément en supprimant cette exception l'administration pourrait ne plus être mesure de contrôler l'entreprise, alors même qu'elle disposait d'indices précis et concordants et là, les termes sont sont importants, qu'il ne s'agit pas d'une simple présomption et ce par le simple effet de plafond Le Mans arithmétique de la durée des contrôles, je rappelle que la mesure expérimentée ici ne vise pas à faciliter la vie des fraudeurs, parce que vous partagez tous mais seulement à alléger la charge des contrôles pour les entreprises que je qualifierais de bonne foi, c'est donc lundi défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur le Président pour exactement les mêmes raisons que celles exprimées par le rapporteur, c'est un avis tout aussi défavorable. Alors 2 avis défavorables des demandes d'explications de vote je n'envoie. Il est maintenu, Jacques collègues demande explication de vote si je vous en prie, monsieur je ne souscris pas donc aux conclusions de de notre collègue, mais je voudrais quand même faire observer qu'il s'agit d'un article. Parmi d'autres, parfaitement contradictoires. Il y a d'un côté, on affiche de la mansuétude de l'attention du Caire comme on dit maintenant vis-à-vis des entreprises. Et puis d'un autre bah, évidemment, il y a six, il a vraiment un vrai problème, ben on a toujours la possibilité de surseoir à ce que prévoit la loi, si on regarde les choses un petit peu en détail, c'est pas le seul article qui est fabriqué comme ça une chose et son contraire : c'est là, c'est là où le gouvernement au Centre.

qui vote pour. Il n'est pas adoptée nous en venons à l'examen de l'amendement numéro 149 Monsieur Bockel présente. Oui, amendement 149 qui est un moment de de cohérence, donc très brièvement, amendement qui reprend la position de fond que nous avons exprimée dès l'examen de l'article 2 qui consiste à faire en sorte que les entreprises qui ne respecteraient pas les règles les plus élémentaires du code du travail soit placé hors Champ de l'application des présumés nouveau droit ouvert par cet article 16 merci. Monsieur le Président, cet amendement vise ajouter la liste des exceptions au plafonnement de la durée, les contrôles expérimentée par le présent article des contrôles destinés à s'assurer de respect des normes internationales et des dispositions d'or de public du droit du travail, il était en réalité pleines mains satisfait par le droit existant et par la hiérarchie des normes que cela a déjà pu être Rassam rappeler lors des débats à l'Assemblée nationale, le droit international, un effet sur le droit national 5 qu'il soit nécessaire de l'expliciter, et il en va de même pour les dispositions législatives d'ordre public, auquel il ne peut être dérogé à l'espèce d'inspection du travail est visé par les conventions liées à la France à l'Organisation internationale du travail qui prévoient le sur le droit national 5 qu'il soit nécessaire de le rappeler, c'est du reste pour la même raison que nous avons supprimé à l'article de et par cohérence, une référence, il est inutile au respect des conventions internationales et s'il était nécessaire et pour vous rassurer définitivement, je vous renvoie aux propos tenus par le secrétaire d'État en séance à l'Assemblée, qui indiquait, je cite, que les contrôles effectués par l'inspection du travail occupe une place particulière et central, et que c'est au tour 2 que devront s'articuler un certain nombre d'autres contrôles, ajoutant qu'il veillerait, monsieur le ministre, à ce que les textes d'application tiennent compte de cette particularité donc il vous est proposé un avis défavorable. monsieur le président, monsieur le rapporteur a tout dit, comme en plus il y a des situations particulièrement pertinente, ça ne peut être qu'un avis identique donc défavorable. 2 avis défavorables, chers collègues, vous maintenez amendement il est maintenu, je vais le mettre aux voix pas demande explication de vote qui vote pour. Merci qui vote contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, j'ai maintenant mettre au voilà le 16 pas de demandes d'explications de vote jamais on voit l'article 16 qui vote pour.

Oui merci monsieur le président, Monsieur le ministre, chers collègues, lors de la discussion générale, j'ai eu l'occasion de rappeler le souci qui est le mien et celui du groupe des indépendants d'alléger les contraintes qui pèsent sur les PME. Il n'est pas normal que les. Contraintes juridiques, techniques soient les mêmes pour des grands groupes internationaux des grands groupes, même français, que ce soit les mêmes qui pèsent sur des PME. Alors que les moyens ne sont pas les mêmes et les moyens humains, les moyens juridiques. Il faut donc tout faire pour faciliter la vie des PME, ce sont ces PME qui permettent, par leur dynamisme aux Allemands de connaître un commerce extérieur particulièrement bénéficiaire, c'est le manque de dynamisme, notamment de ces PME qui permet en France qui contraint en France notre économie à connaître un déficit de son commerce extérieur à 62 milliards de. L'amendement qui vous est proposé est tout à fait modeste, il vise dans ce sens, a limité les contrôles sur les entreprises de moins de 20 salariés, c'est-à-dire sur les PME, à la même durée que celle des entreprises de moins de 10 salariés, c'est-à-dire la période de 3 mois et c'est tout à fait modeste mais ça va de fait dans le sens et dans la logique le limiter les contraintes qui pèsent sur les entreprises de 20 salariés sur leur site.

Merci monsieur le président. bien entendu, nous sommes très favorables à tout ce qui peut alléger en fait l'administration dans les entreprises, toutefois, monsieur Capu et les auteurs de l'amendement numéro 26 propose d'inscrire directement cette limitation dans le code de la Sécurité sociale, alors que le gouvernement propose de recourir à l'expérimentation, je précise que le Sénat déjà d'adopter un amendement similaire, avec un seuil fixé à 50 salariés dans le cadre du dernier Plfss le recours à l'expérimente plantations se justifie lorsqu'on ne connaît pas par avance les effets d'une mesure ici il me semble que les enjeux sont assez claires et on voit mal ce qu'une expérimentation pour prouver la commission spéciale a donc donné un avis favorable à l'amendement numéro 26 de monsieur dont l'adoption fera logiquement tomber celui du gouvernement. Alors

de 10 ou moins 20 salariés si c'était adopté soit aussi expérimental sur la même durée de manière le plus cohérent possible, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé, j'ai demandé à monsieur qui a pu le retrait de son amendement au profit de celui du gouvernement et donc contre la ville, a commis. Alors, nous sommes sur le 26 rectifier bis tout d'abord pas de demandes d'explications de vote, je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable, que le gouvernement proposait le retrait qui votent pour cet amendement. amendement. Merci qui vote contre. Il est donc adopté est celui du gouvernement tombe, les articles 17 17 bis a 17 bis Besson réservés pour les mêmes raisons que la fois précédente. L'article 17 Glisser supprimé après l'article 17 bis nous en venons à l'examen de l'amendement 27 rectifier, monsieur Capu. on est dans la même logique d'alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises, il s'agit cette fois-ci de l'examen des des examens de comptabilité qui sont prévues, vous savez que, on doit l'entreprise doit adresser ses pièces justificatives dans un délai de 15 jours. Il me semble, il semble à mon groupe que ce délai de 15 jours pour adresser les pièces justificatives à l'administration fiscale qui contrôle de chez elle, sur la comptabilité uniquement la les pièces phares de la comptabilité de l'entreprise est un peu court. Notamment en période de congés, l'amendement est très modeste, il propose juste si l'administration on est favorable, on est d'accord, en cas de demande de l'usager, de renouveler une fois ce délai de 15 jours. Donc, il s'est ainsi rédiger éventuellement renouvelés, une fois pour la durée pour la même durée, sur demande du contribuable, voyez donc on facilite la vie des entreprises et c'est avec l'accord de l'administration, voilà le sens de cet amendement. Merci, cher collègue, l'avis de la commission s'il vous plaît. Madame la important. depuis les bureaux du service des impôts les fichiers des écritures comptables appelé fait que dans une entreprise, alors c'est vrai que le délai de 15 jours donné à l'entreprise pour transmettre une une copie des faits que peut notamment période de congés, difficile à tenir, toutefois, en pratique, l'administration tient naturellement compte de ces contraintes et fait preuve de souplesse comme le ministre pourra sans doute nous le confirmer, et nous sommes dans un texte sur la confiance je peux vous le dire, d'expérience personnelle et à chaque fois que j'ai eu, a demandé un délai à l'administration fiscale a toutefois été accordé et notamment quand on est en période de congés, donc il ne se même me semble pas opportun de prévoir dans la loi une possibilité de porter ce délai à 30 jours et c'est pour laquelle c'est plutôt une demande de retrait ou un avis défavorable. confirmer les propos de Madame le rapporteur, mais les demandes de délits sont toujours accordé pour tous les motifs légitimes et notamment ceux liés aux congés maladie inscrire dans la loi la possibilité automatique de proroger jusqu'à rendent jours aurait pour effet de systématiser la possibilité de retarder les procédures de contrôle, donc c'est aussi une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Alors, chers collègues de demandes de retrait. le renouvellement, il visait, avec l'accord, en fait, qui visait à alléger léger à légiférer à rendre à m'écrire dans le texte, ce qui se pratique aujourd'hui, d'après ce qu'on dit, donc je vois pas très bien en quoi une demande de retrait se justifiait maintenant si la Commission maintient sa demande de retrait, vous avez compris qu'on est vraiment en fait il s'agit juste d'écrire dans le texte, ce qui se pratique aujourd'hui, c'est-à-dire leur l'usage demande un nouveau délai et l'administration n'est pas obligé de l'accorder, c'est juste une demande voilà donc si vous demandez si vous maintenez votre demande de retrait je par courtoisie et par délicatesse, je retire à l'abonnement. bien écoutez, il est retiré. Après l'article 17 bis nous en venons à l'examen de l'amendement 203 rectifier monsieur à la parole. mais monsieur le président, Monsieur le ministre. Madame, monsieur, rapporteur, chers collègues, c'est un amendement de bon sens qu'il y a effectivement pour but de prendre en considération l'entreprise qui ne fraudent pas avoir du retard et cet amendement propose tout simplement que, dans le délai d'un mois sur la non fourniture la Direct du formulaire sur le redressement malgré tout, que ces 30 entreprises dès lors que c'est dans le délai du mois et qu'a pas fraude puisse bénéficier de l'exonération des cotisations suffisent par rapport à cette, à cette qui est trop souvent d'ailleurs, il faut rappeler que c'est un document très lourd administrativement, c'est par un simple formulaire et ayons cette capacité dans cette société confiance de tolérance vis-à-vis des entreprises. Quel est l'avis de la commission même l'emporte. Merci monsieur le président. les entreprises qui ont conclu un accord d'intéressement peuvent bénéficier d'exonérations sociales, il faut pour cela que l'accord ait été conclu avant le 1er juillet ou le 1er avril suivant la période d'imposition applicable et être transmis à la Direct dans les 15 jours suivant cette date limite ce délai s'explique en partie par le fait que la direc dispose ensuite d'un délai de 4 mois pour effectuer un contrôle de légalité de l'accord qui lui transmit lorsque l'accord est transmis tardivement les exonérations ne s'applique que pour l'avenir, l'amendement proposé introduit de la complexité des dispositions qui ne sont déjà pas d'une clarté absolue maintient en effet le principe selon lequel l'accord doit être transmis à la direction qu'un jour, mais permet un retard d'un mois dans les faits, cela conduit à décaler d'un mois la date butoir, par ailleurs, dans la mesure où la direc dispose toujours d'un délai de 4 mois pour contrôler la légalité de l'accord et demander, le cas échéant des modifications, le délai pour effectuer ces modifications avant le début de la nouvelle année calendaire serait fortement restreint donc la commission a émis un avis défavorable à moins que l'amendement soit retiré par son auteur. Monsieur le Président, là aussi, le gouvernement partage, mot pour mot l'avis formulé par le rapporteur de la commission spéciale, donc c'est un avis défavorable ou une demande de retrait. Le monde de retrait Notre collègue du plomb, a demandé la parole en explications de vote. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, le délai d'un mois. Pour déposer, alors que l'administration en A4 pour traiter le dossier me paraît pas juste. c'est pas équilibré dans une société de confiance, comment vous pouvez expliquer à quelqu'un qu'il y a un mois, alors que même ses 15 jours donc voulu donner 15 jours de plus qu'un boulet, c'est 4 mois l'administration pour traiter son problème, c'est de la confiance particulière ou du moins de la confiance aveugle géométrie variable selon qu'il a traité de la confiance, donc je voterai cet amendement. à mon à mon collègue donc ça sous-entend que l'entreprise, en fait, elle démarre son examen finalement dernière minute et donc il lui faut un peu plus de 15 jours pour regagner préparer son dossier et un mois non, elle a du temps, donc les 4 mois les 4 mois pour l'administration sont tout à fait normaux en fait pour l'étude parce que l'entreprise à la vue du temps pour pour écrire son son son accord donc il faut lui laisser aussi ce ce délai et sincèrement, de toute façon, ajouter 15 jours ça ne va rien, rien du tout, apporter à l'entreprise, c'est pas pareil que si on lui donner 3 mois donc, sincèrement c'est un avis défavorable, ça donne encore plus de complexité sincèrement. Alors, nous avions une demande de retrait monsieur Gremillet nous dire ce qu'il en pense. Monsieur le président Monsieur mission et chers collègues non je je vais pas le retirer, pour la simple raison qu'effectivement je reprends le propos de mon collègue. c'est pas vraiment équilibré. Encore une fois n'est pas devant une entreprise qui vont les termes en trichant, on est sur un document administratif, qui doit être déposé et c'est une tolérance de 15 jours supplémentaires pour lui permettent. Madame la rapporteure pour lui permettent de continuer de bénéficier d'exonérations, donc c'est pas l'enjeu pour l'entreprise, il est énorme, c'est la tolérance effectivement qu'un document entre guillemets administratifs envoyés puissent arriver effectivement qu'un jour, quand on voit les conséquences que ça, on n'est pas sur un laps de temps, de 4 mois, on est sûr qu'un jour supplémentaire, encore une fois, on dit qu'on parle de du droit à l'erreur et qu'on reconnaît aux entreprises de cette capacité, effectivement, d'avoir cédé mêmes sujets qu'on avait hier sur d'autres dossiers, effectivement vous avez 8 jours de retard. Et pour autant on va pénaliser complètement cette entreprise parce que vous avez eu un jour de retard alors qu'on parle de droit à l'erreur, on est vraiment dans le dans le sens profond de de ce texte alors je comprends pas, et je me trompe de débat, mais je pense pas. Voilà, je pense que je vais pouvoir mettre aux voix, maintenant j'ai bien compris, chers collègues, je vais donc le mettre aux voix, en rappelant que nous avons un avis défavorable de la commission demande de retrait ou défavorables du gouvernement qui vote pour.

qui vote contre Il était adopté. à l'article 18, nous allons à l'examen de l'amendement numéro 150 présenté par Monsieur Bocquet. Oui, donc je vous renvoie bien sûr à l'objet présenté dans le corps de l'amendement, si nous en restons à la seule question des indus ce point que je voudrais aborder, je constate que l'article ne contient aucune mesure relative sur l'accès aux droits de l'ensemble des personnes ne faisant pas jouer précisément leurs droits à la location, pourquoi dans ce cas ne pas avoir procédé à la réécriture de l'article L. 553 tiré 2 du code de la Sécurité sociale, du code qui précise qui signifie clairement qu'existe déjà un dispositif de droit à l'erreur en matière de prestations sociales dont il suffirait peut-être de préciser les contours, un droit à l'erreur dont il nous semble qu'il ne peut se limiter aux questions de la récupération des indus mais doit aussi, selon nous, porter sur la question de l'ouverture des droits pour ceux qui en sont aujourd'hui privés, il s'agit là d'un manque important de ce texte, nous ne pouvons que souligner encore une fois la situation en regrettant que le choc de simplification administrative n'est pas encore touché les formulaires à remplir pour l'allocation logement, par exemple, ou encore le Revenu de Solidarité Active merci.

je partage une partie des observations des auteurs de l'amendement, en effet, il eut été préférable que le gouvernement ne présente un projet de réforme aboutit plutôt que de nous demander une habilitation. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion de dénoncer le nombre d'habilitation que contient ce texte et la commission spéciale en a supprimé certaines pour autant il me semble souhaitable de créer au bénéfice des allocataires un droit à la rectification des informations qui les concernent, lorsque celles-ci ont un impact sur le montant d'un indu dont on leur demande le remboursement, compte tenu des différences entre les règles qui régissent aujourd'hui le recouvrement des indus fonction des organismes concernés, la commission spéciale a souhaité accepter le recours à la méthode des ordonnances, tout en réduisant la durée de l'habilitation qui lui semblait excessive donc la commission est spécial, a donné un avis défavorable à cet amendement de suppression. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, juste un point de précision pour les auteurs de l'amendement, puisque vous dites, mesdames et messieurs que les dispositions à prendre ne relève de relève de la elle FSS alors que, selon nous, ne relève pas de la FSS mais au-delà de ça, le recours à l'ordonnance et le délai de l'habilitation donnée au gouvernement se justifient, selon nous, par le temps nécessaire pour définir manière concertée des dispositions harmoniser sur un Champ très large de prestations et nous précisons que l'ordonnance sera élaboré sur la base d'un bilan précis des pratiques encore à réaliser le bilan, en l'occurrence l'objectif d'amélioration du respect des droits des allocataires lorsqu'il conteste l'exactitude du montant notifier devra se concilier avec la prise en compte des contraintes de gestion et des enjeux financiers de la Sécurité sociale, notamment la branche famille en matière de recouvrement financier des indus et l'ordonnance tout permet d'acter le principe, elle prend le temps de cette concertation, donc c'est un avis défavorable à votre. Alors 2 avis défavorables monsieur Colombain en explications de vote. Je voudrais faire observer que. Je n'imagine pas que l'administration telle qu'elle fonctionne actuellement refuse. des justifications donc concerner une situation, par contre, je trouve que ce texte manque enfin passe à côté, où on ne parle pas d'un problème qui semble quand même devenu essentiel c'est le mode de récupération des indus, c'est-à-dire qu'il y a, lorsque vous avez déjà lu qui court sur des sur des périodes extrêmement longue, quand on n'a pas beaucoup de moyens en fait pas forcément attention à ce au fait qu'on a trop perçu

d'après ce qu'on entend ici ou là et quand même un problème qui se pose, largement aujourd'hui. Pas d'autres demandes je n'en vois pas je me voix l'amendement numéro 150 avec 2 avis défavorables qui vote pour.

Vous aviez demandé la parole, je vous en prie, chers collègues. Merci Monsieur le Président, une explication de vote, c'est un vrai problème, cette question de récupération de recouvrement des indus et la manière que nous présente gouvernement aujourd'hui par cette habilitation à légiférer par ordonnances ne nous convient pas, mais pour parler du fond, on pense que vraiment il faut continuer sur cette sécurisation de donner aux personnes qui sont concernées et souvent ce sont des bénéficiaires du RSA, nous avons été auditionné avec Madame Bruni, la Caisse nationale d'allocations familiales, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps pour les administrations, mais c'est surtout des situations dramatiques qui sont vécues par les bénéficiaires,

Qui vote pour l'article 18 merci. Qui vote contre. Abstention : il est adopté à l'article 19 nous avons 2 amendements identiques en discussion commune 151 Monsieur Guey, je vous en prie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article propose 2 types d'expérimentation, renforcer la mission de conseil et d'assistance auprès des espoirs tant agricole et régionaliser le réseau des chambres d'agriculture, si l'on peut adhérer à l'objectif de renforcer la mission de conseil la régionalisation, quant à elle nous pose question voir problème. Première question, monsieur le ministre, l'intégration des chambres départementales sera-t-elle volontaire ou forcé. Et que comme penser en termes d'aménagement du territoire, cela ne risque-t-il pas d'éloigner encore un peu plus les administrés de ces chambres si ces dernières n'ont plus qu'une antenne régionale dans des des Jeux, région déjà remanié qui sont maintenant gigantesques le transfert, même au optionnel des compétences et est tout à fait discutable dans les nouvelles régions les relais chambre régionale d'agriculture sont dominés par les anciennes régions les plus importantes en termes de population de superficie ou de richesse et le caractère optionnel n'évitera pas la pompe aspirante, aujourd'hui nous avons au contraire besoin de chambre d'agriculture de proximité pour développer de nouvelles pratiques agricoles, la priorité doit être donnée à l'animation de proximité plus qu'à des mécanismes financiers en tous les cas sur un sujet aussi sensible, il n'est pas concevable de passer par une législation pas ordonnance la réforme des chambres d'agriculture, Merritt, nous le pensons, un débat parlementaire, on ne saurait laisser le gouvernement gouvernement agir sans qu'aucune concertation n'ait lieu, d'autant plus comme projet de loi concernant l'agriculture devrait arriver au printemps, ne serait-il pas plus judicieux d'attendre ce entrent véhicule législatif plus cohérent pour traiter ce sujet, c'est pourquoi nous demandons donc la suppression de cet article. Alors selon second amendement de suppression madame Delattre. Oui, merci Monsieur le Président, effectivement cet article entend réformer par voie d'ordonnance, le réseau des chambres d'agriculture, si des précisions positive positive apportées en commission spéciale sur l'accord préalable des chambres départementales pour l'exercice 2 missions au niveau régional, je suis convaincu que le véhicule utilisé, eu égard à la sensibilité du sujet me pose question pose question véritable cavalier législatif, cette disposition ambitionne de régler cette question au coeur des préoccupations des agriculteurs au détour d'un article dans un projet de loi sans véritable lien avec ce sujet afin de préserver la cohérence du texte et de ménager le secteur suite aux atermoiements du gouvernement sur les retraites agricoles notamment, je vous propose, comme je l'ai fait en commission spéciale et lors de la discussion générale de supprimer cet article, s'il s'était agi d'une expérimentation pour impulser des pôles de compétence qui se spécialiser sur un sujet dans certaines régions, pourquoi pas, mais là il s'agit d'un transfert assez floue, assez flou sur les transferts de compétences flou sur les transferts. De ressources humaines et de rajouter qu'en transférant les compétences vous allez transférer les contentieux car ce n'est pas qu'un transfert d'accompagnement et de conseils à mais c'est également un transfert de contrôle et puis je voudrais conclure et et pour marteler que quand il y a une erreur dans un dossier pacsé le paysan qui est responsable et, dans ce que vous proposez, ce sera pareil, alors où est le droit à l'erreur dans ce texte, où est la cohérence. Nous allons dans l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur sur ces 2 amendements de suppression.

d'une part, cet article répond aux attentes de certaines chambres et culture, et je pense notamment à Chambre écriture de de Bretagne. Sur lequel nous avons été sollicités et je pense que certaines entre vous être concerné au 1er chef d'autre part, la Commission il y apporter de substantielles améliorations et en particulier en particulier, j'insiste là-dessus parce que ça me paraît vraiment primordial le fait de s'assurer que les chambres départementales, je dis bien les chambres départementales devront être d'accord pour procéder à des transferts de compétences dans le cadre d'expérimentation, à savoir, ce sont les conseils d'un ministre Sion des chameaux, des d'agriculture départementale qui diront : nous sommes d'accord ou pas d'accord d'intégrer donc la chamade régionales ou de fusionner à la chambre régionale ailleurs la raison pour laquelle la Commission vous proposera également manne demain similaire sur les transferts de personnels, parce que dans les amendements, il y a derrière aussi ce problème de transfert de personnel, par conséquent, le fait de supprimer cet article me paraît tout à fait excessif et c'est pour ça que la commission ou propose un avis défavorable sur les 2 amendements. Merci Monsieur le Président, l'avis est défavorable, même si les raisons ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui amènent la Commission a le formulaire ainsi l'article 19 dans sa rédaction initiale prévoyait effectivement la possibilité pour le gouvernement de prendre une ordonnance de manière à mettre en place une expérimentation sur la régionalisation, d'un certain nombre de fonctions de compétences ou des exercices menés par les Chambres d'agriculture nous regrettons je dis très tranquillement et très clairement que la commission spéciale et fait le choix de soumettre la possibilité d'une telle régionalisation un accord unanime des chambres départementales concernées, nous poursuivons un objectif en réponse à monsieur le sénateur, qui est de faciliter à la fois la mutualisation et le regroupement à l'échelle régionale d'un certain nombre de fonctions supports et j'insiste sur l'objectif, les fonctions support, et non pas les fonctions de conseil et nous avons un 2ème objectif, qui est permettent de faciliter la ou les chambres sont particulièrement volontaire la mutualisation de certaines fonctions du conseil, monsieur le rapporteur à l'instant Chambre les chambres pardon bretonne qui ont fait l'objet d'débat je le je le constate ici comme à l'Assemblée nationale, puisque ces chambres ont, par la mise en réseau d'un certain nombre de compétences pris la décision de confier à telle chambre départementale un conseil spécialisé sur telle domaines d'activité à telle autre un autre domaine de conseils, ce qui est peut-être géographiquement un peu éloigné, mais ce qui permet de concentrer l'effort, c'est d'offrir un accompagnement particulièrement adapté, donc l'avis est défavorable sur les amendements de suppression et je le répète, pour la clarté du débat et la suite de nos échanges à l'occasion de la navette parlementaire avec un regret sur le le verrou avec la commission spéciale adoptée par le fait de, de, de, de, de, de rendre obligatoire, pardon, l'accord de toutes les chambres départementales. Alors rendez-demande d'explication du plomb. Oui, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, si je ne suis pas un régionaliste dans l'âme, j'aurais envie de soutenir cette amendement de suppression de l'article 19. Le rapporteur, comme il l'a dit laisse la possibilité aux chambres de choisir et je suis un démocrate, donc je ne voterai pas la suppression de l'article 19. Par contre, les explications du ministre me conviennent. Pas complètement, je pense que la massification et la mutualisation ne sont pas obligatoirement la source de d'économie et que l'agriculture ne peut pas être traitée comme toutes les activités pour la simple et bonne raison, je donnerai l'exemple de ma région. Auvergne-Rhône-Alpes 12 départements 11 chambres d'agriculture des agricultures aux antipodes entre de la vigne de l'élevage entre presque 100 mètres d'altitude et plus 2700 mètres d'altitude des revenus disparates et tout cela, regroupés dans une chambre régionale qui devrait par le principe d'être regroupés et par le principe d'être régional régler tous les problèmes de régulateur des territoires.

Oui, monsieur le président Monsieur ministre, mes chers collègues. J'ai du mal à comprendre le sens de cet article dans dans ce texte. Parce que la portée est bien plus importantes, et je partage complètement votre propos. Oui, alors je me méfie toujours du du provisoire de l'expérimental parce qu'on a vu dans les débats depuis hier que l'expérimental, en fait, on expérimente pas tant que ça, jusque dans les propositions, il y a eu des refus des positionnements qui est à l'opposé de l'expérimentation. je je partage complètement le propos je veux. Pour la régionalisation. Avec cette France qui soudainement s'est concentrée dans de grandes régions si je prends le grand test, on a même problème. Je n'enlève en rien du tout de ce que de propos de mon collègue Laurent du plomb, c'est exactement le choses dans bon nombres de grandes régions comptez côté constituée. Mais il y a un 2ème problème au-delà de, de, on va avoir débat ici dans cet hémicycle, dans quelques semaines sur les conséquences de et dans le texte sur les états généraux de l'alimentation et qu'est-ce qu'on découvre dans le texte du gouvernement qui, à l'opposé de ce qui est dans le texte la. On propose tout simplement de séparer le Conseil de la vente et on va effectivement alors je je parle sous silence je sous silence et circuits courts mais je, je, je reviens très sérieusement au conseil le conseil, c'est la proximité, le conseil c'est le terrain, le conseil c'est pas des personnes qui sont sur la route en train de faire dès que le Conseil n'oublions pas et peu en plus à 80 kilomètres heure, donc non mais sincèrement sérieusement si on reste les pieds sur terre et et c'est pour ça que je pense que le débat qu'on a, à cet instant, il y aurait eu sa place ailleurs parce que c'est pas de la confiance, là c'est un débat d'organisation territoriale alors je connais très bien la région Bretagne Cain identité qui a une réalité à laquelle il faut répondre, le seul problème c'est qu'on est en train d'une manière indirecte de dessiner autrement l'organisation territoriale des chambres d'agriculture, donc j'ai pas demandé à suppression mais sincèrement, je ne voterai pas pour non plus, je vais m'abstenir mais sincèrement je ne comprends pas, et je souhaite que dans le cas de la commission mixte paritaire, il y a une évolution du texte, parce que franchement, il faut l'améliorer.

je crois que monsieur le rapporteur a tout résumé et je partage tout à fait ce qu'il a ce qu'il a dit dont il y a des craintes exprimées sur la proximité et c'est vrai que l'agriculture et les agriculteurs ont besoin de proximité mais je crois que ce qui est essentiel à retenir dans l'article 19, c'est ce qu'a dit monsieur le rapporteur, l'amendement que nous avons au moins nous au sein de la commission spéciale et qui a été accordé, c'est-à-dire donc l'accord préalable des chambres d'agriculture départementale avant le transfert, donc ça c'est une sécurité, mais qui nous permet d'atteindre cet article qui, je le répète, est à titre expérimental, de voir un petit peu commun où vont se passer et se dérouler les choses parce que ça a été dit, c'est les conseils d'administration, donc dès Chamery culture départementale qui in fine et décideront oui ou non du transfert de la régionalisation. Et les conseils d'administration des chambres et culture mais le sont composées des syndicats agricoles, que ce soit donc la FNSEA, la coordination rurale ou la Confédération paysanne, donc laissons leur la responsabilité de ce choix et voyant dans le temps, comment ça va se passer. Donc on est défavorable, donc au retrait de l'article. Madame Delattre, vous souhaitiez prendre la parole à nouveau. Oui je j'entends bien ce que me dit le rapporteur je pense que, on le verra dans l'article 23, nous avons été capables, nous serons capables d'accepter des expérimentations, par exemple sur les cartes d'identité ou expérimenté sur 4 départements, nous aurions peut-être pu circonscrire cet ce cet amendement par un droit à l'expérimentation de la Bretagne, que je respecte, et qui manifestement manifestement est quasi la seule à vouloir expérimenter ce dispositif donc je trouve dommage que pour une expérimentation nous obliger ont effectivement les chambres d'agriculture à rentrer dans ce dispositif, et on l'a entendu, vous n'allez pas le même état d'esprit que le gouvernement aujourd'hui sont les chambres d'agriculture, demain, ce sont les chambres de métiers, les chambres de commerce qui seront par voie d'amendements proposés ainsi donc moi je vous trouve un peu tous timide, c'est dommage, parce que nous avons vraiment l'opportunité là maintenant de supprimer cet article, chacun prendra ses responsabilités, merci. Eh bien moi j'entends, j'entends les différents arguments. Je l'ai dit, ça a été rappelé, je crois qu'il est nécessaire de ne rien imposer sa la vie des chambres départementales. Ce que je regrette, ce que je regrette, ce qui a été fait par la chambre de commerce. Et je suis désolé mais j'ai, je suis élu dans un département rural mais tout centraliser dans les métropoles. C'est une catastrophe. Et ce que je regrette, a les chambres de commerce et que par exemple.

et le pauvre petit département de l'Aveyron qui est un département d'élevage. Mais le voeu que je formule le voeu que je formule. que je n'espère pas du tout et que si un jour il y avait le charme régionale de l'Occitanie. Que le service élevage soit en Aveyron, rien n'oblige le service et l'hommage à à être transposée au niveau de Toulouse et de Montpellier. Kohl s à la production mais viticole, là où il y a vraiment la production viticole, je prends l'exemple de de l'élevage, ça peut être d'autres productions, je crois que dans ce pays, dans ce pays et saine débat profond que nous devons avoir des moments, on a, on a pris l'habitude de tout centraliser. On l'a vu avec la loi notre. Les transports scolaires centralisé à la métropole toute tous les services des des régions et centralisé à la métropole où quasiment tous, sauf peut-être les transports scolaires, sauf peut-être les traces Ponce, colère, et encore, mais soyons vigilants, en clair, pour revenir au sujet qui nous concerne, ne rien imposer, surtout ne rien imposer, laisser l'initiative aux agriculteurs en paysan du coin qui sont membres de ces conseils mais sera sur le charme culture pour adapter les plus les plus lisible à prenait soin de ne pas hypothéquer l'avenir et par là on ça au personnel qui fait l'objet des amendements suivants : voilà ce que je voulais ajouter. Merci Monsieur Laporte, la parole est à notre collègue sont. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, je crois qu'il faut pas qu'on confonde régionalisation et mutualisation parce que bien évidemment je fais partie de la même grande région que notre collègue du plomb et et on va de 100 mètres c'est vrai, mais à 4807 mètres et c'est vrai que la Savoie et la Haute-Savoie, font partie de la grande région et et c'est vrai que c'est dur, ce sont les agricultures différentes les unes des autres, mais on peut régionaliser en gardant une départementalisation en terme de conseils, il est évident qu'on va faire du conseil en élevage, en Savoie et en Haute-Savoie, le même qu'on allait plaine de la Limagne, etc, c'est évident, c'est, c'est le bon sens paysan qui va faire qui La régionalisation permettra d'avoir un discours et d'imaginer un projet agricole. Régionales : comment on peut imaginer aujourd'hui réfléchir, département par département, on organise une solidarité territoriale par l'agriculture, donc évidemment la régionalisation et pas synonyme de départ possession de la politique agricole départementale. Merci. Merci, chers collègues, je n'ai plus de demandes d'explications de la donc je vais donc pour mettre aux voix, ces 2 amendements identiques de suppression, je vous rappelle que nous avons 2 avis défavorables qui votent pour ces amendements. amendements. Ils ne sont pas adoptées ensuite 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 184 rectifier Madame Delattre.

ça peut ne pas aller dans les grandes métropoles, mais enfin, on l'a vu, hein, pour les régionalisation, moi je suis dans une grande région, la Nouvelle-Aquitaine et les pôles de compétences ont été répartis dans les services de la région entre Bordeaux et Poitiers et Limoges, donc nous allons devoir faire face à ces transferts en tout cas vous allez obliger ses salariés à devoir faire face à des propositions de postes qui vont se retrouver des fois à des heures de route de leur territoire par effectivement cette expérimentation de transfert, alors oui c'est vrai, à la région, j'ai été élu, on a proposé, Bordeaux, Limoges, Poitiers, pour des gens qui étaient donc dans d'autres pôles, ils ont refusé, ils se sont retrouvés sur des postes moins intéressant, donc c'est vrai que c'est un vrai problème de ressources humaines qui qui est posée dans cet article. L'amendement 215 Monsieur Luchon, de la commission spéciale.

l'alinéa 4 qui prévoit de permettre, dans le cadre expérimentation dont les modalités seront définies par ordonnance trace faire ou une mise à disposition de personnels des chambres départementales agriculture vers les chambres régionales.

La commission propose un amendement qui, par souci de cohérence, le texte de la commission spéciale tend à s'assurer qu'aucun transfert aucun transfert ni aucune mise à disposition de personnels ne pourront avoir lieu sans l'accord de la chambre et culture départementales concernées, ça me paraît important, c'est le contraire de ce qui a été fait pour les régionalisation il y a une fusion des régions. Sans m'imaginer les effets de transfert du personnel et là nous demandons vraiment que les et culture départemental si telle était le cas dans le leur avis sur le transfert de personnes. Le sort de s'organiser autrement dit ces transferts de compétences comme de personnels devront donc s'effectuer selon les mêmes modalités c'est-à-dire dans notre corps communs, donc je vous propose, chers collègues de retirer l'amendement 5 84 au profit de celui de la commission donc je viens de de vous commentez vous est proposé, donc un avis défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sont ces 2 amendements, s'il vous plaît. Merci monsieur le président, le gouvernement considère que ces 2 amendements sont des amendements que l'on pourrait qualifier de repli, même si monsieur le rapporteur ne s'est pas associée à l'amendement précédent et donc en cohérence avec la position sur le 1er amendement de suppression l'avis défavorable sur les 2 hommes. J'ai une demande d'explication de vote Monsieur Gremillet. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, je voudrais dire à notre rapporteur, que je me réjouis de son amendement. Parce qu'effectivement il y a un sens d'autant plus que n'oublions pas que la fiscalité sur les chambres d'agriculture et les départementales pas régional et dès lors qu'une chambre départementale fait le choix d'être schémas d'organisation au niveau de son personnel de son conseil auprès des agriculteurs et du secteur forestier, n'oublions pas qu'il travaille aussi pour la forêt et hé bien il l'assume puisque la fiscalité, elle est payée par les agriculteurs au niveau d'un département, donc je trouve que l'amendement, non seulement il responsabilise les acteurs locaux au niveau des départements, il n'empêche en rien une nouvelle organisation territoriale et surtout il fait que c'est ce qu'il décide de s'organiser de tels étaient, mais de telle et telle manière en supportent les conséquences financières sur l'organisation de la chambre d'agriculture, donc je voterai cet amendement, je trouve qu'il est, il de par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure et aux craintes qu'on pouvait avoir, mais encore une fois, c'est dommage de de traiter ce dossier dans ses toiles mais je je vote non. Oui, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, la réponse du ministre en étant défavorable sur cet amendement, nous donne finalement presque un peu de remords de ne pas avoir supprimé l'article. Parce que finalement, quand on se dit on propose à l'amendement qui permet de responsabiliser les gens et comme le dit Daniel Gremillet, d'avoir la possibilité d'y aller ou pas, il y allait et donc de laisser faire la démocratie locale et des territoires, mais comme tout gouvernement dit très clairement : nous sommes contre cet amendement mais ça veut dire que l'idée qu'il a derrière la tête, sa dette comme le Soviet suprême de faire tout ce marché, tout le monde dans le même sens, dans le même rang hé bien là on n'est pas d'accord. monsieur le rapporteur, souhaitait la parole excusez-moi chers collègues. Non mais simplement notre collègue interpelle Monsieur le Ministre, Monsieur le ministre, à mon tour de vous dire de vous glisser une petite réflexion, nous sommes un certain nombre ici d'anciens présidents de département. Mais ne nous voilons pas la face, c'est la machine à la vague de suppression des départements. Mais c'est la réalité, je suis désolé de vous le dire, je suis désolé de vous le dire, ça a commencé par les régions, ça commence par les les pays OTRE les les parcs etc, etc c'est les chambres consulaires et les CCI, où on leur a pas demandé leur avis, voilà là aujourd'hui on essaie de réfléchir sur les Champs et culture et de mettre en place des systèmes qui nous permettra éventuellement de maîtriser jusqu'à présent et est l'objet de ces amendements, en fait partie, mais soyons vigilants. Alors bien sûr que je suis de Bartolone ta liste. Puisque puisque certains mais soyons vigilants simplement sur le personnel aussi sur le personnel, je le rappelle, à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je crois qu'il faut que dans les responsabilités qui sont les nôtres, localement ou où nous avons des amis ici ou là, qui ont des responsabilités, mais faisons et j'ai, j'insiste sur ce point, faisant passer le message que pour nous, une famille Olympe, loi qui restent dans nos départements, c'est vraiment majeur c'est vrai même majeur et que faisons passer ce message que tout ne soit pas centralisé que tous les services ne soit pas centralisé à la métropole. Les transports scolaires, j'ai participé, dans mon département, au transfert de la compétence de transports scolaires. Certaines pas certaines régions ont mis tous les services à la métropole, d'abord, département où elle est arrivée à peu près à sauver, a sauvé les meubles en conservant le service transport scolaire dans le département, pourquoi pour être au plus près du terrain ou des préoccupations pour quelque part faire du clairement sur le transport scolaire, mais soyons vigilants parce que qui dit transport de personnel dit je l'ai dit, je suis désolé de me répéter, dit transfert de pouvoir d'achat des transferts de populations disent de affaires économiques voilà la la problématique. la parole est à notre collègue sont. d'abord, que fait la réorganisation ou les possibilités de coopération à l'intérieur des structures de chambres d'agriculture dans un texte dans une loi de confiance, j'ai du mal, on est normalement sur une organisation on est normalement sur un texte de décentralisation et d'organisation territoriale et j'avoue que c'est, c'est c'est une disposition un petit peu, un petit peu Cavaliere la 2ème chose je je vous écoute, j'écoute le rapporteur, j'écoute un salon d'intervenants et j'ai l'impression qu'il y a un décalage

Transport scolaire c'est pas uniquement un problème de proximité, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait de la mutualisation de la massification dans un certain nombre de cas, on génère des économies et dans un nombre de cas, on génère des coûts supplémentaires sur les transports scolaires, on a besoin des mêmes moyens au niveau départemental et au niveau local pour organiser les transports scolaires, mais en plus on a un service dans les régions, qui est chargé de faire de la formation d'évaluation du contrôle des statistiques etc donc on crée de la technostructure et aujourd'hui le coup et transports scolaires sans amélioration de la qualité des 10 transports coûte plus cher qu'il y a 4 ou 5 ans, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que la centralisation est quelque chose de coûteux, on recrée de l'administration improductives à un autre, un et pour les chambres d'agriculture, moi j'ai j'ai j'ai pas d'avis, mais il faut laisser s'organiser comme elle comme elle le souhaite, et rien n'empêche aujourd'hui une chambre régionale où plusieurs chambres départementales de confier des missions une chambre régionale et qu'on parle de mise à disposition de personnel, on aurait pu penser aussi l'inverse disposition de personnels des chambres régionales en direction des chambres départementales parce que ce genre d'échange doit exister dans les 2 sens, donc c'est un petit peu déboussolés dans ce dans ce débat en tout cas moi je je ne cautionnerait pas c'est évolution parce que je suis profondément décentralisateur et je crois à l'efficacité, humaines et financières d'une gestion de proximité.

pour autant, elles doivent rester dans le département, nous parlions des états généraux de la ruralité et la séparation entre le conseil et la vente, je pense que c'est très bien mais justement ce conseil, il va falloir la portée et la portée, c'est la portée de façon proche des agriculteurs, or on sait que les zones agricoles ça ce qu'on ne pas en nombre d'habitants, ça se compte en kilomètres en kilomètre carré et je pense que le département, c'est la zone la plus grande déjà qu'on puisse faire au niveau de la centralisation pour apporter du conseil, donc voilà, c'était juste pour dire cet article, pourquoi pas, par contre gardé les chambres. D'agriculture départementale est une chose très importante si après, elles veulent mutualiser qu'elle reste libre et c'est pour ça que le texte du Sénat me convient et que je suis vraiment rapporte. Très bien, je n'ai plus de demandes d'explications de vote, je vais commencer par mettre aux voix l'amendement 184 rectifier avec une demande de retrait ou défavorables de la commission défavorable du gouvernement qui vote pour. qui vote pour. Qui s'abstient, il n'est pas adopté aimais trop voilà Mandement 215 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui vote pour. Merci qui vote contre. Gillette adopté je peux maintenant mettre aux voir l'article 19 pas demande explication de vote, je n'en vois pas qui vote pour l'article 19

Merci monsieur le président, cet article introduit un droit à l'information pour une personne mise en cause en cas d'infraction au code de l'environnement et au code forestier une transmission systématique à l'intéressé du procès-verbal constatant les infractions qu'il a commise est ainsi prévu sauf opposition du parquet dans un délai déterminé la dispositions contenues dans cet article, interroge fortement, elle est effectivement une source d'inefficacité de l'action répressive et s'applique dans un domaine régi par nos engagements européens, premièrement ce droit d'accès et déjà organisé de manière générale et équilibrée pour toutes les parties par le code de procédure pénale, sans qu'aucun motif générale ne justifie des dispositions particulières dans le seul domaine de l'environnement aussi les services des parquets et des polices environnementales, sont aujourd'hui débordés et n'arrivent plus à mettre en oeuvre leurs prérogatives avec efficacité en raison de former formalité sans cesse croissante et complexe qui doivent assumer les dispositions de cet article viendrait par ailleurs par ailleurs entravé les investigations lors de l'enquête de police, cette disposition non conforme à nos engagements européens dans le domaine de l'environnement viendrait donc s'ajouter à un contexte de répression insuffisante des atteintes à l'environnement, dont l'érosion croissante de la biographe biodiversité constitue l'une des attaques les plus graves et rappelons que nous faisons partie, nous les êtres humains de sa biodiversité je demande donc la suppression de cet article, il serait plus opportun qu'une véritable politique soit menée en matière de défense de l'lobby de l'environnement avec avec des moyens prévus pour la mettre en oeuvre, merci. Donc cet amendement de le rappeler, vise à supprimer l'article 20 qui prévoit une 13 missions automatiques aux contrevenants d'une copie les procès-verbaux des infractions aux normes environnementales qu'ils ont commises, sauf à ce que le procureur de la République s'y oppose. Il s'agit pourtant d'une bonne mesure qui permettra aux personnes mises en cause, d'être informé au stade de l'enquête préliminaire des infractions commises et de se mettre en conformité avant que d'éventuelles poursuites soient engagées par les procureurs et vous est proposé un avis défavorable. Merci Monsieur le Président, c'est un avis défavorable pour les mêmes raisons, en ajoutant que nous ne partageons pas l'appréciation de l'imprévisible sur le fait que ces dispositions ne respecterait pas les engagements européens et qu'effectivement, comme le rappelait monsieur le rapporteur, l'alinéa 7 de l'article qui quitte ainsi proposé prévoit que le procureur puisse s'opposer à la transmission s'il considère que cette transmission serait de nature à véritablement entraver l'enquête donc l'avis défavorable. Pas de demandes d'explications de vote, je n'en vois pas 2 avis défavorables je mais aux voix l'amendement 127 qui vote pour. Merci qui vote contre.

Président, ce ministre mis chers collègues, cet amendement et là encore, il est de bon sens, cette permettre un exploitant qui vient d'être contrôlé, qui vient d'avoir recevoir du préfet, le procès verbal du contrôle qu'il a subit au titre des installations classées de lui permettent effectivement d'établir le contradictoire et ses d'autoriser sous d'aller au minimum de 15 jours de lui permettent effectivement de faire parvenir à la préfecture, services concernés : le contradictoire sur le contrôle qu'il a subi ça d'autant plus d'intérêt qui est dans le sens de l'objet de la société de confiance et d'autant plus encore qu'il peut permettre, puisque le contradictoire peut permettre d'apporter des réponses qui ne figurent pas notamment dans le train, le cadre du contrôle et parfois d'éviter une mise en demeure qui se réunit-t-il donc de désencombrer complètement l'appareil administratif, c'est l'efficacité cette permettre là encore un équilibre entre le contrôleur et le contrôlé et un délai minimum pour pouvoir agir et importer contradictoire.

actuellement et c'est important ce que je veux dire les exploitants n'ont pas de limite de temps. Non pas de limites tant pour faire part au préfet de leurs remarques sur les contrôles dont ils ont fait l'objet, en imposant aux exploitants d'attendre 15 jours. Avant notre admettre leur réponse et cet amendement vient rigidifier la situation et créer une contrainte pour les exploitants, alors même que certaines d'entre eux peuvent souhaiter faire parvenir leurs observations au préfet plutôt je vais mon cher collègue, c'est soit de retirer l'amendement soit un avis défavorable. défavorable. Istres à la vie du gouvernement s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, la détermination d'intégrer, telle qu'elle propose, monsieur le sénateur, nous paraît en l'espèce inutile puisque le rapport n'est qu'un document administratif formalisant la situation constatée au moment de la visite de contrôle, enfin en informer l'autorité compétente, il faut préciser que tout rapport d'inspection ne donne pas forcément lieu à une mise en demeure et les observations de l'exploitant pourront toujours être entendus, quel que soit le délai dans lequel elles interviennent si la situation constatée donne lieu à une mise en demeure l'exploitation, l'exploitant pardon bénéficiera alors dans le cas de cette procédure contradictoire d'un délai pour présenter des observations, telle que prévue dans le code de l'environnement, donc je m'associe à la demande de retrait et, le cas échéant à l'avis défavorable de la commission. Alors êtes-vous convaincu, chers collègues, retirez-vous l'amendement ou est-ce que vous le maintenez. Dès lors que le rapporteur. Que monsieur le ministre confirme qu'effectivement il y a pas d'aller. Non mais ça va mieux en l'écrivant. l'écrivant. Je suis très sérieux parce que, contrairement à ce que vous dites, Monsieur le Ministre. On le sait qu'il y a pas forcément systématiquement continuité dès lors que l'exploitant est capable justifier Capa erreur. Mais tous ne se termine pas toujours dans cette situation-là, donc, dès lors que le rapporteur et avec Monsieur le Ministre, confirme bien que l'exploitant peut faire contradictoires et si on le contradictoire, aller au-delà des 15 jours je ne peux comment réjouir mais c'était important que ce soit dit notamment dans notre débat, donc je retire cet amendement après fication donnée.

Qui vote pour merci qui vote contre. Qui s'abstient, il est adopté. Après l'article 20 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune nous commençons par le 71 Monsieur Durand la foulée. Une présentation unique pour les 2 amendements dans le droit fil des de nos échanges avec notre collègue Karoutchi tout à l'heure, article après article, amendement après amendement, nous nous sommes en train de relever la lourde mission de construire la société de confiance et cette société de confiance, elle a son vocabulaire que nous commençons à maîtriser qui est fait d'efficacité de bienveillance de simplification, de dialogue, de modernité et au registre des termes que nous avons appris à utiliser, il y a aussi celui de la transparence, passé l'ironie, je veux proposer par cet amendement, nous voulons proposer par cet amendement d'élargir la liste des documents administratifs qui sont communicables au public le principe fixées par les textes en vigueur et que les administrations de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent, aux personnes qui ont fait la demande, ce principe souffre néanmoins d'exception qui sont prévues par l'article L. 300 ce tirer reste 5 du code des relations entre le public et l'administration globalement tous les documents dans la consultation, la communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement au secret de la défense nationale à la sûreté de l'État, la sécurité publique à la sécurité des personnes et la sécurité des systèmes d'information, des administrations, mais aussi les avis du Conseil d'État et des juridictions Al-Misrati veut les documents de la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes et documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, etc, au sein de cette seconde catégorie, nous proposons que les documents qui n'ont pas le statut de documents préparatoires puissent être communicables au public, les avis du Conseil d'État et les rapports et communication de la Cour des comptes, le Champ de notre amendement 71 est clairement circonscrit dans l'hypothèse où le Sénat ne retiendrait pas cette rédaction pourtant relativement modeste, nous proposons un amendement de repli 72 qui circonscrit encore un peu plus le Champ pour prévoir que les avis du Conseil d'État sur les projets de loi, les propositions de loi et les ordonnances soient publiés en ligne et communiqué aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ses avis sont pour l'essentiel déjà publié sur internet, sur Legifrance, mais pour l'instant cette publication est au bon vouloir du gouvernement, donc nous proposons assez simplement de faire de la publication des avis du Conseil d'État sur les projets et propositions de loi et sur les ordonnances, la règle de droit commun, voilà ce que nous attendons de sa transparence. Merci, cher collègue, c'est monsieur le président de la commission spéciale qui va lui donner l'avis de la commission. Oui, qui va tenter de suppléer temporairement le rapporteur Jean-Claude Luche alors le commentaire évidemment il est commun aux 2 amendements, mon cher collègue, d'abord, l'amendement 71, vous l'avez dit tant à ce que les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives. Ainsi que les rapports à diverses communications de la Cour des comptes, ça communicables au public. à défaut, par l'amendement 72, vous souhaitez que seuls les avis du Conseil d'État sur les projets de loi les propositions doit les ordonnances soient publiés. Alors je partage évidemment et je pense que nous partageons parfaitement l'objectif de transparence de ces 2 amendements mais il semble toutefois qu'il pose 2 problème de constitutionnalité en 1er lieu il est nécessaire de modifier la Constitution pour rendre obligatoire la publication des avis rendu par le Conseil d'État, c'est d'ailleurs ce qu'a proposé le groupe de travail sur la révision constitutionnelle, présidée par le président Gérard Larcher, en second lieu, de la même manière, tous les rapports et communication de la Cour des comptes ne peuvent être rendus publics, l'article 47 2 de la Constitution distingue en ce sens, les travaux de la Cour des comptes menée pour l'assistance au Parlement et au Burundi au gouvernement des rapports qu'elle doit rendre public pour contribuer à l'information des citoyens certaines transmission de documents pourraient en outre concerner des domaines sensibles tels que la défense nationale et pour ces raisons. Monsieur le sénateur, je demande le retrait de ces amendements, ou à défaut un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, le gouvernement reprend à son compte les amendements, les arguments pardon présentée par le président de la Commission spéciale et précise d'emblée que nous avons peut-être une divergence d'appréciation sur le caractère des avis du Conseil d'État vous avez dit vous souhaitiez la publication de ce qui ne relève pas des documents préparatoires à nos yeux les avis relève des documents préparatoires, je voudrais aussi préciser, mais j'ai eu l'occasion de le faire la semaine dernière à l'occasion de l'examen de la proposition de loi organique présentée par le groupe, qui a donné lieu à ce même type d'échange. Que ceci d'une relation de confiance entre l'administration, les usagers repose sur un meilleur accès aux documents administratifs et c'est un souci partagé et que depuis le conseil des ministres du 19 mars 2015, les avis rendus par le Conseil d'État sur les projets de textes sont en principe publié sur le site Internet Legifrance, cependant, il est nécessaire que le gouvernement concernent en la matière une marge d'appréciation au regard notamment de la préservation du secret des délibérations du gouvernement et cela renvoie de considérations évoquée par le président de la Commission spéciale les avis du Conseil d'État ne peuvent donc constituer des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration canton rapport et communication de la Cour des comptes, dans la mesure où les rapport public thématique des annuelles sont publiées sur son site internet, l'exigence de transparence dont fait état l'amendement nous semble assez largement satisfaite, la possibilité de communiquer les autres documents produits par la Cour des troncs qui notamment les rapports particuliers portant sur les comptes et la gestion des entreprises publiques qui contiennent éventuellement des informations pouvant conduire à une procédure devant le juge pénal ou la Cour discipline budgétaire et financière, ce par ailleurs de porter atteinte au bon déroulement, ces procédures, ce qui nous incite à la plus grande réserve l'amendement numéro 72 va dans le même sens et donc c'est un commentaire qui vaut pour les 2 donc, si je m'associe la demande de retrait du président de la Commission spéciale, il y a défaut sera un avis défavorable.

Nous voterons pour cette proposition en soulignant puisqu'on est si sourcilleux sur la Constitution, pourrait peut-être se souvenir qu'il y a un article 34.

qui vote pour. Qui s'abstient, il n'est pas. Adopté, je vais pouvoir mettre on voit maintenant l'article 21. Les explications de vote, je n'en vois pas qui vote pour. qui vote pour. Il s'abstient, il est adopté à l'article 21 bis, l'amendement numéro 217 présenté par monsieur le président de la commission spéciale. Coordination Monsieur le Ministre favorable qui votent pour cet amendement 217. Merci qui contre. Qui s'abstient, il est adopté, nous allons voter sur l'article 21. La demande explication de vote qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient, il était adopté les articles 22 et 22 bis sont réservés à l'article 23 monsieur Kern, qui souhaite s'exprimer demandes de parole. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, moi je voudrais revenir au niveau de l'examen de cet article sur le problème de la gestion de la délivrance des cartes grises de véhicules que nous avons connu en fin d'année dernière, effectivement, depuis le transfert des services rendus par les services déconcentrés de l'État dans la délivrance des cartes grises à l'Agence nationale des titres sécurisés, début novembre, le système d'immatriculation des véhicules semble être gérée de manière calamiteuse, le bug de fin d'année a été dantesque puisque le stock de certificat d'immatriculation en attente s'est trouvé un niveau intolérable et garages ont été bloquées, les concessionnaires aux abois et les clients du attend de pouvoir rouler avec leur voiture, nouvellement acquise, certains ont même annulé le rachat, une petite partie du réseau a effectivement été débloqués, mais pas vraiment une victoire puisqu'il ne s'agit que du serveur consacré aux professionnels garages concessionnaires station de lavage habilitées par la préfecture à faire les demandes car de carte grise pour les particuliers en attendant pour les particuliers, c'est toujours la même galère le guichet de la préfecture consacrée à l'immatriculation des véhicules étant définitivement fermé les particuliers n'ont donc d'autre choix pour obtenir leur carte grise que de faire appel au service d'entreprises privées du secteur automobile, le service informatique de celle-ci étant lui en état de marche pour c'est particulier ça tout de même un coût supplémentaire conséquent face à un site défaillant ANTS Point gouv pour le citer, certainement à cause d'un lancement trop précipité, on ne peut rien faire, quels sont donc les garanties que peut apporter le gouvernement en ce domaine. monsieur le Ministre, vous souhaitez répondre à notre collègue. Oui, Monsieur le Président, très brièvement puisque nous avons eu des échanges à nombreuses reprises notamment à l'occasion de l'examen du PLF comme de l'examen des 2 PLFR dans votre assemblée, comme à l'Assemblée nationale, le nombre d'équivalents temps plein, mise à disposition de l'agence que vous citez, Monsieur le Sénateur, a presque doublé au cours des derniers mois, les systèmes informatiques que vous décrivez comme défaillant, ont été reconfigurée retravailler de manière à ce que le retard qui est réel et qui se chiffraient à 800000 cartes grises à une époque qui est aujourd'hui heureusement révolue puisse être résorbé, un travail de vrais option se poursuit, nous avions indiqué à l'occasion de l'examen du PLFR que d'ici la fin du 1er semestre 2018 l'intégralité du stock de retard pourrait être absorbé et ainsi pouvoir offrir aux usagers et nos concitoyens, un service de meilleure qualité, personne ne nie les difficultés qui ont été rencontrés par la plateforme que vous avez cité par le système qui a été mis en place l'objectif que nous poursuivons une marque les moyens nécessaires pour faire en fait en sorte d'y apporter une réponse, c'est passé par des moyens budgétaires des moyens humains et pas reconfiguration du système informatique engageant que l'efficacité enfin au rendez-vous. Merci monsieur le président de la commission spéciale. dans en préambule de ce débat, je veux confirmer je veux même vous alerter, parce que il y a 2 soucis : le 1er c'était un retard ralentissement et donc de l'insatisfaction, mais c'est aussi les services de l'État honteux attiré mon attention sur le sujet des observations de fraude supplémentaires par les pièces qui aujourd'hui arrive de manière dématérialisée là ou par le contact humain et par les services de la préfecture, je dirais l'appréciation Censier sensorielles et tactile permettez sur un simple document m'ont-ils dit d'ailleurs à 80 pourcent de détecter des fraudes donc j'attire l'attention puisqu'on est dans un une démarche de la société de confiance qu'on a beaucoup évoqué que ça reviendra, la question de la fraude, l'État devant être garant de la démarche de qualité, soyons attentifs à ce sujet parce que c'est un sujet qui était important, même s'il est sur la vie quotidienne et de la même manière, madame la rapporteure m'expliquer que dans les retards parfois les les concessionnaires ont dû prendre à leur charge des loyers au profit des clients puisque les clients ne disposait pas de leur véhicule, c'est pas ce qu'on appelle l'efficacité ni la célérité des services dits de l'État. Nous allons pouvoir en venir à l'examen de l'amendement numéro 185 rectifier Madame Delattre nous le présente. Merci Monsieur le Président, oui certains articles prévoit une expert est en augmentation dans 4 départements du Nord, Yvelines et Val-de-Loire Une expérimentation de simplification dans la démarche de délivrance des cartes nationales, identité des passeports et des permis de conduire et des certificats immatriculer qui alors la simplification envisagée par rapport à la procédure actuelle n'est pas d'une flagrant d'évidence quel est véritablement l'impact sur la charge des communes parce qu'encore une fois, on pense à l'usager, mais de l'autre côté de la balance quel sera, effectivement, cette plus-Value au groupe RDSE, nous pensons que cela ouvre à des difficultés d'autant que, comme vous l'imaginez, se passer de la délivrance de titres permettant notamment de circuler sur le territoire commune car d'entités dire entrer ou d'en sortir, se passer de cette, de ce justificatif de domicile, nous paraît compliqué nous paraît dangereuse et, comme vous l'avez entendu c'est une expérimentation qui va se tenir, notamment dans un petit département transfrontaliers comme le Nord, donc nous proposons de supprimer cet article. Quel est l'avis de la Commission sur cet amendement de la rapporteure. cet article prévoit, dans le cadre des demandes de titres le remplacement, à titre expérimental de la fourniture d'un justificatif de domicile par la transmission d'informations permettant l'identification du demandeur auprès d'un fournisseur de prestations attaché à son domicile, l'expérimentation proposée n'a pas d'impact sur la gestion de la délivrance d'éthique par les communes, il s'agit juste d'une simple simplification très mineure pour les usagers en facile expérimentation vise à supprimer la fourniture d'un justificatif de domicile, lors d'une demande de titans les services qui sont chargés de l'instruction d'éthique continue de vérifier le domicile déclaré par l'usager demandeurs selon la procédure qui est définie par l'article 23 et cette nouvelle manière de vérifier le domicile des demandeurs de Titan n'empêchera pas toute fraude comme précédemment, d'ailleurs, hein, mais ça rendra inopérante la falsification des factures parce que ça ça existait concernant cette expérimentation, je souhaite toutefois attiré l'attention de monsieur le ministre sur la contrainte pour les fournisseurs, qui représente les développements informatiques nécessaires à sa mise en place, même si elle est limitée cette contrainte génère une certaine inquiétude, une consultation approfondie des fournisseurs susceptibles d'être concernés par l'expérimentation préalable à sa mise en oeuvre serait aussi la bienvenue, donc c'est un avis défavorable. seule président Madame la sénatrice de lettres poste 3 questions importantes qui vont permettre de préciser la portée et l'intérêt du dispositif de simplification de cet article et je l'espère, madame, vous vous rassurer, vous abordez d'abord le sujet sous l'angle d'éventuelles charges nouvelles pour les communes au contraire et en complément de. Qui a dit : Madame le rapporteur, la disposition proposée constitue plutôt une mesure de simplification pour l'administration, puisque le dispositif de vérification automatique de l'adresse du demandeur, par le biais d'une interface avec le service des impôts ou un prestataire de services devrait alléger le travail d'enregistrement du document par les services des mairies pour les demandes de CNI ou passeport concrètement, en effet, l'agent Mérimée aura plus besoin de scanner et d'enregistrer le justificatif de domicile dans le dispositif de recueil de demandes, ensuite, ce sont les services de l'État madame la rapporteur le disait, seul compétent pour instruire les demandes de titres, c'est-à-dire laisser verte et dépendant du ministère de l'Intérieur qui vérifieront l'existence et la régularité de la déclaration du domicile, ce sera plus Saint-Paul les âgés pour les services de la mairie qui n'auront ainsi plus à manipuler le papier et le nouveau dispositif sera plus sécurisé sur ce point je vous aussi vous en assurer l'usager devra toujours justifier de son domicile, il le fera sous une forme différente dans l'intérêt d'améliorer la lutte conte la fraude documentaire puisqu'un certain nombre de documents papiers fournis font l'objet de falsification et dans des proportions relativement importante en dématérialisé en la procédure on élimine ce risque de pacification, par ailleurs, le texte du projet de loi prévoit explicitement que l'usager fournit une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à son domicile, ça peut être un numéro d'abonné ou un numéro de contrat, ce qui écarte des justificatifs qui ne permettait pas d'apprécier ce lien jusqu'alors donc au bénéfice de ces explications et en complément de celle donnée par Madame le rapporteur, c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Alors que faites-vous, chers collègues, il est maintenu le moment alors je vais pouvoir le mettre aux voix, je vous rappelle que la commission a émis un avis défavorable et que le gouvernement fait de même, qui vote pour, pardon, vous souhaitez la parole, je vous en prie, vous l'avez. merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, je voulais quand même vous faire remarquer que, au moment où on a retiré aux mairies notamment dans les zones rurales, la possibilité de faire des titres d'identité, c'est ces cartes nationales d'identité qui était le meilleur moyen de lutter contre la fraude, parce que dans une commune rurale, nous connaissons nos habitants et nous savons qu'ils habitent là aussi il n'habite pas là on les éloigne et ensuite il faut qu'on invente des systèmes pour vérifier que c'est bien, donc voilà, c'est pour ça que je voterai cet amendement. Alors, mais on voit l'amendement 185 rectifier 2 avis défavorables, je vous le rappelle, qui vote pour. Voilà les derniers sont décidés, on peut compter. Il qui vote contre

merci Monsieur le Président, je ne sais pas si comme moi vous avez décroché votre téléphone pour essayer d'avoir un prestataire et d'avoir un justificatif de domicile, mais vous verrez que c'est très simple, je l'ai fait la semaine dernière au bureau, on téléphone à EDF, on dit j'ai je suis ne nouveau locataire d'un appartement que faut-il faire bah rien, vous nous donnez numéro du compteur et on vous envoie le contrat hé bien à ce type de justificatifs de domicile est utilisée pour faire les pièces d'identité, et je ne parle pas des régions où ça va être expérimenté est utilisée pour faire le permis de conduire est utilisé pour avoir des prestations est utilisé par les squatteurs pour dire : regardez le contre est mon nom est utilisé pour des tas d'documents donc dans le cadre de la procédure que vous souhaitez mettre en place. Et pour justifier, justement, vraiment nous demandons pas une complication dans cet amendement, pour la plupart des abonnés qui sont de bonne foi, mais nous demandons à ce que le prestataire fasse ce minimum de vérifications, ce dossier, et cette question nous l'évoquons au Sénat depuis des années parce que il y a des usurpations d'identité que l'on ne peut pas prouver et qu'on arrive, on est en train de se battre, parce que justement le justificatif d'EDF, de GDF ou autre chose est établie au nom, et la personne se bat pendant des années pour essayer de retrouver il est est utilisé dans des tas de cas donc EDF dans une question j'avais posée au gouvernement en 2014 EDF m'avait répondu qu'il y aurait dorénavant un code qui justifiait l'attestation que le contrat existait bien pour le domicile, je demande pour valider toute la démarche qu'effectivement les opérateurs procèdent à la réalité de l'installation de la personne dans le domicile et non pas sur un simple appel téléphonique, je vous invite vous et les services de faire le test, et vous verrez comment c'est facile de prouver que vous habitez un appartement que vous n'habitez pas. Alors quel est l'avis de la commission madame la rapporteure. Merci monsieur le président, ce sera un avis défavorable, parce que cet amendement contraint les fournisseurs de biens et services attachés domicile missiles à établir une attaque n'attestation provisoire des domiciles à vérifier auprès du précédent titulaire du contrat, la même adresse le changement titulaire alors on entend bien votre votre objectif de sécurisation des des justificatifs, mais il me paraît pas envisageable de demander à des enquêtes entreprises privées d'effectuer untel, travail de vérification qui est du ressort des services instructeurs des des titres, c'est la raison pour laquelle on la Commission a donné un avis défavorable à votre. Monsieur Oui, Monsieur le Président, l'avis est défavorable de la même manière, d'autant plus que le gouvernement n'est pas tout à fait convaincu que votre proposition, madame la sénatrice sont en lien Direct avec le texte du projet de loi que nous examinons ce texte porte sur une la justification du domicile dans le cas de l'instruction d'une demande de titre, vous faites plutôt référence aux obligations qui devrait être celle d'un fournisseur de services, il conclut un contrat avec un particulier, c'est la raison pour laquelle il nous semblait que le le lien a été un peu éloigné, vous avez cependant raison sur le fait que la vérification de l'adresse soit importante et le dispositif 2 des points accueil qui est un code-barres sécurisé permettant d'audition 2 d'authentifier pardon des documents utilisés par exemple par EDF, Bouygues Telecom ou encore Engie mises en place par le gouvernement il y a quelques années, a permis de limiter le risque d'effacer de face, de falsification, pardonnez-moi des justificatifs et le projet de loi se situe pour nous à notre niveau, en prévoyant que l'usager délivré à l'administration une information qui permettent son identification auprès d'un fournisseur et donc en en complément de ce que dit Madame le rapporteur l'avis défavorable à moins que vous retiriez amendement. Cassien. Il y a, vous vous doutez bien, j'avais pas retiré l'amendement, d'autant que Madame le rapporteur, me dit que c'est des services instructeurs de titres qui vont vérifier mais les services instructeurs de type se fonde sur le juste et Verratti de domicile, or ce justificatif de domicile n'est absolument pas vérifiée, donc à partir du moment où il est pas vérifier, c'est toute la chaîne qui n'est pas en place, or on fait reposer

faite constaté à plusieurs reprises les faits, alors j'ai pas fait tous les fournisseurs, j'ai téléphoné, je l'ai vu aussi à l'occasion, déménagement, vous donnez votre nom vous donnez numéro du compteur, c'est pas trop compliqué et vous recevez dans les 2 jours, le fait que vous avez un nouveau contrat, il vous suffit de payer le contrat et vous avez, vous existez à ce domicile et après ça, c'est toute la chaîne, y compris la chaîne d'usurpation d'identité qui est en cours, donc je maintiens cet amendement j'espère, j'espère qu'avec ce gouvernement, puisqu'avec le précédent, il m'a pas entendu, il puisse se pencher un peu plus

Ministre, apporter mon soutien à cet amendement parce que je trouve que ça coule sous le bon sens à un moment donné on peut pas accepter de voir partir tout un tas de procédures avec des papiers qui perd, qui permettent d'aller usurpé l'identité en allant chercher un permis de construire autre chose avec une adresse qui correspondrait à quelque chose de fictif, on fait exactement la même chose pour plein d'autres pour j'étais pas plus tard que lundi sur ma commune dans une tranchée, qui étaient faites par des employées pour changer les réseaux d'eau et d'assainissement, une colonne de gaz. Bon, ça s'est mis en place il y a un système de clapets qui arrêté bien sûr on a Brandt dans le combat pour une colonne de gaz qui fait un centimètre et demi de diamètre on a déplacé les pompiers, on a déplacé, bien sûr, Gaz de France

donc on a enlevé l'appel, l'entreprise qui travaillaient n'a pas pu travailler pendant plus de 24 ans, et c'est une autre entreprise qui est venu habilité qu'on a imposé à l'entreprise qui s'occupe du gaz aujourd'hui pour ni réparer le les tuyaux, alors on voudrait nous dire qu'on peut mettre tout un tas de contraintes aux entreprises pour certaines choses et puis sur des choses comme celles-ci, parce que c'est le bon sens et parce que c'est simple et bien on ne peut pas le faire. Je voudrais rappeler que la réorganisation des services d'instruction des des titres justification, c'était de dire on va lutter contre l'usurpation d'identité, qui est un véritable fléau.

non mais attendez, quand vous faites une demande et vous dites voilà vous donner une justification par exemple votre abonnement à la au service des autres communes, on vous le refuse,

je ne sais pas s'il faut, nous, on va le voter ce ce cette cette amendement parce qu'il y a vraiment là un vrai qu'un problème est encore une fois, c'est parce que il y a beaucoup trop d'usurpation d'identité. C'est une des raisons officielles à c'est la raison pour enfants et c'est pour éviter cela,

Bon bien écoutez, je vais pouvoir mettre aux voix cet amendement 13 rectifier avec. Madame l'emporteront à nouveau.

non mais vous pouvez alors moi je veux bien vous allez vous allez voter l'amendement mais ça changera rien du tout, c'est vrai que c'est un, c'est un sujet, je pense qu'il faut le regarder, il faut éviter de le mettre ici sincèrement et que Monsieur monsieur le ministre engage à essayer de trouver une solution, mais sincèrement, là, ça sert à rien de médecins alors on on est en train de dire que dans ce texte, il a tout et n'importe quoi mais finalement on en ajoute encore donc sincèrement, moi je, je préférerais vraiment que vous suiviez l'avis de la commission merci. Alors cette fois-ci, je vais mettre aux voix cet amendement 13 rectifier 2 avis défavorables venez d'entendre à nouveau Madame la Laporte qui vote pour.

Qui vote pour l'article 23 merci qui vote contre qui s'abstient, il est adopté l'article 23 10 une demande de paroles de Madame de remédier. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, le 10 avril 2015 lors des discussions de la loi Macron, j'ai présenté un amendement relatif au permis de conduire des Français de l'étranger, cet amendement a été adopté à l'unanimité par notre Haute assemblée avec l'avis favorable de la commission spéciale exprimée par notre collègue Madame Dominique Estrosi Sassone mon amendement s'inspirait d'une résolution adoptée par l'Assemblée des Français de l'étranger, en mars 2015, sur le rapport de notre collègue Ronan Le bleu à leurs conseillers à l'AFE la résolution demandait au gouvernement de permettre aux postes consulaires de délivrait des duplicata de permis de conduire en cas de vol ou de perte des relevés d'informations restreint ainsi que des permis de conduire, internationaux, elle demandait une simplification de la procédure de rétablissement des droits à conduire pour les Français qui ont été titulaires d'un permis de conduire, français et qui revient en France l'AFE demandait encore que les échanges réciproques de permis de conduire soient favorisés, notamment dans les États ou provinces de pays fédéraux et que l'échange du permis moto soit étendue quand l'échange du permis voiture existe déjà, enfin elle demandait 15 fascicules d'information et une rubrique du site internet du ministère des Affaires étrangères, aborde tous les cas de figure, et soit régulièrement mise à jour, monsieur Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, sur ces bancs me répondaient qu'il était favorable, mais qu'il préférait régler la situation par décret, il s'est engagé à ce moment-là à propos à promouvoir le décret d'ici le mois de juillet, il s'est engagé à faire réaliser des études sur la compatibilité de plusieurs mesures contenues dans mon amendement avec le droit européen, il m'assurer que si cette compatibilité était reconnu il corrigerait le projet de décret alors qu'en cours d'examen danser alors je suis intervenu à plusieurs reprises auprès de lui pour obtenir la publication du décret qui est intervenue, mais n'a pu couvrir toutes les situations, l'article 23 bis adopté par l'Assemblée nationale, opportunément amendé par notre commission spéciale démontre que toutes les demandes de nos compatriotes n'ont pas encore été satisfaites, il fait un pas de plus, je ne peux que l'approuver puisque j'avais moi-même demandé ces mesures avec mes autres collègues sénateurs des Français d'étrangers, dont Richard Yung, qui avait soutenu mon amendement j'ai un regret par rapport à l'article 23 bis, il s'agit d'abord d'une mesure expérimentale, alors que le compatriotes expatriés attendent une mesure définitive depuis des décennies l'expérimentation doit durer 18 mois, elle aurait même duré moins longtemps si notre commission n'en avait précisé le point de départ, j'espère que le gouvernement en fonction dans 18 mois aura la sagesse de pérenniser cet article et d'aller même plus loin : je salue néanmoins cette nouvelle avancée que je voterais. Parole est à notre collègue Richard Yung.

Merci monsieur le président, dans l'article 23 bis met en place une expérimentation qui permet aux Français de l'étranger, de justifier de leur domicile par un certificat de résidence qui est délivré par le consulat pour obtenir un duplicata de permis de conduire, français ou un certificat d'immatriculation pour un véhicule détenus en France, le gouvernement nous a indiqué une difficulté concernant l'application de cette expérimentation au certificat de d'immatriculations en effet la délivrance de ce certificat est obligatoirement associé au paiement d'une taxe au profit des régions dont le taux est fixé par celle-ci, dans ce cadre, il est nécessaire de disposer d'une justification de l'adresse en France du demandeur, il n'est donc pas prévu que les Français qui résident à l'étranger, demandent un certificat d'immatriculation de véhicules alors en accord avec le gouvernement et afin de préserver les ressources des régions est donc proposé de ne pas inclure les certificats d'immatriculation dans le Champ d'expérimentation. Merci, cher collègue, Monsieur le ministre vie du gouvernement s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, la, la vie est évidemment favorable puisque c'est le fruit d'un travail et d'un échange comme l'a souligné Madame le rapporteur. Très bien, des demandes d'explications de vote. Je n'en vois pas qui votent pour cet amendement de la commission avis favorable du gouvernement. Merci qui vote contre. Qui s'abstient-il être adopté, je vais mettre au bout à l'article 23 bis, ceux qui votent pour. Qui vote contre qui s'abstient il adopté après l'article 23 bis, l'amendement numéro 83 rectifier bis qui le présente. Madame Lepage, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, la production du certificat d'existence chaque année pour les pensionnés de retraite établis hors de France, pose de nombreux problèmes, notamment en raison d'un acheminement postal souvent difficile ces difficultés retarde, voire empêche le versement des pensions de retraite dont enfin leur pension de retraite s'il n'arrive pas à produire dans les délais, le certificat d'existence avec toutes les conséquences financières, sociales et humaines que je vous laisse imaginer la multiplicité des caisses de retraite signifie donc qu'ils doivent effectuer plusieurs fois, la démarche est ainsi les risques de retards se sont multipliés dans le droit en vigueur les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d'existence, elles ne le font pas, selon les témoignages recueillis, cet amendement vise donc à rendre obligatoire la mutualisation de la gestion des certificats d'existence pour entraîner un partage des informations d'existence d'une personne entre toutes les caisses de retraite, cela éviterait aux Français établis hors de France, de devoir produire autant de certificats d'existence qu'ils ont de caisses de retraite. Merci, chers, quel est l'avis de la commission la rapporteure. Merci monsieur le président, sera une demande de retrait, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a prévu l'obligation pour les bénéficiaires d'une pension de retraite, servi par un organisme français et résidant hors de France, de fournir au maximum une fois par an, un justificatif d'existence à leur caisse de retraite des échanges d'information étaient mis en place avec un certain nombre de pays européens, afin que les caisses n'ait plus besoin de demander untel justificatifs la loi de financement pour 2013 a également prévu la possibilité pour les régimes obligatoires, pardon, de mutualiser la gestion de ces certificats afin que les polypensionnés ne soit pas tenue de transmettre plusieurs justificatifs dans des conditions qui ont été précisées par un décret du 13 décembre 2013 il ressort de nos échanges avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qu'un projet de mutualisation de la gestion des certificats d'existence pour l'ensemble des régimes est actuellement en cours et devraient déboucher courant 2019 le ministre aura sans doute le confirmer dans un instant étant en cours d'être satisfait, je vous propose donc de de le retirer, j'ajoute qu'il y a aussi un certain nombre d'amendements qui concernait le même sujet, prévoyant notamment la dématérialisation des justificatifs d'existence qui ont été déclarés est recevable car elle relevait du domaine réglementaire mais la question n'en est pas moins réel le ministe pourrait nous indiquer aussi les mesures qui sont envisagées par le gouvernement en ce sens, donc : demande de retrait. Alors Monsieur Nivel sollicité sur cet amendement. Merci Monsieur le Président, c'est aussi une demande de retrait pour votre amendement Madame Lepage puisque je confirme les propos de Madame la rapporteure au-delà des différentes dispositions qui ont été adoptés, qui ont été rappelés, un système de mutualisation, est en cours de constitution dans le cas du Groupement d'intérêt public Union retraites il va déboucher courant 2019 pour permettre aux assurés de ne transmettre qu'un certificat Ekinci ainsi soit totalement mutualisées donc votre objectif sera satisfait par ce groupe Cegos, ce groupement d'intérêt public, pardon pour ce qui concerne l'interpellation de de madame la rapporteur c'est un sujet sur lequel le gouvernement se penche compris pour faciliter la vie des usagers, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir, y compris par voie réglementaire pour ce qui relève du réglementaire, le chantier mais qu'à qu'à son début, aujourd'hui, mais je peux vous assurer de l'engagement du gouvernement à pouvoir avancer et y compris d'ailleurs à à tenir compte d'un certain nombre de propositions qui ont été faites et qui avaient été formulées dans des rapports d'origine parlementaire, je pense notamment au rapport de Madame Hélène Conway Mouret il qui avait été déposé il y a quelque temps, et dont une partie des mesures seulement été mise en avant. Monsieur, donc vous avez la parole. Merci monsieur le Président, je viens découvrir qu'on ne pouvait pas faire de prise de parole sur un article additionnel, on ne connaît pas assez la procédure donc je profite de l'explication de vote pour revenir pour dire d'abord que je soutiendrai l'amendement qui a, qui a présenté ma collègue pour dire que j'avais présenté moi-même un amendement qui visait la dématérialisation des certificats de vie cet amendement a été retoquée au nom de l'article 41 bon alors on peut discuter pour savoir mais je voudrais dire que pour ma part, je considère que l'argumentation n'est pas fondé à bord parce que un certificat de décès doit être considéré comme un certificat de de naissance ou de ou tout ça fait partie des des procédures normales de de la vie administrative et le fait que on me le on me le renvoie en disant ça ne fait pas partie des actes d'état civil, je trouve que c'est pas quelque chose de tout à fait acceptable, je voudrais dire aussi qu'il y a un certain nombre de de mention de dématérialisation dans différents codes de la propriété industrielle, le Code du commerce, le code général des impôts alors dans certains cas la dématérialisation peut-être législatif dans d'autres cas, elle ne l'est pas, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures et donc je voulais élever une protestation légitime en la matière. Alors, Madame Lepage, vous avez 2 demandes de retrait. Pour le d'abord pour la dématérialisation ai j'appuie tout à fait ce que vient dire mon collègue Richard Yung, il y a vraiment 2 poids 2 mesures, pour ce qui concerne l'Europe très de mon amendement, je dois dire que il y a bien, il y a quelques années de cela Monsieur Baroin m'avait fait la même promesse sur les certificats d'existence et voilà, j'ai, je l'avais cru, j'ai retiré mon amendement et il ne s'est rien passé, Monsieur monsieur le ministre, je veux bien sûr, je veux bien vous croire, mais quand même je suis prudente et donc je ne retire pas. Voilà l'amendement est maintenu, je vais donc le mettre aux voix. Alors, de demandes de retrait ou défavorables commission gouvernement qui vote pour. qui vote pour. Qui s'abstient, il était adopté l'article est ainsi rédigé : article 24, une demande de paroles de Madame Conway Mouret. Merci monsieur le président Monsieur Miss, mes chers collègues, comme mon collègue Richard Yung vient d'exprimer, je je regrette mais aussi très fortement que nous nous ait opposé l'article 41 pour rejeter l'ensemble de nos amendements, j'en avais d'ailleurs déposé 4 pour cette article qui est maintenant vide qui avait été repris par mon groupe politique, bon, en même temps, il est surprenant que l'on oppose au législateur le domaine réglementaire, alors même que ce texte a l'ambition de couvrir tous les domaines en nous permettant de lever un grand nombre de blocages identifié de longue date et dont nous sommes régulièrement saisi par nos compatriotes, alors j'aimerais ici détaillées pour justement ses compatriotes qui vivent à l'étranger et qu'ils sachent bien que je les oublie pas que nous ne les oublions pas, et j'espère, Monsieur le Ministre, que vous engagerais vos services à vous saisir de ces points qui sont peut-être réglementaire et que vous les mettrez en oeuvre alors le 1er visait à simplifier les démarches de demandes de bourses pour les étudiants français résidant hors de France, l'ensemble du dossier rempli et télécharger doit ensuite être envoyée par les étudiants, par voie postale aucune housse des lenteur de transmission de leur dossier entre les pays de résidence et la France pénalise ses étudiants dans leurs demandes de bourse c'est amendement répondait ainsi au souci de simplification des démarches administratives que vous proposez et dans ce cas d'assurer aux étudiants, demandeurs de bourse de voir leur demande prise en compte simplement dans le délai imparti, puisqu'il propose la dématérialisation de la procédure le 2ème amendement visait à compléter une procédure de dématérialisation je vais trop vite relatives aux CAF en effet à l'heure actuelle, cette dématérialisation n'est que partielle, les documents téléchargés en ligne doivent ensuite être adressée aux caisses d'allocations familiales en version papier dans le nombre de pays, on observe malheureusement la lenteur de l'acheminement postal qui porte préjudice aux bénéficiaires, le 3ème visait à simplifier les démarches pour l'obtention de la carte vitale, en ligne avec un envoi dématérialisés, des pièces justificatives pour l'obtention de cette carte, cela pour des personnes éloignées des consulats ou ayant des problèmes de mobilité et enfin le 4ème amendement prévoyait de permettre une pré-affiliation à la caisse primaire primaire d'assurance maladie et ceci pour les Français ont prévu de revenir de manière durable et certaine, en France, on nous a opposé que la mobilité tête une preuve d'instabilité, moi je pense que la mobilité au contraire une richesse qui se nourrit de l'expérience étrangers et qui fait grandir notre pays à chaque retour. Merci monsieur le ministre, vous souhaitiez répondre notre collègue. Oui, juste un mot pour dire à Madame la ministre, que nous, moi, que je connais les amendements qu'elle avait déposé, puisque nous avons eu l'occasion, l'un et l'autre d'échanger leur sujet puisque vous étiez venu les présenter et défendre l'intérêt de ceux-ci, je n'ai pas et le gouvernement n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de telle ou telle amendements aux yeux du Sénat, bien évidemment, mais je puis vous assurer que, conformément aux échanges que nous avons eu après beaucoup des amendements que vous déposez peuvent être traitées par voie réglementaire, et comme nous avons eu l'occasion de de vous le dire mais j'ai, je saisis l'occasion pour le dire devant tous les sénateurs et toutes sénatrice, en particulier ceux issus est élu par les Français de l'étranger, nous aurons à mettre en place prochainement un groupe de travail pouvoir ensemble sur quel sujet, nous pouvons avancer et donner une suite à votre proposition d'amendement par voie réglementaire. Voilà, j'ai pour mettre aux voix à l'article 24 heures qui vote pour. Qui vote pour merci qui vote contre. Qui s'abstient, il est adopté à l'article 25 l'amendement 171 rectifier Madame Delattre. Monsieur Président cet article 25 prévoit 2 dispositifs : d'une part, l'extension des dons par SMS aux à Sion oscillations cultuelle loi 1905 sous le même régime que les organismes faisant appel à la générosité publique et d'autre part, l'obligation pour ces associations cultuelles d'établir des comptes annuels alors si ce second point, alinéa 3 va dans le bon sens et auraient dû d'ailleurs être introduit bien avant dans la loi le 1er point en revanche très inquiétant, à notre avis, c'est pourquoi nous vous proposons de supprimer les alinéas concernés 1 4 et 5 aujourd'hui les organismes faisant appel à la générosité publique bénéficie d'un régime d'agrément allégé pour l'utilisation de services de paiement dématérialisé introduit par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, il apparaît que ce régime n'offre pas de garanties suffisantes concernant l'usage à venir de ce mode de paiement et poserait s'il était étendu aux associations cultuelles de véritables risques en terme de sécurité, manque de transparence de ce moyen de financement comme le paiement en liquide de cartes prépayées liquide qui pourrait paraît provenir de manoeuvres de blanchiment d'argent, manque de transparence concernant la provenance et l'utilisation du don identité du donateur du bénéficiaire finalité du don de telles opérations devrait, a minima, faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution plutôt que de bénéficier de ce régime allégé et puis vous l'avez surtout compris dans mes propos discussion Générac cet article est pour nous un cavalier législatif visant à modifier la loi de 1905 qui établit la séparation des Églises et de l'État, qui reste un texte constitutif de notre République une modification de la loi de 1905 sur le financement mériterait donc un temps d'études et de débats dédiés et non une discussion au débotté, ce que nous regrettons vivement. Alors quel est l'avis de la commission, même le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, déjà au niveau de cet article touche pas du tout à la laïcité en je voudrais rassurer, rassurer les collègues. Absolument pas, absolument pas, d'un mode d'un mode de paiement, c'est une mesure d'égalité de traitement entre différents types d'associations, passant par une modernisation technique du recueil de dons

même principe, exactement la même chose, blanchiment d'argent, moi je suis désolé, hein, il peut, il y a pas, il est pas davantage au niveau des cultes que dans les autres associations, donc c'est un autre sujet, c'est un autre sujet, donc cette nouvelle faculté ne présente pas pas davantage de risques, donc pour les associations, que les organismes faisant appel à l'âge générosité publique qui sont autorisées depuis 2016 et après moi je vais vous dire hein, c'est pas des millions d'euros, hein, ces dons serait plafonné à 300 euros par mois et par personne, toutes associations confondues et 50 euros pardon alors effectivement, même de la moi j'ai bien entendu à la Commission, vous voyez une énorme machine, avec des des milliers de de personnes qui achèteraient des cartes prépayées pour blanchir de l'argent et le passé par ce biais-là, voilà, vous avez beaucoup d'imagination, je pense que même peut-être que vous allez susciter des vocations, moi je pense qu'il faut faire attention, pas, je ne vois pas pour quelle raison il faudrait prévoir un régime d'agrément plus strictes pour les associations cultuelles cultuel que pour les autres, à ce moment-là, il faut faire pareil pour, pour tout le monde, ce que je suggère dans donc dans le niveau de l'objet de l'amendement, sans toutefois le proposer dans dans son dispositif, donc c'est un avis défavorable pour pour votre amendement et sincèrement je pense que de toute façon, les associations cultuelles, elle reçoit des dons de d'autre d'autre nature, donc c'est juste une possibilité plus moderne. Merci Monsieur le Président, comme j'ai eu l'occasion de le dire à Madame Delattre, en réponse à son intervention discussion générale je partage avec elle cet attachement à la laïcité attachement viscéral pour ne pas dire radicale à cette belle notion de la laïcité et comme je vous le disais, aussi je me reconnais que dans une fidélité totale à l'article 1er notre constitution, et notamment son 7ème où, justement, la laïcité pour appeler plus exactement pour rappeler combien notre nation doit y être attachés, j'espère pouvoir vous rassurer sur la portée des dispositions qui sont. Conduite par l'article 25 le bénéfice du mode simplifié de collecte de dons est ouvert en faveur des associations cultuelles par cet article, selon les mêmes modalités de mise en oeuvre et d'encadrement pour les organismes faisant appel à la générosité publique ces modalités constituent de réelles garanties et en particulier en termes de transparence, le fournisseur de réseau ou de services de communication électronique doit adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel résolution une déclaration préalable contenant une description des services proposés

à l'instar des organismes faisant appel public à la générosité des associations cultuelles seront soumises à une obligation déclarations préalables, représentant de l'État et de tenue de comptes annuels pour pouvoir disposer d'un numéro de SMS devront déposer un dossier sur une procédure établie auprès de l'Association française du multimédia mobile qui est demandé par les opérateurs téléphonie mobile pour coordonner l'ouverture de service du service de dons par SMS, comme l'a rappelé Madame le rapporteur, les dons sont limités à 50 euros, avec un plafond mensuel fixé à 300 euros par personne et tout don supérieur à 5 euros doit être confirmé par un second SMS suite à l'envoi du ou des SMS, le donateur reçoit un SMS de confirmation du don contenant un certain nombre d'informations et notamment un lien vers les conditions générales d'utilisation du don par SMS édictées par les organismes bénéficiaires ce même organisme bénéficiaire devra mettre en place une communication appropriés sur les démarches liées au don par SMS mais aussi un dispositif permettant l'identification du donateur, la saisie de ses coordonnées pour délivrer des reçus fiscaux et gérer l'après-dématérialisé de l'abonné qui transmet le SMS de confirmation de l'opérateur pour bénéficier du reçu fiscal, ce qui écarte très largement les craintes que vous avez évoquées en matière de financement de telle ou telle activité, la transparence de l'affectation des dons est garantie par l'obligation d'établir des comptes annuels que l'alinéa 2 de l'article 25 du projet de loi. Prévoit de généraliser alinéa 3 pardon, pas de que vous ne remettait pas en cause, par votre amendement, donc je crois vraiment que nous sommes sur une modalité pratique, il n'y a pas, et je fais référence à des arguments que vous avez évoqué en discussion générale de volonté, ni même de risque de mettre à disposition des associations cultuelles, un outil spécifique ou particulier qui ne bénéficierait pas d'autres c'est un alignement sur le droit d'autres associations, ça n'a en rien une distorsion aux principaux tant par la loi de 1905 par notre attachement commun je crois à la laïcité. Merci monsieur le ministre. Alors, je vais pouvoir mettre au fond monsieur Lalonde pardon. Monsieur le Président, sans mettre en doute les, les, les convictions profondes laïque du ministre et les explications de la rapporteure néanmoins du moment que dans une loi, on va prévoir quelque chose et qu'on dit culturelle c'est qu'a priori ça manquait. C'est qu'on a voulu insister sur un fait particulier et d'un autre côté, le fait de d'un d'être dans un pays où le principe et la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire à chacun des individus de faire un certain nombre de choix pourquoi devrait-on mettre en place un système qui permettra à un moment donné de par le fait d'un don de bénéficier d'une réduction fiscale. Et donc je voulais simplement dire que la le, le, le, la position de Madame de Latran est aussi la nôtre.

et de modifier l'article 29 et ça ce n'est pas quand même comme ça autour, même s'il s'agit d'une loi pour un État au service d'une société de confiance, ça ne se fait pas comme ça, c'est, c'est trop, trop grave surtout que tout à l'heure à l'article 38 on on va nous demander d'exclure les associations cultuelles de listes d'intérêt général, donc voilà, difficile de s'y retrouver vos arguments Monsieur le Ministre, non pas qu'on va. Alors Monsieur le Président. 2 petites précisions : d'abord la première sur l'objet même que je veux rappeler, il s'agit simplement d'inscrire une modalité pratique dans le Code monétaire et financier, donc ça il y a, il y a pas de d'autres d'autres objets, que celui-ci, et puis le 2ème puisque j'entends qu'on a besoin de rappeler, si besoin était, l'attachement de chacune et chacun, ici, il y a pas de brevet de laïcité, je crois que nous avons tous démontré dans le passé j'espère continuer de le faire dans l'avenir l'attachement sur tous ces bancs. à la valeur de la laïcité dans notre République, donc ne ne, ne nous trompons pas débat. On a un amendement, on peut être pour on peut être contre mais n'essayons pas de dévoyer le débat, je crois que le ce n'a pas besoin de ça et puis, pour tout vous dire, on a encore beaucoup de travail, il faut prendre le temps. On va moins vite qu'hier, donc je nous invite à continuer à être constructif sage serein, et puis si possible, aller dans le même sens que celui qui est proposé par notre rapporteur. Alors, je vais pouvoir mettre aux voix cet amendement 171 rectifier avec 2 avis défavorables qui vote pour.

qui vote pour. Il n'est pas adoptée. Nous passons à l'examen du 21 rectifier Bissau monsieur Morel présente. Merci beaucoup président cet amendement que j'ai l'honneur de vous proposer et qui a été signée par plus de 70 sénateurs, que je remercie reprend une proposition issue du rapport que nous avions rendu en 2015 au nom de la délégation aux collectivités locales sur le financement des lieux de culte par les collectivités et il vise tout simplement à prévoir la transparence sur le financement des lieux de culte aujourd'hui quand se construire un lieu de culte et disons les choses clairement, une mosquée dans une commune, ne sait pas qui la finance, on ne sait pas qui est derrière ce projet, alors très souvent, on nous dit que ce sont des dons qui ont permis de financer cela, mais parfois il y a tellement d'argent liquide qui circule que que Tracfin est amené à se poser des questions, donc ce que nous proposons, c'est tout simplement que lorsqu'il y a un projet de construction d'un lieu de culte il à un bilan financier qui soit au terme de cette construction produit bilan financier certifiés par un commissaire aux comptes, beaucoup ont considéré au cours des derniers mois des dernières années, qu'il faudrait interdire le le financement des lieux de culte, notamment par des États étrangers, je crois qu'avant d'envisager ce genre de mesure, il faut déjà connaître la réalité de la situation et la réalité de la situation, ça passe par la transparence, qui me paraît sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs une impérieuse nécessité. donc, cet amendement soumis tout projet de construction d'un lieu de culte, à l'élaboration d'un plan de financement prévisionnel et certifiés par un commissaire aux comptes et retraçant ainsi l'origine des fonds fonds modalités étant fixé par décret en Conseil d'État, donc il reprend une recommandation, la numéro 7 du rapport de la délégation collectivités territoriales du Sénat sur les collectivités territoriales et financement des lieux de culte, alors cette disposition concerne indirectement, le financement des associations cultuelles qui est traité aux articles 25 ici et 38 du projet de loi, il s'agit toutefois d'un sujet spécifique sur lequel je n'ai pas pu mener d'audition, je sais par ailleurs qu'il a une réflexion actuellement en cours au niveau de l'exécutif en conséquence je souhaite connaître l'avis du gouvernement, sur cet amendement, c'est en tout cas ce que la Commission a souhaité, Monsieur le Ministre. régime général du régime juridique des cultes, la proposition vous faites et qui est issu d'une recommandation de du rapport que vous avez cité aussi est intégré dans sa réflexion, mais à ce stade et au moment où nous parlons, le travail n'est pas suffisamment avancé pour que nous puissions avoir un avis définitif, la réflexion est en cours, ce n'est pas une manière de l'écarter, bien au contraire, c'est plutôt une demande de retrait de l'amendement en vous garantissant que cette idée est prise en compte par le ministre de l'Intérieur, dans le cadre de la réflexion qu'il mène avec les différents cultes sur le régime juridique.

pour savoir s'il faut ou pas de la transparence, c'est quand même assez extraordinaire de dire j'ai pas idée du fait de savoir si c'est utile ou pas, la transparence 1er point 2ème point monsieur le ministre, vous nous dites, j'ai noté une réflexion est en cours mais aussi, ça fait 3 ans que les gouvernements successifs nous dit ça, j'ai déposé ce rapport au début de l'année 2015 et comme l'actualité était quand même un petit peu compliqué du point de vue notamment des des attentats je, je, j'ai mis un petit peu de côté les propositions de ce rapport, parce que je voulais pas qu'il ait d'amalgame entre l'actualité de ce rapport, qui est un travail de fond que nous menions depuis 2 ans, on a eu ensuite un débat dans l'hémicycle, le gouvernement de l'époque a dit on va engager une réflexion, le ministre de l'intérieur de l'époque, organisé des tables rondes, des réunions qu'est-ce qui s'est passé. Rien, et 3 heures après pour une mesure aussi simple, aussi évidente que de se dire : il faut peut-être savoir comment ces ces lieux de culte sont financés tout ce que vous trouvez à de répondre au nom du gouvernement, c'est une réflexion est en cours, franchement, au bout de 3 ans continue à répéter ça en boucle, ça me paraît vraiment pas sérieux ni raisonnable ce genre d'arguments qui ici peut dire je suis compte la transparence qui, s'il peut dire que ça n'est pas nécessaire de savoir comment sont financés les lieux de culte quand on sait très bien, comme je l'ai dit que Tracfin s'interroge quand on teste très bien que quand on connaît les sources de financement, on sait qui est derrière ces lieux de culte, avec tout ce que ça peut impliquer en termes de de sécurité, terrorisme, on est pour la transparence, on est pour l'opacité, c'est ça la vraie question, donc, évidemment, je maintiens cet amendement et j'espère qu'il sera voté. parole ce président ben après. Simplement pour dire que nous soutiendrons cette proposition de bon sens. Très bien le président bat la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, en ce qui me concerne, je ne voterai pas cet amendement en dépit des intentions louables qu'il contient ses intentions, quelles sont-elles, manifestement, lutter contre le développement de mosquées salafistes financés par des États du Proche-Orient ou des ressortissants de ces États cette motivation, elle était tout à fait pertinente nul ici ne la conteste, mais par la généralité de la prescription, qui est ainsi posée, on voit que par rapport à plus d'un siècle d'application de la loi de 1905 on franchit à travers cette disposition une limite qui n'a jamais été franchie, n'oublions pas que nous légiférons non seulement pour les salafistes et l'auteur principal auteur de l'amendement, a bien expliqué que c'était sa principale motivation : la lutte contre le terrorisme, mais nous légiférons aussi pour toutes les religions de notre pays, l'Islam la religion juive, la religion protestante la religion catholique, jusqu'à présent, c'était la liberté qui prévalait est-ce que véritablement au nom de la transparence, on doit remettre en cause la liberté, nous avons des moyens et nous l'avons fait encore récemment dans la loi pour sortir de l'état d'urgence, de contrôler ses mosquées qui appelle au Crime, mais nous ne devons pas pour autant englobée dans une mesure qui restreint la liberté du culte toutes les religions qui ont droit de cité depuis si longtemps en France.

Oui, en entendant le président de la commission de des lois, je me demande si j'ai pas bien compris le le texte de l'amendement, l'amendement dit tout projet de construction par des groupements locaux par des associations cultuelles d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, c'est l'objet d'un plan de financement prévisionnel mentionnant dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, l'origine des fonds et certifiés par un commissaire aux comptes, point, il dit pas qu'on va contrôler, voire interdire voir limitée telle ou telle financement c'est simplement une question de transparence, moi ça me paraît à notre époque on exige la transparence pour des Budgets bien plus mince que celui de la construction de la Médicis religieux, ça me paraît tout simplement naturel que de demander ça, ça devrait d'ailleurs existait avant, sans qu'il ait besoin de de d'événements malheureux comme on en a connu depuis 2 ou 3 ans. La parole est un blâme V rien. Merci monsieur le président, monsieur ministre oui je voulais dire effectivement rebondir là-dessus, ça n'interdit pas, ça n'autorise pas, c'est juste pour savoir : et si demain le Vatican veut financer une église, libre à lui, il y a pas de problème. La parole est à monsieur du Rhin. en revanche, le débat qu'on a sur cet article 25 illustre bien quand même les limites du texte, sur lequel on enfin travailler. La France qu'on a le plus entendu depuis qu'on a commencé à travailler hier, c'est la disposition vous présenter l'amendement l'article ne relève pas de l'objet du texte, mais l'objet du texte, c'est quoi la nature des débats qu'on a le caractère hétérogène, la confusion quelques qui préside à nos débats sur un nombre de sujets dont on sait, plus ils sont dedans dehors Cissé législatif réglementaire ou si ça relève de l'organisation de l'administration finit par poser un problème et au fur à mesure que nos débats progresse, on sent se déliter cette belle société de confiance qu'on nous proposait donc voilà, moi je suis entrée plutôt avec enthousiasme et envie dans dans l'étude de ce texte et un certain nombre de débats n'amène à considérer que finalement la montagne accouche d'une souris, c'est assez décevant et parfois même, comme sur cet article un peu dangereuse. La parole est à monsieur Loïc Hervé. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mais mes chers collègues, moi je crois que GIAT à cet amendement, mais j'ai voter sans aucune difficulté, car on est tous attachés évidemment principe de laïcité mais aussi au libre exercice des cultes, mais je me souviens quand même qu'il y a quelques mois, j'étais encore maire d'une commune en Haute-Savoie et qui avait un projet de ce type-là et que le maire que j'étais à l'époque il était fort dépourvu de n'avoir aucun aucune information de ne pouvoir en avoir aucune sur un projet de ce type-là, alors bien sûr le le l'amendement s'il est adopté, il sera applicable aux témoins de Jéhovah aux mormons ou, tout à tous ceux qui veulent construire des bâtiments parce que vous pourrez très fraudé des églises catholiques qui, on en construit plus beaucoup en France depuis quelques années, c'est ainsi, c'est ainsi, mais ça arrive et je crois pas que ce soit d'ailleurs, l'Église catholique qui se qui se mobiliseraient contre un quelles propositions il y a pas de régime d'autorisation, il y a pas de régime d'interdiction, la liberté du culte est consacré dans notre droit au plus au plus haut niveau et donc je pense que ce besoin de transparence proposée par notre collègue Hervé Maurey, est une bonne chose et donc je voterai sans aucun état d'âme. Bon, je n'ai plus de demandes de parole cette fois-ci c'est certain, donc je vais mettre aux voix l'amendement 21 rectifier bis, vous l'avez compris avec 2 avis défavorables qui vote pour.

il est adoptée après l'article 25 l'amendement 34 rectifier qu'inquiète même de remédier vous le présenter. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, l'article 38 de la Constitution dispose que la ratification d'une ordonnance doit résulter d'une disposition expresse, je vous propose de ratifier l'ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations qui attend depuis 3 ans, le 28 septembre 2016 j'ai rapporté le projet de loi de ratification devant la commission des lois du Sénat qui l'a adopté, la majorité de l'Assemblée nationale a préféré reprend le texte de mon rapport par amendement dans la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, malheureusement, le Conseil constitutionnel a écarté comme cavalier législatif dans cette loi, la ratification de l'ordonnance du 23 juillet 2015, ce n'est donc toujours pas fait depuis 3 ans malgré la volonté contraire de notre commission des lois et du parlement tout entier pour des simples raisons de procédure, c'est la raison pour laquelle je vous propose de ratifier cette ordonnance dans les termes mêmes de mon rapport, y compris en matière d'organismes faisant appel à la générosité publique votre commission des lois avait examiné avec la plus grande attention les dispositions de l'ordonnance relative aux organismes faisant appel à la générosité publique l'ordonnance les réformer dans le sens d'un allégement des contrôles auxquels ils sont soumis à la commission des lois n'avait pu accepter, en effet, d'une part, le nouveau dispositif, dépassé les limites de l'habilitation à légiférer par ordonnance consenti au gouvernement, d'autre part, l'ordonnance a procédé à un allégement important des contraintes imposées de ces organismes, l'allégement porte notamment sur la traçabilité des fonds collectés, il a donc paru à votre commission des lois de soulever des réserves alors que la loi de 1991 adoptée à la suite du scandale de l'ARC garantit une transparence financière indispensable, j'ai donc jugé et sur ce point, la commission des lois, m'a approuvé en septembre 2016 qu'une telle réforme ne s'imposait pas dans le monde où le vivant, l'opinion publique attend des autorités, avec raison, la transparence et le contrôle de telles opérations tant l'État que les donateurs doivent pouvoir exercer une vigilance par des moyens de contrôle suffisants, voilà pourquoi mon amendement rétablit le dispositif antérieur à l'ordonnance de 2015 sa modification ne peut avoir lieu sans un bilan complet de la loi de 1991 et seulement dans le cadre d'un texte spécifique permettant de mesurer l'opportunité d'un allégement aussi important des contrôles. Merci, quel est l'avis de la commission, même la rapporteur. Merci Monsieur le Président, la ratification repose sur le texte qui a été élaboré par la commission des lois du Sénat à la suite d'un travail approfondi qui a été menée sur le projet de loi de ratification de cette ordonnance amendement comprend également la suppression des dispositions excédent le Champ de l'habilitation et c'est donc un avis favorable qui a été donné par la commission spéciale. Monsieur le président, le le gouvernement considère que la ratification des ordonnances évoqués par Madame la sénatrice devrait trouver sa place dans une autre procédure dans ce texte, c'est pour cette raison, c'est un avis défavorable. La demande d'explication de vote donc un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui votent pour ce 34 et qui qu'inquiet. Merci qui vote contre qui s'abstient, il est manifestement adopté l'article 25 de supprimer l'article 26 2 amendements identiques de suppression discussion commune le 96 Madame Robert. merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, lors de l'examen de la loi Création Architecture et Patrimoine, et de son vote en 2016 nous avons voté un amendement qui permettait à l'État aux collectivités locales et à leur groupement d'expérimenter pendant 7 ans, un dispositif qui leur permettait de déroger à certaines normes, à condition qu'elles soient remplacées par des objectifs à atteindre, obligation de résultat en quelque sorte, lorsque la discussion est arrivée au Sénat puisque c'était à l'assemblée, nous y avons rajouté ici collectivement les organismes HLM, c'est une expérimentation qui était limité dans le temps et qui étaient bien encadrés aujourd'hui par ce parti qu'on nous propose sans aucun bilan sans aucun verrou en terme de durée en termes d'acteur ou même en terme de chambre dérogation de supprimer ce dispositif alors on voit bien que dans le cas des ordonnances et c'est plus une réforme des normes de construction qui va être en vigueur en 2 temps, mais quand même plus qu'une dérogation temporaire, on voit bien que les maîtres d'ouvrage en avait circonscrit note d'expérimentation à la sphère publique, elle est étendue à la sphère privée, en l'occurrence les promoteurs et puis le chant d'aller d'application, il est complètement illimités, donc ce n'est plus qu'on avait appelés nous au sein de la commission culture, mais que la ministre et l'ensemble du Sénat, le permis de faire, c'est-à-dire le droit d'expérimenter de désormais en quelque sorte, alors bien sûr c'est un outil de souplesse, on le voit bien. Mais je voudrais attirer votre attention mais, chers collègues, quid de la qualité architecturale, quid de l'innovation, une forme d'évaluation qui permettrait un moment notamment sur les questions énergétiques, de travailler et de progresser, on peut désormais, mais en même temps être attentifs à la qualité architecturale, on voit bien ce sera coûtera peut-être moins cher, ça ira plus vite, mais attention, alors en plus, moi je ne comprends pas, et je voudrais que le ministre réponde pourquoi le gouvernement se prive aujourd'hui d'un outil cet outil expérimental en fait qui permettait sans délai. Avec des solutions innovantes qui pouvaient être capitalisées et servir de base, peut-être à des modifications législatives ultérieures pourquoi aujourd'hui il se prive de cet outil, alors qu'on sait très bien que les ordonnances ne verront le jour qu'en 2020. Et que, on aurait pu la encourager vraiment, hé bien le recours aux permis d'innover ou de faire en facilitant la la dispute la mise en 9 du dispositif que nous avions ici collectivement, je dis bien collectivement voté alors effectivement, tous ces éléments nous conduisent à demander la suppression de cet article, merci. Merci, cher collègue pour le groupe CRC. Monsieur aux audiences. Je suis président, Monsieur le ministre, l'article 26 heures place concrètement une obligation de moyens pour une obligation de résultat ainsi plutôt que de respecter des normes, des listes de matériaux des princes et une construction, comme l'a dit ma collègue visant à protéger les bâtiments entre autres contre les incendies, le projet de loi instaure un permis déroger aux travailler sans filet, c'est le cirque les dérogations envisagées porteront sur la performance énergétique et environnementale, l'aération et la qualité de l'air, etc, mais aussi sur la santé et la sécurité des bâtiments et des personnes, ou encore la prévention des risques naturels et technologiques etc, comme le souligne l'avis du Conseil d'État cet article peut susciter une réserve alors qu'une expérimentation, on l'a dit, est en cours, qu'elle n'a Empruntis qu'elle n'a en pratique pas commencé à être mise en oeuvre et qu'elle a donc produit aucun résultat cet article sans bouclier que les règles de la construction dans la complexité, le nom peuvent effectivement interrogé ne sont là ne sont pas là que pour encadrer l'acte bâtir mais aussi pour garantir les occupants contre l'incendie, le résultat du respect de chaque norme conduit à ce que l'ouvrage doit être accessible aux personnes handicapées protéger contre un incendie, le tremblement terre etc, comment penser transiger avec la sécurité contre le risque d'incendie, par exemple, enfin, ce nouveau rapport aux normes de construction fondée sur l'atteinte d'un résultat conduira l'exigence d'une démonstration préalables et d'un contrôle atroce tuerie fait par un organisme impartial, la tâche des constructeurs ne sera en rien simplifié et la responsabilité prise par ces organismes de contrôle ne sera pas négligeable, loin s'en faut, le libre choix des moyens risquent ainsi de se payer en terme d'insécurité juridique Compte-tenu de la plus grande liberté qui sera donnée à l'organisme qui on appréciera le résultat, ce que nous vous demandons c'est comme ma collègue de supprimer cet article sur merci. Alors qu'est l'avis de la commission je rapporteur sur Sud, 2 amendements de suppression. Ces 2, ces 2 amendements proposent pour des raisons différentes, de revenir sur la position de la Commission spéciale en supprimant les habilitations portant sur les ordonnances relatives à ce que certains appellent le permis de faire en matière de construction, ça a été rappelé. La commission il y a défavorable. Et je rappelle que le dispositif que permet l'article 26 ne revienne à nos à abaisser le niveau d'exigence mais concerne uniquement les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre même but, voilà l'avis de la commission. Merci Monsieur le Président, l'article 88 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté, la liberté de la création à l'architecture et le Patrimoine ainsi que son décret d'application du 10 mai 2017 ont initié une démarche globale d'expérimentation pour la construction et l'architecture, force est de constater que leur mise en oeuvre est jugée trop lourde et délicate par la profession, si bien, c'est peut-être là le début d'un bilan Alistair malheureusement qu'aucune demande de dérogation n'a été déposée à ce jour, depuis la parution du décret de mai 2017, le présent permis de faire élargit le Champ d'application la dérogation, tout en veillant la simplicité du dispositif à sa rigueur au regard des objectifs de sécurité et d'environnement, comme l'a rappelé monsieur le rapporteur, le dispositif actuel présente plusieurs difficultés dans sa mise en oeuvre, la limitation du Champ d'application logement social et aux équipements publics, le faible nombre de normes concernés ou encore la lourdeur du système d'instruction et de contrôle, considérant que la loi du 7 juillet 2016 ne permet pas d'apporter les modifications souhaitées par voie réglementaire, le présent projet de loi prévoit que le gouvernement puisse prendre par voie d'ordonnance des mesures réglementaires qui autoriseront le maître d'ouvrage à déroger à certaines règles de construction, l'on abandonne, que l'on abandonnera nécessairement liées aux objectifs de qualité esthétique ou architectural que vous avez évoquées Madame Robert, par ailleurs, le projet de loi permet effectivement au gouvernement de réécrire directement par voie d'ordonnance, le livre 1er du code de la construction et l'habitation c'est pour ces raisons que le gouvernement est attaché au maintien de cet article.

Je voudrais quand même attirer l'attention sur la ligne A de de du de l'article 26 donc là. L'ordonnance fixe les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage de bâtiment peut être autorisé dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance etc donc on va avoir une réglementation intermédiaire dans un sur un problème aussi sensible que ça on attend même pas que l'ordonnance ratifiée

à ceux qui découleraient de l'application des règles ordinaires et qu'il pour que tout ce que ces moyens sont innovants, etc, franchement c'est c'est une précision extraordinaire. Je vous en prie. Je voudrais simplement dire que le permis de faire qu'on avait voté ici, ce n'est plus du tout celui-ci et j'aimerais bien qu'on n'usurpe pas ce nom parce que le certains architectes d'ailleurs s'en sont émus sur ce la la disposition de l'article présent ce n'est pas du tout le même esprit, nous, nous avions justement faire en sorte que soit une expérimentation encadré à la fois dans le temps et sur ces objets après le mystère, la culture a pris un décret, il manque un autre décret, on ne peut pas aujourd'hui, alors même que l'expérimentation n'est pas en cour, dire que c'est trop lourd et ça a pas été fait parce que, à mon avis, c'est un argument qui ne tient pas, vous savez tout à l'heure, nous avons un amendement de repli, ce que je vous proposerai monsieur Minister qu'on trouve un compromis, c'est-à-dire qu'un moment hé bien en termes de pouvoir réglementaire, on puisse du coup allégée mais garder l'expérimentation parce que c'est un outil qui peut se mettre en avant maintenant et qu'on est pas obligé l'2020 que la ratification effectivement mi-2020 pour les ordonnances et qu'on puisse un moment évalués évalués sur des process innovant, s'ils sont efficaces, voire même efficient aujourd'hui en matière de normes de construction et je trouve ça plutôt intéressant qu'on puisse s'engager sur une expérimentation. Pas d'autres demandes d'explications de vote, donc je vais mettre aux voix, ces 2 amendements de suppression 2 avis défavorables qui vote pour. qui vote pour. Il s'abstient, ils ne sont pas adoptées, l'amendement 18 rectifier Monsieur Detraigne. Amendement précision avis de la commission. c'est un avis défavorable, mais en fait, cet amendement propose de remplacer les termes règles de construction par norme de référence, actuellement utilisés par l'article 26 par les termes normes réglementaires sur le 1er point substituer au terme réglerait de construction, les termes normes réglementaires reviendrait à empêcher toute dérogation et nous en avons parlé une commission à une norme législative, le gouvernement peut déjà créé un régime dérogatoire aux normes réglementaires, il n'a pas besoin d'une habilitation adopté une ordonnance pour se faire, au demeurant le Champ normes auxquelles pourrait être dérogé sera défini en concertation avec les professionnels sur le second point, qu'elle, interrogé à ce sujet par votre rapporteur, moi-même, le gouvernement a précisé que les termes le terme norme de référence renverrait pour la plupart des cas à des normes de nature réglementaire n'est que par exception des normes professionnelles rendu d'application obligatoire par arrêté pourraient également être concernés, voilà l'avis de la commission. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, c'est le même avis et je rejoins monsieur le rapporteur, si c'est une précision l'est de taille, il y a et nous ne partageons pas ce qualitatif ce qualificatif là nous craignons même que le renvoi aux normes que vous proposez soit plus source de confusion de précision, nous rejoignons l'argument du rapporteur le il s'oppose à cela reste 11 ans au dispositif que nous avons proposé, si vous voulez bien nous craignons que ce que vous proposez ne soit pas aussi opérant en quelque sorte. Retirer 2 amendements dans l'objet d'une discussion commune le 153 qui le présente monsieur Ouzoulias. un un amendement de de repli mon amendement de repli incendie ou de sauvegarde les les fédérations nationales des sapeurs-pompiers, l'Association des brûlés de France, la Fédération française des métiers de l'incendie que nous avons tous entendu nous disent passer d'une logique de moyens une logique d'objectifs, ça reviendrait à jouer aux apprentis sorciers avec la sécurité des bâtiments et la vie de nos compatriotes, il nous appelle et nous rappelle et je le cite : c'est en souvenir de ces centaines de morts dans les incendies que les énorme se sont renforcés au fil des années cette réglementation précise a fait ses preuves, le nombre de victimes par incendie a été divisé par 2 en 30 ans si près de 600 victimes sont toujours à déplorer chaque année, c'est essentiellement dans les habitations anciennes pour lesquelles la réglementation et la moins exigeante avec l'article 26 l'atteinte d'un objectif en terme de sécurité ne pourra être vérifié qu'en cas de sinistre, on l'a dit, je le répète postériori et après l'accident, il est donc dangereuses de procéder de la sorte en matière de sécurité le tragique incendie de la tour Graine file à Londres en juin 2017 nous rappelle que le laxisme réglementaire un coût en vies humaines, c'est pourquoi les auteurs cet amendement, souhaite que les exigences fondamentales concernant la résistance mécanique, la stabilité et la sécurité en cas d'incendie soient exclus des possibles dérogations merci.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues par cet amendement, il s'agit de sécuriser et de renforcer le processus d'examen de validation des autorisations de dérogations prévues par le présent article qui vont à la charge de la preuve de la nature équivalente au cadres prescripteurs Yves de la dérogation mises en Oeuvres revient au maître d'ouvrage, mais l'État doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour contrôler ses preuves avant la délivrance d'autorisations d'urbanisme et après l'achèvement du bâtiment.

les préoccupations qu'il exprimait selon bien évidemment légitime et le permis de faire ne saurait un aucun cas conduire un abaissement des exigences des règles en matière de sécurité des personnes et débile, nous sommes je crois là-dessus tous d'accord, le gouvernement a confirmé et et tout à l'heure monsieur le ministre, j'espère, nous le confirmera, nous a confirmé à plusieurs reprises au cours des débats parlementaires, que ce dispositif ne reviendrait pas à jouer aux apprentis sorciers pour reprendre les termes de l'objet de la même demande, il s'agit simplement d'insister sur les objectifs à atteindre, plutôt que les moyens à mettre en oeuvre, autrement dit de s'assurer, dans l'attente du résultat, le ministre c'est un engagé devant notre commission spéciale à consulter les professionnels et en particulier ceux des métiers, samedi, vous l'avez rappelé mes chers collègues, c'est ce qui sont, qui nous ont alerté à plusieurs reprises, voilà pour l'amendement 5 53 moins cher collègue Claude Kern sur la manne demande 35, ils entendent dans le cadre de la seconde ordonnance prévues par cet article, mettre en place un contrôle de l'attente des résultats. Avant avant. La délivrance de l'autorisation d'urbanisme, ce contrôle révélerait sur croit l'objet de l'amendement de l'État, l'État aurait la responsabilité de ce contrôle et un sorte de le faire sur le fond, il est déjà prévu que la preuve de l'atteinte des résultats devraient être apportées en amont du document d'urbanisme et comme évoqué précédemment, les dispositions relatives au contrôle des constructions non pas vocation à être notifié à la baisse par l'ordonnance sur la forme, a toujours sur certains amendements là à l'joute à une modalité de contrôle supplémentaires de l'attente des résultats cet amendement me semble Anne tâcher d'inconstitutionnalité. Car il est temps de ce fait le charme de l'habilitation donnée au gouvernement. Pour tout ceci, la commission Greiner a émis un avis défavorable pour les 2 amendements. Mais je vais simplement Monsieur le ministre, à toutes fins utiles, pouvez-vous demain et si notre haute assemblée nous rassurer, parce que c'est important, c'est l'objet des 2 amendements nous rassurer sur le fait que d'une part, vous avez pris qui a été pris par par le le ministre Darmanin lorsque nous l'avons reçu à une commission spéciale le rassurer sur le fait que d'une part, et il n'y aura aucun abaissement du niveau d'exigence d'énormes. D'autre part, les ordonnances seront rédigés et j'insiste sur ce point, seront rédigés en concertation avec la simple des professionnels concernés. Graham des petites entreprises du bâtiment de la promotion immobilière : les professionnels de la sécurité samedi et je pense à nos différences, à 10 qu'il y a dans les départements et également aussi et les représentants des compagnies d'assurances et avec toutes ces garanties, Monsieur le Ministre, donc, et après avoir. Auditionné entendu sollicités donc la commission a émis un avis défavorable. Alors monsieur Méliès l'avis du gouvernement sur ces 2 amendements. Merci monsieur le président, si vous me permettez, je commencerai par l'amendement numéro 35 du sénateur Kern, pour dire tout simplement que je partage les arguments du rapporteur et c'est une demande de retrait ou un avis défavorable pour les mêmes raisons compte concernant l'amendement numéro 153 présenté par le groupe SRC simplement rappeler d'abord. Que la possibilité de satisfaire aux exigences de sécurité incendie par des solutions d'effet équivalent est déjà en partie rendue possible par l'article 105 de l'arrêté de 1986 sur les bâtiments d'habitation, dire que l'habilitation complète ce dispositif en généralisant mais dans la mesure où l'écriture proposée n'autorise en aucun cas et ça répond à la une des interrogations du rapporteur à minorer les objectifs à atteindre, notamment sur l'essentiel de la sécurité des biens et des personnes, il n'y a pas de raison d'exclure ce thème du Champ d'application de la mesure, les acteurs, professionnels de la sécurité incendie, les compagnies d'assurance et les associations des brûlés de France ont été reçus la semaine dernière par le ministère de la cohésion des territoires, de même que parle pas cabinet du ministre de l'action et des Comptes publics engagement a été pris et il a été convenu avec eux de travailler train d'engager, pardon, un travail de coproduction pour veiller à la production de textes donnant toutes les garanties de sécurité et donc, pour répondre aux 2 interpellations du rapporteur aucune volonté bien évidemment d'abaisser les objectifs et les normes en matière de sécurité et engagement de travailler avec tous les acteurs concernés pour que le texte réponde à cet objectif, donc l'avis défavorable à moins que cet amendement ça retirer.

Oui, merci Monsieur le Président, alors avec les explications mais malgré mon étonnement de soi-disant de l'anticonstitutionnalité de cet amendement, qui est ces derniers temps, trop souvent mise en avant, je vais quand même retiré cet amendement. L'amendement retiré et nous avons ensuite 3 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune le 9 rectifier monsieur Kern. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la dérogation pour les maîtres d'ouvrage du bâtiment à certaines règles de construction se réserve vise à simplifier les démarches des entrepreneurs meurent pas moins qu'il faut impérativement encadrer ce dispositif notamment pour des raisons de responsabilité et d'assurance à travers cet amendement, nous voulons permettre à une instance collégiale de s'assurer la façon dont il pourrait être dérogé à ces règles. Je vous remercie pour l'amendement 126 madame Préville. cet amendement permettrait à une instance collégiale de s'assurer de la façon dont il pourrait être dérogé à ces règles n'étant pas rassurés par ailleurs, il me semble nécessaire, voire indispensable qu'une instance technique composé de professionnels compétents puissent être mises en place pour s'assurer de l'effectivité de la mise en oeuvre de cette disposition, merci.

quand même significative d'instaurer une autorisation pour les maîtres d'ouvrage à déroger à certaines règles, mais il faut le sécuriser. Alors quelle est la commission sur ces 3 amendements, monsieur le rapporteur.

aux préoccupations des auteurs de l'amendement en exigeant que l'attente des résultats soient évalués dans un cadre M. partial et en conformité le code des assurances, et ce pour la première, comme pour la seconde ordonnance surtout et combien de noter que le régime dérogatoire considéré comme particulièrement lourd mis en place dans le car, dans la loi de 2009 16 E relative à la liberté de la création à l'architecture et au Patrimoine, ne prévoit pas le passage par une instance collégiale, dans la mesure où le dispositif de l'article 26 ne veut ne veut plus de se se veut plus efficace que celui prévu par la loi, il serait probablement mal visé de prévoir un processus encore plus lourd, au demeurant, les dispositions relatives au contrôle des constructions n'ont pas vocation à être modifié à la baisse par l'ordonnance qu'il s'agisse du contrôle du respect des règles de construction établi sur la base de l'article L. 1 du code de la construction et de l'habitation ou des commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, la commission a donc émis un avis défavorable à ces amendements, cela étant dit, monsieur le ministre, nous sommes tout ouïe pour vous écouter, sur ce point particulier. particulier. Je ministre vous avez la parole pour nous donner l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président, l'Europe vous dire monsieur le rapporteur, que laisse de l'espoir, je n'aurais pas beaucoup, a ajouté aux arguments qui sont les siens pour demander le rejet de ces 3 amendements le gouvernement partage totalement les propos du rapporteur, et je précise simplement mais cela a été dit par le rapporteur de la même manière que la façon dans l'art. Si les telle qu'il a été amendé telle qu'il a évolué dans le débat nous semble plus efficace pour de disposer d'un système qui soit plus opérant plus souple aussi que celui de l'établissement d'une instance collégiale nationale et pour vous garantir donc les ordonnances prises sur le fondement de cet article détailleront les conditions d'expertise et d'impartialité des organismes en charge d'attester l'équivalence des résultats qu'il n'y aura pas de révision à la baisse des objectifs tels que vous l'avez mentionné et ce sera certainement plus simple que par la mise en place d'une instance nouvelle donc, la vie aussi défavorable. Alors 2 avis défavorables, ce que. Pas de demandes d'explications de vote, je peux mettre aux voix, ces amendements qui vote pour. Qui vote contre.

Bien, merci Monsieur le président Monsieur ministre, bon, vous avez compris que cet amendement est un amendement de repli que par cet amendement, on vous demande de garder l'expérimentation telle qu'elle a été voté, ici lors de la loi crée création Architecture et Patrimoine, je voudrais vraiment rajouter que un décret sorti le 2ème d'un décret n'est pas sorti et donc ou bloquent l'expérimentation, je pense que le pouvoir réglementaire pourrait

puisque l'Artic 6 ça été maintenu de pouvoir quand même garder tout de suite l'expérimentation et du coût de la mettre en oeuvre de type de faire une évaluation et d'en tirer un bilan pour qu'on puisse légiférer un peu plus intelligemment merci. Quel est l'avis de la commission sur l'emportera. ça été rappelé cet amendement propose de supprimer l'habilitation du gouvernement a supprimer dans le cas dans la première ordonnance le dispositif expérimental dérogatoire mis en place par la loi de 2009 16 E relative à la liberté de la création, l'architecture et du Patrimoine, dans la mesure où l'article 26, poursuit la même logique que cette expérimentation, mais selon des modalités plus souple et j'en application plus large, on peine à distinguer l'intérêt qu'il y aurait à maintenir un régime dérogatoire qui n'auraient plus lieu d'être, comme l'ont montré les travaux préparatoires le régime mis en place par cette loi apparaît trop lourd et s'enchaînent : l'application semble trop restreint, ce qui explique l'absence de mise en oeuvre de ce dispositif, à ce jour, la commission a donné un avis défavorable sur cet amendement. Je le ministre du gouvernement, s'il-vous-plaît. Merci Monsieur le Président, et il y a un constat, une divergence d'appréciation sur les modalités et l'efficacité des modalités de de mise en oeuvre de la loi de juillet 2016 entre les signataires de l'amendement présenté par Madame Robert et le gouvernement, c'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à l'amendement de suppression tout à l'heure et que, par cohérence aussi sommes opposés au gouvernement est défavorable à l'amendement de repli vous propose à cet instant. 2 avis défavorables. Demande explication de vote qui vote pour. Qui vote contre. Il n'est pas adopté l'amendement numéro 50 du gouvernement Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, ce que nous proposons avec cet article et cela a été évoqué est un changement de paradigme pour les maîtres d'ouvrage, les concepteurs, les constructeurs et les contrôleurs bâtiment ce changement s'appuie sur l'idée que les constructeurs de bâtiments sont des professionnels compétents et responsables innovant aussi prêt à proposer une nouvelle manière de construire, pourvu qu'on leur donne un cadre le cas doit être ouvert mais précis, les débats autour de la sécurité incendie, notamment, ont souligné tout l'enjeu qu'il y avait à définir précisément l'étendue des dérogations qui pourront être accordées et les limites de ce même dérogation les ordonnances qui seront prises suite au vote de la loi devront par ailleurs encadrer les organismes qui seront chargés de la preuve de l'attente des résultats, le temps pour réaliser les ordonnances de réécriture du code éthique c'est 18 mois dans le projet initial, la commission spéciale soucieuse d'une mise en oeuvre à pied d'cette disposition a je crois voulu bien faire en ramenant ce délai à 12 mois si nous pouvons vouloir conduire avec l'ensemble des acteurs une concertation de qualité, il ne faut cependant compter plus 12 mois puisqu'il faut s'y ajoute un temps de consultation obligatoire aussi par cet amendement, le gouvernement sollicite le Sénat pour établir le délai de 18 mois qui nous sera octroyée pour permettre l'écriture désordonnée. Alors Monsieur rapporteur La Commission entend-elle du gouvernement. Alors Monsieur le ministre, au risque de vous décevoir, donc, la commission de la donner un avis défavorable puisque tout simplement nous souhaitons conserver le délai de 12 mois, je rappellerai simplement que nous avons adopté une commission ce délai parce que

travailler avec les professionnels, c'était le cas pour la question de la prévention incendie Sécurité pour les autres domaines vous vous-même, monsieur le rapporteur, ainsi que les membres de la commission spéciale avait exprimé à plusieurs reprises particulier, une consultation pardon qui soit particulièrement fourni et dense pour que les ordonnances prises puissent être de bonne qualité, efficace et apporte la souplesse que les uns et les autres espèrent ce dispositif-là au risque d'inciter à la la préparation des ordonnances est accompagné d'un délai de consultation obligatoire et le temps qu'il resterait sur 12 mois, souhaite rassembler, décidé de maintenir les dispositions adoptées en commission spéciale serait un temps à nos yeux trop court pour pouvoir mener à bien les consultations avec l'importance que nous souhaitons leur donner l'importance que vous appelez de de vos voeux, donc c'est vraiment avec ce souci d'efficacité et en renvoyant l'évaluation évidemment des ordonnances au au débat de ratification, que je me permets d'insister pour que vous puissiez c'est possible reconsidérer votre avis afin que nous puissions disposer de de 18 mois. Je ne sais pas si je dois réinterroger la commission non je n'ai pas nécessaire, elle maintient son avis défavorable, je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 50 du gouvernement : avis défavorable de la commission qui vote pour.

Je suis président, mes chers collègues, l'article 26 a pour objet de permettre d'identifier parmi les normes réglementaires de construction, celle qui pourraient être transformée en obligation de résultat, il s'agit non pas de supprimer des normes réglementaires existantes, mais de créer en parallèle, en quelque sorte de nouvelles règles, avec un fonctionnement différent, cette initiative ne doit pas conduire à assimiler les organismes commandité par le maître d'ouvrage pour instruire le dossier dérogation à l'instance qui validera la proposition dérogatoire or toute initiative dérogatoire doit être examiné et validé par une commission expert impartial, ce qui ne peut être atteint que par le biais d'une commission nationale d'évaluation, c'est l'objet de cette. Je rapporteur de l'avis de la commission s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président, moins chers collègues, c'est quasiment le même amendement que notre collègue tout à l'heure Claude. Ceci dit, un but de s'assurer du caractère notre impartial de l'évaluation de la TNT, résultat : cet amendement propose qu'elle soit effectué par une commission nationale d'évaluation, ce que vous ne de rappeler sous la responsabilité de l'état de la composition est fixée par décret le caractère impartial de l'évaluation est déjà prévue par l'alinéa 8 et prévoir une commission nationale d'évaluation pour le régime dérogatoire transitoire, comme pour le nouveau régime de droit commun mis en place par la seconde ordonnance paraît disproportionnée, je suis désolé, mon cher collègue, donc il est proposé un avis défavorable. Le ministre. 2ème un avis défavorable, Monsieur le Président, pour les raisons évoquées par le rapporteur et en écho au débat que nous avons eue sur la Série 3 amendements parce qu'identique tout à l'heure.

Merci qui vote contre qui s'abstient, il est adopté l'article 26 Bis supprimer le 26 terre je suis saisi l'amendement 51 du gouvernement Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, il s'agit d'un amendement de suppression puisque cette disposition qui pouvait présenter un aspect séduisant premières analyses soulève cependant plusieurs difficultés présente tout d'abord un intérêt limité dès lors qu'elle est redondante avec le dispositif d'autorisation environnementale qui a déjà permis d'instaurer un interlocuteur unique pour l'ensemble des procédures, or celles relevant du droit de l'urbanisme, plus de 12 autorisation Amérique sont ainsi désormais incluse dans l'autorisation environnementale, il y a un amendement, vous sera d'ailleurs proposé plus tard pour ratifier l'ordonnance et ancrées l'autorisation environnementale elle conduirait ainsi à inclure uniquement 2 autorisations d'urbanisme délivrés par l'État, c'est l'approuvant le projet d'ouvrage électriques et celle qui relève également d'État pour le bâtiment, les bâtiments publics et l'énergie, or cette intégration des autorisations d'urbanisme a déjà été expérimentée dans le cas de la procédure autorisation unique en 2015, 2016, la mission du port qui a tiré le bilan d'expérimentation préconisait d'abandonner cette intégration en raison des grandes divergences existent entre les 2 procédures qui repose sur des corpus juridique très différents et c'est donc en toute connaissance de cause que l'intégration de l'autorisation d'urbanisme dans l'autorisation environnementale a été abandonnée et que la solution retenue pour le cas particulier des éoliennes terrestres a été la suppression de l'autorisation d'urbanisme, compte tenu de ces éléments, il est proposé la suppression de cet article, la disposition dont nous vous proposons la suppression n'aurait donc vocation à modifier le droit existant que dans les cas très résiduel où subsiste un permis état donc pour le méthaniseur les centrales solaires et les projets situés dans une commune au règlement national d'urbanisme ou dans le cadre d'une opération d'intérêt national et pour ces derniers

l'avis de la commission mais défavorable. Monsieur le ministre, vous nous proposez, si un amendement de suppression, alors qu'il a été sous-amendé à nationale. Ce faisant, non seulement il revient sur sur sur sa position, je parle, Monsieur le Ministre, mais aussi et surtout, il revient celle sur celle de la commission spéciale, je rappelle que c'est le s'il avait donc cet article et et rejoignent le dispositif de l'article 7 de la proposition de loi de l'eau collègue François Calvet Marc Denis sur la stabilisation du droit de l'urbanisme.

Qui vote pour merci qui votre contre qui s'abstient. Il est adopté l'article 27 est réservé à l'article 28, une demande de paroles de Madame Préville. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'expérimentation de nouveaux modes de gouvernance ou de dérogations aux règles de terre territorialité pour des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant déjà opté pour les formes de rapprochement de regroupement ou de fusion prévue par la loi du 22 juillet 2013 relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, je m'interroge sur la méthode qui est à nouveau un recours aux ordonnances, le Parlement, à mon avis, devrait pouvoir accompagner étudier les modalités d'organisation de l'enseignement supérieur, avant d'être mis devant le fait accompli par des ordonnances d'autre part, je m'interroge : n'y a-t-il pas un risque de voir soit émerger ou se renforcer une véritable université à 2 vitesses qui accentuerait les inégalités territoriales, on peut facilement imaginer la création de grands pôles, laissant à la marge les petits établissements qui à terme n'auront que peu de moyens pour assumer leur mission, donc, Monsieur le ministre, j'attends vos réponses merci. Alors quelle est la vie. Non, c'était une prise de parole, j'ai un peu vite, on est sur 154 maintenant, qui sera présenté par monsieur Ouzoulias monsieur Ouzoulias rapporteur je vous ai fait vous levez trop vite. Monsieur le président, Monsieur le ministre ma collègue vient de le dire, il s'agit de de nouveaux de de permettent par les ordonnances des expérimentations lourdes puisqu'elle concerne la fusion des établissements dense donc, enseignement supérieur et on a le sentiment que l'objectif chez générale et de répondre aujourd'hui un mot d'ordre qui est partagée par tout le monde, plus c'est gros, plus c'est beau

prendre par la plus de fusion qu'une, on parlera peut-être de diffusion et le seul argument qui nous est donné pour la constitution de ce mastodonte, c'est le critère de taille je trouve vraiment triste dans notre pays, de constater que le classement de Shanghai, c'est tellement inscrit aujourd'hui dans nos cerveaux, qu'il est devenu l'unique principe organisateur de l'enseignement supérieur français avant de poursuivre dans cette marche forcée vers la fusion, il eut été de bonne politique, Monsieur le Ministre d'évaluer ce qui a déjà été réalisé en la matière et je pense notamment aux communes, les communautés d'universités et d'établissements qui sont aujourd'hui un échec patent et dénoncée par tout le monde cet article tels que vous nous présentez prévoit la la remise d'un rapport qui nous présentera au Parlement un 1er bilan de ces expérimentations, monsieur le ministre, je vous propose une autre méthode, vous nous présentez d'abord un bilan de toutes les expérimentations qui ont été engagés et ensuite seulement nous discuterons de vos propositions législatives pour corriger les dispositifs antérieurs, merci.

de s'y opposer, donc c'est un avis défavorable. j'espère en tout cas de de répondre à certaines interrogations de Madame très vite, l'expérimentation de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement est attendue par nombre d'établissements d'enseignement supérieur et force est de constater que les formes de regroupement de regroupements qui ont été mises en place par la loi du 22 juillet 2013 se rebelle d'aujourd'hui insuffisante pour permettre aux établissements de mener à bien leur projet qui s'il s'inscrit notamment dans le cas des investissements d'avenir porte également sur les formes de regroupement, qui ne sont actuellement pas prévue par la loi, c'est la raison pour laquelle, afin d'éviter de figer le nouveau mode d'organisation, l'expérimentation nous apparaît comme le meilleur moyen de permettre une évolution, c'est la raison pour laquelle nous sommes attachés au maintien de cet article. Alors 2 avis défavorables. Je vous en prie mis volontiers chers collègues. se trompent pas travailler comme ça on peut pas accumuler expérimentation sur expérimentation sans un moment donné, devant le Parlement, essayer de faire un bilan de ce qui a été fait, puisqu'ce qui ne fonctionne pas vous engager des nouvelles exportations sur des bases qui sont très similaires à celles qui ont déjà échoué le résultat, je le connais, je peux vous le donner, donc un moment donné, il faut arrêter, il faut raison garder et reprendre tout le dossier pour l'analyser de façon raisonnable. D'autres demandes d'explications de vote sur cet amendement, je n'en vois pas gel maison voilà 154 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre. Il n'est pas adopté l'amendement 52 maintenant du gouvernement Monsieur le Ministre. monsieur le président, c'est la même logique, un amendement précédemment présenté les les délais octroyée par le Parlement au gouvernement pour prendre l'ordonnance d'application de l'article 58 ont été ramenés à 6 mois avec les délais de consultation obligatoire et la volonté de concertation, c'est encore plus compliqué que quand la commission spéciale ramène le délai de 18 à 12 mois donc c'est un amendement pour que ce délai de un an, soit rétablie. Alors l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais nous souhaitons raccourcir les délais, donc je maintiens mon avis nous maintenons je parle au nom de la commission spéciale notre délai à 6 mois avis défavorable, donc c'est votre proposition. Avis défavorable je mais on voit l'amendement 52 qui vote pour.

Merci président, Monsieur le Ministre, Michel collègues alors cet amendement a pour objet d'offrir aux établissements publics d'enseignement supérieur dans les projets de coopération de coordination sont matures, les moyens de se structurer, de se regrouper sur le temps long, ce dispositif ôte la possibilité pour les établissements de renforcer leur intégration pouvant aller jusqu'à la constitution d'un seul établissement alors que de nombreux établissements regroupement se positionne pour répondre aux appels projet d'initiative d'excellence dans le cas du pays il y a, il y a un risque que certains établissements se retrouvent en période probatoire du fait d'un mode de gouvernement passé intégrative ou du fait d'un cadre légal adapté, si ce n'est instable, il y a six logique dans le la logique d'un texte fondé sur la confiance d'offrir aux établissements publics d'enseignement supérieur, le meilleur cadre légal,

des présidents de la conférence du présent université et ça serait également un comble dans la mesure où l'intitulé l'intitulé du projet de loi que le gouvernement ne fasse pas confiance aux établissements et à la communauté universitaire dans son ensemble. Quel avis de la commission sera porteur. Merci Monsieur le Président, cet amendement propose de créer directement et immédiatement dans la loi, sans passer par une ordonnance ni par une expérimentation un cadre dérogatoire pour le groupement d'établissement de la Seine-et-Marne supérieurs. Je partage l'idée et je crois que là ça ne la commission partager l'idée de permettre aux établissements engagés dans les programmes d'investissements d'avenir de mener rapidement à bien de leur projet et c'est la raison pour laquelle notre commission spéciale a réduit le délai d'habilitation qui durant à l'article 28 de à 6 mois, néanmoins, il me semble que cet amendement propose de créer un cadre dérogatoire particulièrement vaste sans justifier précisément les besoins auxquels il entend répondre il me semble donc il existe un risque de voir se créer autant de statut que de regroupements 5 que ces statuts réponde réellement aux besoins des établissements. C'est donc avec une certaine prudence, voire beaucoup de sagesse. Que la commission n'a donné un avis défavorable. merci Monsieur Président pour la, pour la même raison, le gouvernement, un avis défavorable, quand bien même la commission spéciale avec sagesse aussi si, si, vous le savez mais quand bien même la commission spéciale et réduit les délais pour rédiger l'ordonnance qui est évoqué dans cet article, nous ne pouvons souscrire à la démarche proposée par le sénateur Grosperrin, donc c'est un avis défavorable. Ce Grosperrin, vous avez la parole. Merci président alors j'entends bien mais rendent ce modèle expérimental au niveau de la loi, expose l'ensemble des sites à l'issue de l'expérimentation et ça risque de faire disparaître tous les établissements créés en vertu de ce modèle, sans exception, donc c'est plus sécurisant de considérer l'expérimentation plus sur le plan réglementaire que sur le domaine législatif. Mattel, l'amendement oui, donc je vais le mettre aux voix des demandes d'explications de vote, je n'en vois pas donc le 129 rectifier 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre. Ben écoutez il est adopté. Il est adopté. à l'article 29, une demande de paroles de Madame Élisabeth Lamure tout d'abord. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous arrivons au chapitre qui s'intitule des règles plus simples pour le public, or ce titre prometteur risque de décevoir les entreprises, en effet, à part 2 articles qui propose de revenir sur des sur-transpositions de normes européennes ce chapitre ne comprend pas grand-chose de nature à simplifier la vie des entreprises, nous aurions donc pu aller plus loin avec plusieurs de mes collègues, j'ai déposé à cet effet, un amendement pour confier à un organe ad-hoc, le soin de simplifier et améliorer le droit pour les entreprises notamment en traitant les problématiques de sur-transpositions cet organe ferait le pendant, au Conseil national d'évaluation des normes, créé en 2013 sur une initiative parlementaire, est chargée du contrôle et de l'évacuation de l'évaluation des normes applicables aux collectivités locales en nous déplaçant dans plusieurs pays voisins, avec mes collègues de la délégation aux entreprises, nous avons observé que de tels organismes ont déjà été mises en place au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne je l'ai indiqué hier dans la discussion, l'action du NK est en Allemagne, a notamment permis d'alléger la charge administrative dans ce pays de 14 milliards d'euros en 5 ans mon amendement qui reprenait la proposition de loi que nous avons déposée en septembre avec Olivier Cadic, avait pour objet de réactiver le Conseil de la simplification pour les entreprises qui a existé de 2014 à 2017 mais en renouvelant ses missions et sa composition, il serait ainsi chargé de contre-expertise et les études d'impact produite par l'administration et de proposer des simplification du droit en vigueur, malheureusement, cet amendement a été déclaré il recevables en application de l'article 40 de la Constitution, au motif que l'émission de ce conseil serait trop large pour être absorbés à moyens constants, par les services du 1er ministre pourtant ces services, assurait le secrétariat du Conseil de la simplification entre 2014 et 2017 je regrette donc que le débat ne puisse avoir lieu sur cette proposition d'autant plus que lors de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, la députée Alice Toorop avait également déposé un amendement proposant la création d'un conseil d'amélioration du droit pour les entreprises qui a pu lui être discuté en séance, je regrette, donc il y a en quelque sorte 2 poids 2 mesures. Merci, la parole est à même, Sophie Calle polio. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, messieurs dames les rapports. Les rapporteurs cet article 29 rend possible l'expérimentation du relayent c'est ce que avait souhaité le précédent gouvernement concernant le répit des aidants, donc je salue la mise en place expérimentale de ce dispositif qui est attendue par de nombreux acteurs de l'autonomie, je m'étonne qu'il trouve sa place dans dans ce texte, parce qu'il y avait d'autres mesures, bien plus, il a la confiance de nos concitoyens dans leur administration, qui n'ont pas pu figurer mais passons alors à la première lecture de ce texte était un petit peu inquiète parce que l'article 29, proposer un cadre juridique dérogatoire visant à donner au dispositif toute la souplesse permise par le droit européen mais sans présenter un certain nombre de garanties ni pour les professionnels, ni pour les personnes aidés, quelle protection alors pour les salariés de l'aide à domicile, aucune, d'autant que personne ici n'ignore que la branche de l'aide et des services à la personne connaît un taux d'accident du travail 3 fois supérieur à la moyenne est en progression de 45 pourcent sur ces 10 dernières années, je tiens donc à saluer le travail de notre rapporteur Madame Gruny qui a permis le retour du cadre sécurisé de l'application de la convention collective du particulier employeur parce que je crois à l'intérêt de ce dispositif modifié donc Jean soutiendrait l'adoption je souhaiterais obtenir quelques précisions bien commis en exergue par votre rapport ma chers collègues, ma chère madame, rapporteur, quid des dispositions relatives à la formation des baluchons honneur, c'est-à-dire des professionnels leur formation initiale comme continue est une exigence qui devrait être sanctuarisée enfin combien d'expérimentation pourront être envisagées sur nos territoires, quels seront les modalités d'évaluation de ces expérimentations, si ce n'est l'évaluation comptable de la CNSA, monsieur le ministre, les acteurs locaux, plus que jamais mobilisés sur le grand chantier de la perte d'autonomie, attendent des réponses sur ces questions, je vous remercie. Voilà, nous allons maintenant pouvoir passer à l'examen de l'amendement 155 rectifier qui le présente.

on on a des éléments de réponse, si vous me permettez, en en un temps très court, j'explique pourquoi ça vient d'être dit, on a eu des travaux de l'Assemblée, on a pu regarder ça a été dit, là, on aurait des salariés qui ne serait plus soumis aux stipulations relative au régime d'équivalence, temps de pause durée maximum, quotidienne, hebdomadaire travaille aussi de nuit, la durée minimale de repos quotidien est prévue par les conventions, des accords collectifs applicable aux établissements et services qui les emploie, donc ce qui nous anime, si les réponses nous sont données, nous retirons cet amendement à partir du monde de Lindsay, élément de garantie, il s'agit pas de débattre de cette solution de répit pour les pour les aidants familiaux, c'est pas le sujet, c'est l'ambiguïté, un peu d'ailleurs de cette partie du texte, il s'agit pas discuter de cette cette solution là, c'est de savoir quelles garanties y a ça a été dit, je rappelle le chiffre quand même dans la branche de l'aide des services à la personne, c'est là, on connaît un taux d'accident du travail 3 fois supérieur à la moyenne. 94,6 accidents du travail pour 1000 salariés sans progression de 45 pourcent ces 10 dernières années, donc voilà, si nous avons ces réponses-là, donc on peut trouver cette souplesse ici à travers la prise de parole qui a été fait, présent à un moment, si nous avons ces éléments-là nous retirons notre amendement.

comme vous bien entendu monsieur bien étonné trouvé cet article concernant l'aide au Proche-Orient et dans des personnes dépendantes dans un texte donc dont l'objet est toute autre, y compris le titre de la section la section c'est pas moi qui qui alors je rappelle par ailleurs que le Sénat a supprimé en 2015, un article similaire qui était proposé dans le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement nos rapporteur Georges Abkhazie et Gérard Roche avait à l'époque, considéré que l'expérimentation proposée n'était pas viable, faute notamment de financement parce qu'on va pas se voiler la face, le sujet, il il faut croire que le raisonnement de nos collègues avaient convaincu le gouvernement et la majorité des députés de l'époque, puisque l'article en question n'avait pas été réintroduit réintroduit dans la suite de la navette les réserves exprimées en 2015 sont toujours d'actualité et notre rapport exprime notre scepticisme face à cette expérimentation, toutefois, la commission spéciale a souhaité lui laisser une chance afin de pouvoir tirer un bilan, nous avons ensuite améliorer le texte proposé en prévoyant l'application de la convention collective du particulier employeur et en prévoyant une évaluation par la CNSA. on a, on a essayé d'améliorer un peu d'encadrer, moi j'entends bien les les difficultés il y a beaucoup de questions qui se posent, parce que justement on change aussi de conventions collectives

donc on s'est dit que supprimer complètement c'était certainement gênant voilà on espère que le gouvernement entendra nos nos diverses, inquiétude et de nous accompagner, nous nous permettre d'accompagner aussi cette expérimentation, voilà ce que je voulais vous dire donc, pour nous, forcément un avis défavorable à votre amendement. Merci monsieur le ministre, pour le gouvernement, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président Madame Attali pour lui en tout à l'heure, a dit l'intérêt qu'il y avait à ce dispositif notamment pour soulager les aidants, et leur donner des solutions qui sont très tendues depuis longtemps, cette disposition avait été introduite dans le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, mais elle avait été retiré en première lecture, puisque le rapport annexé de la loi renvoyé une études préalables et l'organisation d'une concertation et se renvoient à l'étude, qui avait justifié que cet article ne soit pas réintégré dans la navette, le gouvernement précédent a confié à Joëlle Huillier, député de l'Isère, jusqu'en 2017 émissions relatives aux conditions de mise en grève du relais agent France et ce rapport a été rendu en février 2017, soulignant à nouveau l'intérêt du dispositif pour les aidants, et les personnes aidées recommandant la mise en date d'une expérimentation, c'est pour ces raisons que le gouvernement ne souhaite pas la suppression de l'amendement. La commission spéciale introduit un certain nombre de dispositions et notamment la question de la accord la convention collective, nous souhaitons aussi mettre à profit la période d'expérimentation qui sera borné par une forme de clause de revoyure pour bien vérifier justement pour les belges sonneurs, pour reprendre l'expression pour l'ensemble des personnels concernés, qu'il n'y a pas d'effet de bas qu'on puisse, à l'occasion de la clause de revoyure et de l'éventuelle généralisation de cette expérimentation que nous souhaitons, sur le fond, corriger d'éventuelles c'était de bord et garantir la sécurité juridique que vous appelez de vos voeux, nous avons aussi comme projet du fait d'expérimentation, d'ouvrir les concertations nécessaires avec les conseils départementaux qui sont en première ligne sur la question de l'accompagnement des familles et des personnes qui sont sujettes à dépendance de manière à déterminer dans le cadre de l'habilitation à déterminer comment et dans quel volume l'expérience l'expérimentation pourrait être menée à la fois pour vérifier les éventuels effets bord et faire en sorte d'aller plus avant, peut-être dans la sécurité juridique de ce dispositif, donc pour toutes ces raisons, nous souhaitons le maintien de l'article, nous prenons l'engagement que les textes soient travailler avec l'ensemble des acteurs et en tout 1er lieu avec 7 et ceux qui sont intéressés de très près leur financement, je pense à la scène et 5 hommes aux conseils départementaux et avoir une durée d'expérimentation qui nous permettent de nous prémunir contre les effets de bord que j'ai évoqués de manière à ce que celles et ceux qui sont directement concernés, qui travailleront dans ce secteur puisse être pleinement sécurisé accompagner le sud l'expérimentation.

On maintient l'amendement va nous dire qu'on fait un amendement qui dessert un besoin qu'on connaît tous qu'est-ce que c'est cette solution de répit pour les aidants familiaux et de l'autre côté, excusez-moi, mais on n'a aucune réponse, ou alors un un travail un peu quand même léger puisqu'on a déjà eu une expérimentation, donc il fait l'aborder la question du de, de, de la du droit collectif, donc vous pouviez dans le texte, nous dire voilà l'expérimentation s'est faite le besoin est réel partout et bah, examinons les conditions législatives par exemple du temps de pause du du temps de travail des conditions ont cessé les populations les plus fragiles, on le sait ça, donc on peut pas se cacher derrière son petit doigt, j'ai dit à leur augmentation de 45 pourcent des accidents de travail chez ses salariés, c'est les plus fragiles. Dans ce baluchonnage donc on va le retirer mais franchement ça manque de de sérieux et de rigueur. Alors l'amendement est retiré, nous examinons maintenant le nul au 219 de la Commission spéciale présentée par même. merci Monsieur le Président, avant de m'expliquer mon amendement qui sera court, je voulais juste juste rappeler, Monsieur le ministre, que le vrai problème, c'est le financement, je l'ai déjà dit mais je vous le rappelle, et quand vous évoquez les conseils départementaux, moi je suis du département de l'aine on est on pleure à partir du mois de novembre pour qu'on nous aide financièrement au niveau de l'État, parce qu'on a n'arrive pas bouclé, budget, donc voilà, c'est une grande brune interrogation et sincèrement il faut vraiment regarder ce sujet parce que c'est un un sujet de société essentiel mais avec un financement derrière sinon je pense que on en a, on sera au même niveau dans à la fin du du quinquennat alors si j'en viens mon amendement, c'est un amendement de de cohérence en fait on a ajouté ici une précision qui relatives à l'application de la convention collective du particulier employeur aux prestations de relais, il y a, je pense qu'on a modifié le texte et en fait, il y avait un peu un point à corriger, voilà, c'est ni plus ni moins que ça,

défavorable dans la mesure où nous considérons qu'il enferme son adoption fermerait un peu trop le dispositif, notamment dans le cadre expérimental et cela n'enlève rien aux éléments que j'ai apporté tout à l'heure. Donc, avis défavorable pour cette raison-là, sur la question du financement permettez faire cette parenthèse, il se trouve que, lundi, l'association des départements de France, a été reçu par le 1er ministre un certain nombre de membres du gouvernement et j'ai participé à cette rencontre pour justement étudier la manière dont nous pourrions stabilisée, consolidée et conforter le financement des allocations individuelles de solidarité par les départements, puisque nous savons que le déséquilibre ou les difficultés de financement de ces prestations relève désormais d'une période extrêmement longue, nous travaillons sur les bases de la mission animée par note votre collègue Alain Richard et et le préfet Dominique Bur et nous avons fait un certain nombre de propositions à l'association des départements de France, pour que la prise en charge du reste à charge, calculé selon ce qu'on appelle le scénario de c'est-à-dire à hauteur de 600 millions d'euros par an, puissent être abordées les discussions sont en cours mais je puis d'ores et déjà vous affirmer que lors de cette réunion, le 1er ministre a proposé comme entrer dans la discussion, une aide de l'État au département qui serait augmenté de 200 millions d'euros par an pendant 3 ans pour aller jusqu'à la réforme de la fiscalité 200 millions d'euros par an, cela représente plus que la moyenne des fonds d'urgence qui ont été votées au cours des 6 dernières années puisque, au cours des 6 dernières années, les fonds d'urgence ont été en moyenne de 140 millions d'euros pour permettre aux départements de faire face aux difficultés de financement, notamment en fin d'exercice, là, nous considérons qu'avec un accompagnement des tas d'au moins 200 millions d'euros, cela permettrait aux départements de faire face aux difficultés au moins conjoncturel qu'ils rencontrent et dans la perspective à la fois de la refonte de la fiscalité locale, mais aussi du travail qui va être lancé auquel le 1er ministre a rappelé son attachement de mise en du même d'une allocation sociale unique qui serait l'occasion d'une refonte de l'ensemble de ces dispositifs donc le travail avance et le 1er ministre et le président de la DDE de la dérive, on coupe sont convenus, l'un et l'autre que l'idéal serait de pouvoir aboutir avant la fin du mois de mai sur ces questions-là et trouver un accord. Alors un avis défavorable je vous voilà grandement de la commission ah pardon madame Meunier, je vous en prie. Si Monsieur Président une explication de vote Monsieur le ministre nous voterons

mais qui, quand même, mais un peu de concret dans cette bonne idée parce que la personne qui va venir aider la personne âgée, elle est volontaire, salariés, enfin bon, on a discuté de cela en audition et il faut quand même derrière des bonnes idées, être aussi pragmatique et avoir les moyens de réaliser c'est expérimentation et donc nous pensons que l'amendement présenté par la rapporteure va dans ce sens et nous voterons donc cet amendement.

soutiendrai je reviens intervient justement concernant les explications de Madame Bruni au niveau de la Commission spéciale et c'est vrai que les problématiques de vieillissement de population de dépendance, c'est vraiment du sujet particulièrement important que la commission spéciale organisée a suivi que le fait aussi, la commission des affaires sociales au niveau du du Sénat mais concernant l'au l'au niveau des finances publiques et Monsieur le Ministre, vous êtes intervenu concernant les compensations ou le fonds d'urgence, c'est vrai qu'en loi de finances pour 2018, le niveau de notre commission des finances du Sénat, on avait vu gérer les dispositions de l'État en faveur de certains départements concernés Madame Bruni a parlé de son département, moi je parle du département voisin, les Ardennes et il y a des départements qui sont dans une situation, je ne suis plus conseil général depuis 2015 mais j'irai au fil des mois et des années, malheureusement, la situation de certains départements s'est fortement dégradée financièrement sur des mesures du dispositif à caractère social de noms ou le reste à charge reste quand même important, à la charge des départements et c'est vrai que le fonds d'urgence de mémoire son 1000000 d'euros, bon je ne je ne suis pas sûr non plus que les départements et perçu ces derniers temps, ce fonds d'urgence pour un certain nombre de départements, une vingtaine au moins concernés, mais de l'autre côté, je dirais : il y a vraiment nécessité de prendre en compte, je dirais les les situations très difficiles de des collectivités départementales d'aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, mais il y a, il y a quand même des attentes fortes au niveau de des départements, de par leurs engagements financiers ou outil de la solidarité, mais néanmoins je soutiendrai cet amendement. Alors je n'ai plus de demandes d'explications de vote, je mets au voile amendement 219 avec un avis défavorable du gouvernement amendement de la commission qui vote pour. Merci qui vote contre qui s'abstient et manifestement adopté l'amendement suivant le 32 rectifier bis de nombreux signataires c'est madame madame qui nous le présente. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, donc le soutien des aidants, des personnes en perte d'autonomie, comme l'a justement rappelé Madame le le rapporteur de la commission spéciale un grenier est une question de société, c'est un enjeu fort de l'interdisant Sion, social et médico-social, dès lors, la prise en compte des besoins spécifiques et notamment des besoins de répit doit passer par le déploiement de dispositif adapté et sécurisé alors aujourd'hui l'expérimentation prévue par cet article va dans le sens d'une meilleure prise en compte de la situation des étangs, mais cette prestation d'une suppléants supplémentaires ne peut s'apprécier uniquement sous l'angle de la dérogation au droit du travail, c'est la raison pour laquelle, sans remettre en cause l'intention louable de l'article 29 il convient tout de même d'apporter quelques garanties vis-à-vis des personnes et des des aidants, et de la famille, leur famille, c'est le sens de cet amendement. Merci, quel est l'avis de la commission Hamelin. Merci Monsieur le Président, alors l'argumentaire des auteurs de l'amendement, soulignent les interrogations que suscite ce dispositif et qui sont bien réels, cet amendement apporte diverses dispositions de nature à mieux encadrer l'expérimentation du relais, il y a je, néanmoins, on peut craindre qu'en encadrant Alex et l'expérimentation on en Vienne à décourager les initiatives, l'amendement fait notamment peser sur les établissements expérimentateurs, une responsabilité relative à l'information des personnes aidés et des aidants et à la coordination des intervenants, quand on connaît les difficultés que connaissent aujourd'hui les Epad, on peut craindre que ces derniers se refuseront à participer à un dispositif expérimental qui demanderait un surcroît de travail au profit de personnes extérieures de même le suivi médical renforcé qui est proposé correspond à des inquiétudes que je partage, mais il semble difficile à mettre en place dans le mode de mandataires les intervenants étant des salariés du particulier employeur employé pour une période assez courte alors malgré un certain scepticisme, la commission spéciale a souhaité autoriser l'expérimentation et elle souhaite laisser une certaine souplesse au dispositif, le bilan qui en sera tiré permettra, le cas échéant de le préciser, donc je vous propose de retirer cet amendement, à défaut, la commission a émis un avis défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Merci monsieur le président, c'est le même avis, une demande de retrait mais je saisis l'occasion que vous nous donnez pour prendre 3 engagements devant vous d'abord pour dire que le caractère expérimental et l'évaluation devront permettent d'apprécier les impacts, tant pour les personnes âgées ou handicapées accompagne que pour leurs étangs et les salariés assurant les prestations qu'on a trop duré, dans le cahier des charges, il sera prévu dans ce qui est des charges un suivi régulier du relayeur au cours de sa prestation et la possibilité de pouvoir à tout moment, avoir une écoute, que ce soit pour répondre à une situation difficile pour laquelle il a besoin de conseils, voire dans les cas les plus extrêmes comme un accident ou une dégradation de l'état de santé de la personne aidée bénéficie d'un remplacement ou d'un soutien en plus des conditions dites de droit commun de la même manière, la question de l'organisation des prestations dans leur nature, ou leur fonctionnement, les conditions minimales de diplôme, de formation, d'expérience exigée seront abordés dans l'est de l'élaboration du décret d'application qui fixera le cahier des charges de l'expérimentation et donc sur ces points, nous prenons l'engagement d'aller dans le sens que vous souhaitez dans l'île dans de poursuit des objectifs que vous recherchez sans encadrer l'expérimentation de manière aussi drastiques que l'adoption d'autres amendements aurait comme conséquence, donc c'est une demande de retrait ou, à défaut, évidemment, un avis défavorable. Alors Madame Canayer de demandes de retrait, que faites-vous. Oui effectivement, donc, j'entends les engagements du gouvernement qui sécurise le dispositif et la volonté de Madame le rapporteur, que nous partageons, de donner de la liberté pour pouvoir pouvoir mettre en place cette expérimentation attendu donc je retirer cet amendement. L'amendement est donc retiré, nous allons pouvoir voter sur l'article 29 pas demande d'explications de vote, je n'en vois pas qui votent pour cet article. Merci qui vote contre qui s'abstient, il était adopté l'article 31 après l'article 30 je suis saisi l'amendement 156 monsieur Ouzoulias, vous nous le présente. Si Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'amendement que nous vous proposons maintenant a été cosigné par des députés de l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale et il vise à renforcer l'efficacité du dispositif de la loi de décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique qui prévoit des sanctions spécifiques pour les sociétés, transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires et qui manquent à leurs obligations en matière de dépôts de leurs comptes la publicité des comptes, vous le savez, revêt une importance particulière dans le secteur agricole et agroalimentaire en raison d'une répartition très inégale de la valeur ajoutée, cette question a été au coeur des discussions dans le cadre des états généraux de l'alimentation, certains acteurs de ce secteur continue cependant de manquer à leurs obligations, en raison notamment de sanction particulièrement faible, c'est pourquoi le présent amendement propose de les renforcer en supprimant l'intervention du président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges de produits alimentaires et en confiant directement au président du tribunal de commerce, la mission d'adresser à ses sociétés des injonctions sous astreinte lors des débats à l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre, vous avez répondu cette question sera au coeur de la discussion qui accompagnera l'examen du texte de la loi sur l'agriculture ici issu des états généraux de l'alimentation, vous allez nous faire la même réponse et nous ou disons comme ça a été dit à l'Assemblée nationale, qu'il nous semble que sur ces problèmes-là, il y a une urgence et donc nous maintiendrons notre amendement, quel que soit votre demande merci. Voilà qui est dit, quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement même d'être rappelé en même temps permettre au président du tribunal de commerce d'enjoindre sous astreinte à une société commerciale commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires de déposer ses comptes auprès du greffe, le montant de cette astreinte irait jusqu'à 2 pourcent du chiffre d'affaires journalier réalisée en France, il reprend le dispositif de la loi de décembre 2009 16 E relative à la trace à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, mais là où celui-ci permettrait au président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges de produits humanitaires de saisir le président du tribunal de commerce celui-là permet à ce dernier de se saisir lui-même, cet amendement fait écho. Vous le savez, toutes et tous à l'actualité récente d'une entreprise française. Qui dont l'activité concerne l'agroalimentaire. Lors de l'audition de l'entreprise Lactalis s'. Nos collègues de la commission des affaires économiques, un certain nombre d'entre vous y participer, la question de l'absence des pour, des comptes au greffe a d'ailleurs été soulevée à plusieurs reprises. Je m'interroge néanmoins sur la pertinence de cet amendement à double titre. Premièrement, je suis réservé sur le fait que, compte tenu de l'actualité sur le fait de réagir à chaud, sans réflexion globale sur une refonte du dispositif de la loi de 2016, lequel d'ailleurs commence à produire ses effets, un tribunal de commerce, sachez-le, a été saisi et l'entreprise Lactalis s'pour ne pas le nommer, a récemment commencé à déposer, certaines de ses comptes, Deuxièmement, cet amendement introduirait dans un chapitre du code de commerce relative Alain-Sam mais de sociétés commerciales, une disposition spécifique à c'est le transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires. C'est ainsi que. La commission a émis un avis de sagesse. Merci Monsieur le Président, c'est sénateur, je ne vais pas vous demander le retrait puisque vous avez déjà répondu à cette question et je ne vais pas renvoyer non plus au texte qui sera issu des états généraux de l'agriculture, je vais simplement les difficultés que nous posent votre amendement en tout cas son intégration dans le présent texte. Le président du tribunal de commerce dispose déjà d'un pouvoir général d'injonction en cas de non-dépôt des comptes annuels applicable quel que soit le secteur d'activité, d'abord dans un objectif de sanctions, en application de l'article L 123 sentir un du Code de commerce et dans cette hypothèse, le président est saisie par tout intéressé ou par le ministère public et dans un 2ème objectif, un objectif de prévention, en application de l'article L 611 tirs, 2 du code de commerce et dans cette hypothèse, le président se saisi d'office s'agissant d'un dispositif destiné à contraindre les grands groupes du secteur agroalimentaire a publié leurs comptes annuels, il ne nous paraît pas avoir sa place, le rapporteur a évoqué dans un chat pique du code de commerce relatif à la prévention des difficultés de l'entreprise, s'agissant d'une question prioritaire saisie par le conséquence constitutionnelle en effet relevé comme instituant cette faculté de saisine d'office, le législateur a poursuit un objectif d'intérêt général de détection et prévention des difficultés des entreprises et je renvoie la à la QPC du 1er juillet 2016, ce qui rend difficilement opérant l'intégration de la disposition vous souhaitez dans cet article, or il est évident, si, si, ça rend inopérants, parce qu'il est évident que ce n'est pas en raison de leurs difficultés financières que les entreprises que vous visez refuse déposer leurs comptes, enfin il est un craindre un risque d'inconstitutionnalité sur le fondement de la rupture de l'égalité devant la loi, puisque votre amendement créant pour les seules sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires, une obligation plus rigoureuse que pour les autres sociétés commerciales soumise à l'obligation de dépôt de comptes en application des articles L 232 tiré 31 L 232 tiré 33 du code de commerce, pour ces difficultés que je ne. Pas donné un avis favorable à votre amendement, vous voyez, notamment sur l'intégration de telles dispositions dans l'article du Code du commerce, que vous citez, que nous avons aussi du travail à faire pour pouvoir, à l'occasion d'un autre véhicule législatif peut-être celui issu des états généraux, pouvoir donner satisfaction à vos demandes. Donc un avis de sagesse de la commission défavorable du gouvernement allemand est maintenu, j'avais bien compris, pas de demandes d'explications de vote, je vais le mettre aux voix qui vote pour.

Qui vote contre qui s'abstient, il est adopté à l'article 32 l'amendement numéro 159 qu'il présente pour le groupe CRC. Monsieur ou 1er 1er point cet cet article m'a rappelé un certain nombre de souvenirs. Les tribulations les

on a botté en touche pour Dexia, une première fois, c'est parce que précisément, un certain nombre de communes, collectivités avait eu avait eu gain de cause devant le tribunal de Nanterre parce que les contrats sur ces fameux prêts toxiques ne ne comportait pas de la mention du du taux du TEG.

donc je ne peux pas ne pas me me dire cette cette disposition peut-être sera accueillie très favorablement par les banques, on va comme c'est pas mon objet 1er, je préfère garder la législation telle qu'elle existe et puis 2ème 2ème point mais ça le collègue qui présente l'amendement 93 développeront il y a effectivement aussi une certaine forme d'atténuation des exigences en matière de notation le droit français, pour l'instant étant étant quand même plus sérieux, plus strictes que ce qu'on nous propose de mettre en place. Quel est l'avis de la commission madame la rapporteure. Merci monsieur le président, alors votre amendement supprimerait l'ensemble de l'article 32 alors que l'objet évoque seulement la question du taux effectif global, dit TEG il me semble que l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale et le bon, le TEG sera bien conservé, surtout les prêts à taux fixe, qui constituent la quasi-totalité des prêts aux PME et les banques comme les représentants des des PME que nous avons rencontrés sont favorables à cette solution, comme ça, c'est comme ça, cher collègue, donc, de ce fait, la Commission, en fait, a donné un avis défavorable à votre amendement. Je le ministre pour le gouvernement, s'il vous plaît. Merci monsieur le président, le gouvernement partage l'appréciation de la Commission sur cet amendement sur l'article en général, donc la vie, tout aussi défavorable. 2 avis défavorables Monsieur Collombat et la parole.

c'est pas avec les taux des prêts à taux fixe, bon. Et donc voilà, et je comprends, franchement je ne je ne aussi si je comprends très bien et je comprends très bien que les banquiers soient ravis de la du cadeau que vous leur faites. Monsieur Barre, Merci monsieur le président, il y a quand même aussi l'idée dans cet article. Le droit français assure sur transposer le les directives européennes, je crois que dans cette instance sont, on le rappelle à ses régulièrement et on s'en émeut, hein, ici au Sénat, de dire c'est c'est voilà cette manie d'aller au-delà, finalement des des directives européennes, donc cette partie-là est intéressante j'ajoute aussi que c'est dans le cas quand même de l'attractivité de de la place de Paris et vous savez que dans le cadre du Brexit je pense que nous sommes tous attachés à, à ce que on puisse renforcer l'attractivité de la place parisien. Alors 2 avis la rapporteure vouliez ajouter quelque chose. juste signaler à mon collègue que là on est que sur la partie théologie et pas sur les agences de notation, c'est l'amendement suivant. Monsieur Savoldelli m'demandé la parole. Eh bien, merci Monsieur le Président pour prendre un un exemple concret pour montrer qu'on a su se rassembler à d'autres moments sur le sujet que par Yves Collombat développer si j'ai bonne mémoire et vous allez voir que vous êtes concernés, Monsieur le Président, c'est quand on avoue rappeler, on a eu un débat sur le TEG sur des crédits aux particuliers. Nous avions mis en évidence le problème des vents qui est de contrats promis de prêts immobiliers de contrats d'assurance sur ces prêts, il s'agissait quand même pour pas prendre à la légère ce que dit mon collègue et ami Pierre-Yves Collombat, il s'agissait d'un petit pactole quand même de 6 milliards d'euros, mes chers collègues, et si j'ai bonne mémoire, nous y sommes attaqués ici avec vous, président d'alliés et mon collègue Bourquin pour n'en citer que 2 parmi d'autres, donc voilà donc la question telle que nous la prenons n'est pas seulement la question du seul groupe communiste républicain écologiste et citoyen.

agences de notation, mais parce que le débat sur le l'été j'ai déjà eu beaucoup lieu à l'Assemblée nationale, donc on n'a pas forcément voulurent avoir le même débat mais nous sommes dans la même la même analyse que nos collègues donc nous soutiendrons l'amendement de suppression et en forme de repli, nous avons aussi l'amendement sur l'agence de notation. Donc on est bien sûr le 159 il n'y a pas d'autres. Voilà donc cette fois-ci je l'mais on voit 2 avis défavorables, je vous le rappelle, qui vote pour.

relatives aux agences de notation ont pour but d'aligner le droit français sur le droit de l'Union européenne, alors que ce dernier est moins complet sur la méthode, nous saluons le travail qui a été fait par la commission spéciale lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, car la supprimer la mesure initiale, qui consistait à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance encore une toute mesure en vue de simplifier le régime de responsabilité des agences de notation, pas d'habilitation aller à légiférer par ordonnance, mais en revanche, l'Assemblée nationale a souhaité une suppression franche et directe le d'un certain nombre d'articles du Code monétaire et financier, notre amendement tend à revenir sur le fond de cette décision, le droit français impose aux agences de notation de crédit, un engagement de leur responsabilité civile plus extensive que celui du règlement européen sert à trois, notamment sur la nature de la responsabilité engagée, le requérant peut ainsi choisir d'avoir recours à la responsabilité délictuelle de l'agence, malgré l'existence d'un contrat, en outre, la loi française n'implique pas la nécessité pour le requérant d'apporter la preuve de l'impact de la notation le droit français va donc plus loin que le droit européen puisqu'il ouvre une responsabilité large qui sera qualifié par le juge saisi de la question, alors que le droit européen se base sur une approche au cas par cas. Par conséquent, si l'article 32 était adopté en l'état la spécificité du droit français en la matière, disparaîtrait entraînante alors une responsabilisation moindres des agences de notation et l'application d'un droit, nous refusons cette logique, considérant que le droit français en matière de responsabilité des agences de notation n'est pas contraire mais complémentaires au droit européen, qu'il n'y a pas de conflit d'interprétations possibles, nous vous proposons donc en conséquence de maintenir telle qu'il existe le régime français de responsabilité des agences de notation et ainsi de supprimer ces animé à quand on sait les problèmes qui ont eu lieu en raison de parfois de une certaines divagations d'agences de notation, on voit bien l'intérêt qu'il y a à les responsabiliser au maximum. Très bien quel est l'avis de la commission. Madame l'emporte. Merci monsieur le président, donc, cet amendement propose de revenir sur la suppression des dispositions du code monétaire et financier qui prévoit un régime de responsabilité délictuelle pour les agences de notation assortie d'un large pouvoir d'appréciation du juge résultant de la loi du 22 octobre 2010 sur la régulation bancaire et financière, ce régime de responsabilité nationale diffère du régime européen harmonisé intervenu ensuite par l'intermédiaire du règlement sur les agences de notation 10 je suis défavorable à cet amendement car les spécificités du régime français de responsabilité des agences de notation ne sont plus ni justifier dès lors que le régime est un est harmonisé au niveau européen et que la supervision des agences de notation est assurée depuis le 1er juillet 2011 à l'Autorité européenne des marchés financiers, ni pertinent dès lors qu'elles sont susceptibles de réduire l'attractivité de la France dans un contexte où le Brexit appellent à une reconfiguration des places financières continental, donc c'est un c'est un avis défavorable. monsieur le président, le gouvernement partage les arguments de Madame la rapporteure et ajoute simplement j'ajoute simplement pardon que nous considérons l'espèce qu'il s'agit là d'une sur-transposition de la directive, c'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement. 2 avis défavorables. Pas de demande d'explications de vote, si j'ai Savoldelli. ça va être très rapide, mais l'autre collègue sénatrice président, Monsieur le Ministre. Je pense qu'elle a tout à fait raison. C'est que la loi française s'avère nettement plus protectrice des intérêts débiteurs que le texte européen d'ailleurs, des fois on nous trompe un petit peu sur la marchandise irai dire alors après des fonds, ils mettent des des vocables différent peut faire un peu de sémantique. Mais moi, je considère qu'il faut pas qu'on sait s'amuser par un abus de langage. C'est pas laisser croire en général que le droit communautaire sera comme le plafond législatif. Et que nous ne saurions dépassé alors qu'en fait qui n'le plancher, donc les sénateurs et les sénatrices nous les parlementaires, nous faisons notre travail. Donc, faut pas confondre le plancher et le plafond. Donc c'est un socle minimal et nous sommes en devoir si nous considérons que c'est juste d'améliorer ce socle minimal, donc l'argumentation, excusez-moi, madame, le rapporteur, Monsieur le ministre, pour moi, allez-y recevable.

à chaque fois on nous réplique, maintenant il y a le Brexit et on va en de moins en moins loin sur la question de la régulation de la finance sur la place de Paris sur la question des agences de notation pour attirer

et donc c'est important de pouvoir défendent la place de Paris et y compris dans le cas du Brexit j'ajoute que, il y a un autre lieu pour renforcer le le cadre européen, vous dites on peut aller plus loin, mais dans ce cas-là, modifions la directive européenne, il y a une assemblée qui le Parlement européen qui peut m'être qui peut m'être si il le veut, le niveau de la réglementation européenne au niveau de la réglementation que vous proposez pour la France, et dans ce cadre et dans ce cas là on aura un cadre commun mais j'ai l'impression que dans vos discours dans votre expression, j'ai l'impression toujours que nous sommes tout seul, je crois que c'est de bon sens de dire on ne sur transpose pas et on tient compte des réalités actuelles. Cette fois-ci plus personne vraiment. Non, et sur l'amendement numéro 93, mon cher collègue, donc cette fois-ci je mais on voit qu'ils votent pour. Qui vote contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée. Alors maintenant, sur l'article 32 et demande explication de vote Monsieur combat j'ai bien compris que vous souhaitiez vous exprimer. Oui, parce que je suis pas sûr que on réalise bien la situation. On a l'impression que, bon, ben, la crise est derrière nous regarder tout report, c'est très bien, je vais dire, sauf que le système financier il est. Toujours aussi volcanique. Même peut-être encore plus. En 2007. La spéculation est repartie de plus belle. Est ce qu'on nous propose, ce que le gouvernement nous propose. Eh bien si, comme en 2007, il faut suivre.

Et un bon matin on va se on on va se réveiller avec une crise quelque part qui deviendra une crise systémique. Mais alors là, comme en 2009 comme en 2010 comme en 2011 dire ou alors il faut réformer tout ça il faut réguler,

vous croyez que c'est sérieux, vous croyez oui à court terme, à court terme, il y a eu qui adhérent à faire ça, c'est sûr. Mais à court terme, c'est pas long et alors qu'on mette ce type de disposition dans un texte comme celui-là, Texas surprise. Franchement, je préfère ne pas donner de qualificatifs, enfin c'est une escroquerie quand même bon on met pas on on prend pas de telles décisions dans un texte comme celui-là, quel rapport avec la société de confiance, on est pas dans la société de confiance, hein, on est dans la société de dissimulation.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre mis chers collègues cet article à expérimenté pour une durée de 3 ans, une procédure simplifiée de consultation du public pour certains projets nécessaires à une activité agricole, je me félicite de la rédaction adoptée en commission qui a supprimé cette partie-là et qui a cette cette procédure donc excluait par la suppression de l'enquête publique des citoyens débat et à commencer tout simplement par tous ceux qui sont les vulnérables numérique et le paradoxe, c'est qu'il s'agissait de projets agricoles et qu'il s'agissait pour ces projets agricoles de recourir à une consultation par voie numérique d'autre part, j'ai une inquiétude sur l'amendement qui va être débloquée déposé par le gouvernement et qui ne respectent pas la sagesse de la chambre haute, comment donc pallier l'exclusion de certaines populations, le plus souvent rurales qui ne peuvent accéder à cette consultation électronique et puis comment remplacer une enquête publique classique qui permet à nos concitoyens d'avoir accès à de l'information en Direct si je puis m'exprimer ainsi, auprès des commissaires un enquêteurs notamment assortie de l'opportunité de pouvoir débattre et d'entendre des points de vue contradictoires propres à se forger une opinion, donc en effet, cette proposition de repli de mises à disposition dans les préfectures et sous-préfectures pour consultation sur support papier ignore totalement la réalité des routes et des distances à parcourir pour se rendre en préfecture dans les territoires comme notamment le mien plus particulièrement là où j'habite dans le nord du Lot, je suis à 3 quarts d'heure de la sous-préfecture de Figeac, à une heure et quart de la préfecture de Cahors, voilà merci. Alors, nous allons pouvoir passer à l'examen de l'amendement numéro 200 cas du gouvernement Monsieur Millon. Merci monsieur le président, il s'agit effectivement de réintroduire l'article 33 d'expérimentation, la participation électronique dans un nombre limité de région pour les procédures donnant lieu à, information et participation, il s'agit pour nous de concentrer l'expérimentation sur quelques régions afin de permettent d'apprécier les effets d'un remplacement d'enquête publique par une participation les chroniques, y compris pour les services administratifs concernés et sur l'attractivité induites par le dispositif de concertation, il il s'agit aussi d'élargir son Champ au-delà des seules activités agricoles, il a ainsi proposé d'élargir le Champ d'application à tous les projets, requérant une autorisation environnementale, la précision apportée par l'Assemblée nationale sur le Champ géographique, donc il doit être tenu compte dans l'organisation de la procédure pour l'étendre à l'ensemble de la zone d'impact du projet, à savoir la commune d'implantation et celles sur lesquelles les impacts environnementaux n'est pas repris l'article L 123 19 prévoit déjà que le public est informé par un avis mis en ligne, si par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés, l'article R-123 tirer 46 tirer un prix pour son application précise que la vie est affichée dans les mairies des communes dans le territoire et susceptibles d'être affectés par le projet, enfin, le dispositif proposé garantit la prise en compte des citoyens éloigné du numérique, en prévoyant les mêmes dispositions que celles qui figure aujourd'hui aux articles L. 123 19 et suivants du Code de l'environnement, relative à la participation publique telle que la mise à disposition dans les préfectures et sous-préfectures pour consultation suspens sur support papier et la possibilité d'adresser ses observations par voie postale, ce sont les conditions qui existent aujourd'hui, qui sont ainsi reprises. Merci quel avis la commission passionnant porteur. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, d'être rappelé cet amendement prévoit de rétablir l'expérimentation qui vise à faire en sorte que les projets soumis à l'autorisation environnementale et qui ont donné lieu de concertation préalables, sous l'égide d'un garage, fasse l'objet a lieu a lieu et place d'enquête publique d'une procédure de participation du public par voie électronique, mais contrairement à la version initiale de l'article 33 du projet de loi qui prévoyait que cette expérimentation ne concerne que les projets agricoles cet amendement va beaucoup plus loin puisque cette nouvelle procédure concernerait l'ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, le remplacement de l'enquête publique, par une procédure de consultation par voie électronique concernerait donc nombre bien plus important, 2 projets. 3 raisons ont incité la Commission spéciale à supprimer cette expérimentation, la 1ère c'est la participation du public au moment de l'théorisation des projets par le biais de l'enquête publique reste déterminante pour assurer l'acceptabilité des projets pour les porteurs de projet à consulter le public le plus en amont possible doit donc pas se faire au détriment de l'enquête publique, deuxièmement la concertation préalable avec garant et de nature différente de l'enquête publique réalisée par un commissaire enquêteur, en effet, les gares, Anne désigné par la commission nationale du débat public ont pour fonction principale de veiller à la bonne organisation de la consultation du public alors que les commissaires enquêteurs enquêteurs rôle plus approfondis, puisqu'ils animent le débat public et qui se prononce à la fin de l'enquête sur l'opportunité du projet par un avis motivé cet avis motivé permet d'ailleurs d'éclairer la décision de l'autorité administrative, troisièmement, la procédure d'enquête publique permet aux citoyens qui le souhaitent de rencontrer les commissaires enquêteurs pour leur faire part de l'eau et de participer à des réunions publiques en présence éventuellement du porteur de projet, cette dimension présidentielle qui fait défaut à la procédure de consultation par voie électronique est importante puisqu'elle facilite les échanges et permet aux citoyens éloigné du numérique d'être associés à la prise de décision pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement. Alors, amendement du gouvernement : avis défavorable de la commission pas demande d'explications de vote, je n'en vois pas qui vote pour cet amendement.

Merci qui vote contre qui s'abstient, il est adopté à l'article 33 bis, l'amendement 61 qu'il présente monsieur leurs jetons. Oui, c'est un amant qui précise et qui dit que pour dans le cadre de la participation publique, c'est le maître d'ouvrage qui doit financer les publications, donc c'est un amendement qui complètent et qui dit : qui finance les publications telles qu'elles sont prévues.

Merci qui vote contre qui s'abstient, il est adopté, article 34 l'amendement numéro 160 qu'il présente, je vous en prie. Merci monsieur le président, il s'agit d'une suppression d'articles depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs s'emploient à moderniser le droit de l'environnement afin de répondre aux critiques régulières des porteurs de projets industriels énergéticiens ou encore aménageur qui considère que le droit de l'environnement peut être un frein au développement de leur activité, l'article 34 échappe à cette logique est habilite le gouvernement dans la perspective de favoriser un développement rapide des NRJ renouvelable en mer à simplifier et accélérer par voie d'ordonnance, les diverses procédures nécessaires conjointement avec la procédure de mise en concurrence à l'implantation des installations de production nous pensons pour notre part que la transition écologique, développement des énergies renouvelables, sont devenus des oeufs, les sujets majeurs pour le pays et l'ensemble de nos concitoyens s'ils jouent des choix engageant pour plusieurs décennies de lourds investissements d'infrastructures, c'est un choix de civilisation, en somme, il apparaît donc 4 cavaliers de traiter ce sujet par ordonnance et d'éviter ainsi un débat public et parlementaire. D'autant que ces dernières années différentes ordonnance en la matière ont été ratifiées par le Parlement, la dernière date d'il y a quelques semaines à peine, cette position est conforté à la lecture des amendements déposés sur l'article 34 entre autres par le gouvernement qui l'autoriserait à renégocier, voire à postériori des appels d'offres d'éoliennes Offshore déjà attribués, le tarif, je cite, accordé aux lauréats des appels d'offres de 2012 et 2014 et très élevé et une correspond plus au prix actuel de l'éolien en mer, entraînant des rémunérations excessives pour les candidats retenus pour conclure à chaque modification du droit positif par voie d'ordonnance, il y a une réduction des possibilités d'intervention des élus locaux dans le débat et de leur pouvoir de concertation, c'est pourquoi nous pensons qu'un véritable projet de loi dédiée aux énergies renouvelables et à l'éolien en particulier devrait être présenté à la représentation nationale, en lieu et place d'ordonnances éparses, sans cohérence merci. Monsieur le rapporteur, quelle est la ville, les commissions, s'il vous plaît. Même d'être rappelé cet amendement vise à supprimer l'habilitation donnée au gouvernement pour réformer le régime juridique des énergies marines renouvelables au motif que cette habitation ne mettrait pas permettrait pas, je cite, un débat public et parlementaire. J'ai déjà eu l'occasion de de rappeler à une commission, mais ma position sur les habitations qui du reste est partagé par ma collègue Pascale Gruny nous considérons un effet que l'habilitation législative peut se justifier lorsque la forme est excessif demande est excessif demande technique ou que ses modalités sont encore incertaines, mais qu'elle doit impérativement être encadré par le législateur d'un sur-le-champ comme à sa durée est limitée également au strict nécessaire, c'est précisément ce à quoi nous avons baigné d'un samedi du texte en l'espèce, le recours à une habilitation, dans le cas présent, me semble acceptable, d'une part parce que les contours de la réforme ont été clairement explicités, notamment depuis la réécriture de l'article, intervenu à l'Assemblée et, d'autre part parce que la sa mise, Hanovre concrète nécessite encore un certain temps de réflexion et de concertation, je signale par ailleurs que notre commission a dû réduire la durée de l'habilitation. Quant au débat public et parlementaire. Mes chers collègues, nous sommes bien dans l'hémicycle du Sénat. Et nous nous débattons. Sur le sujet. Hein c'est testant. Bien évidemment, mais ce débat, il y a eu lieu également à une commission et avant cela à l'Assemblée nationale et il aura encore lieu lors de la ratification des ordonnances et puis de la remise du rapport d'évaluation prévues au présent article qu'2000, tous ces éléments, il vous est proposé un avis défavorable. Monsieur lui dis ce que est la vie du gouvernement s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, c'est un avis qui est aussi défavorable en soulignant combien le gouvernement considère que le développement des énergies renouvelables en mer devra contribuer fortement atteint l'objectif de 40 pourcent d'énergies renouvelables dans la consommation française d'électricité en 2030, mais en soulignant aussi qu'actuellement, le délai entre la désignation du lauréat et la construction du parc éolien estimez est estimé à 10 ans et qu'une simplification de la perte de la procédure permettra une réduction substantielle de délai et donc sera vecteur d'économies importantes dans les coups de soutiens publics accordés, donc nous ne pouvons accepter de voir supprimer cet article 34. Alors 2 avis défavorables chez ou encore augmenter l'amendement.

et que je pense que les énergies renouvelables, l'éolien en particulier, on peut pas l'aborder comme ça. Daïc de la parole. Oui pour dire je suivrai le rapporteur et tout le monde sait à quel point je suis extrêmement attentif au développement de l'éolien, je crois que le problème, c'est que le débat est très empoisonné mais on va y revenir après la la dernière décision du gouvernement sur le prix de rachat, ce qui n'est pas du tout le même débat, mais il faut reconnaître que sur la question de la simplification et notamment aussi pour l'éolien terrestre il y a un vrai travail de concertation et là effectivement l'ordonnance arrive après ce travail, qui semble être respecté par le gouvernement, donc là je pense qu'on peut rester continuer à faire confiance au gouvernement tout en disant qu'évidemment l'annonce qui a été faite sur le prix de remise en cause de ce qui avait été décidé fragilise la confiance, mais malgré tout on va rester sur l'idée que le travail d'obus avait été fait avec les industriels et qu'effectivement, on est obligé de reconnaître que c'est beaucoup trop long pour la la mise en oeuvre des des projets, donc je suis, elle rapporte. Pas d'autres demandes de paroles ou d'explications de vote donc jamais aux voix l'amendement soit 100 162 avis défavorable qui vote pour. Merci qui vote contre. Merci, il n'est pas adoptée, nous avons ensuite 2 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune j'ai Cuypers pour le 16 rectifier bis. Oui, monsieur le président, Monsieur le ministre, telle qu'il a été modifié à l'Assemblée nationale par amendement du gouvernement, l'article 34 traduit la volonté de ce dernier, de permettre l'évolution du cadre de développement des énergies marines renouvelables, il a pour but d'aboutir à un nouveau processus de développement et d'autorisation des installations en mer équilibré dans la répartition des rôles entre l'État et les producteurs, il est de ce fait, de proposer aux lauréats des appels d'offres un permis enveloppe qui le pain qui leur permettra de modifier leurs projets dans les limites définies une fois les autorisations bien sûr obtenus il contribuera ainsi à la mise en place d'un schéma de réforme des coups et des délais, des projets décidés le développement des énergies renouvelables marines est en effet indispensable à l'accélération de la transition énergétique et au développement de la production d'énergies renouvelables, à l'instar d'ailleurs du photovoltaïque, mais les EMR resterait soumise à 2 autorisations une autorisation environnementale et une autorisation d'occupation du domaine public Marine donc afin de parachever le processus de simplification, initié par l'article 34, il est donc nécessaire de parvenir à une autorisation unique en mer qui regrouperait l'autorisation environnementale et le titre d'occupation du domaine public maritime, les opportunités de recours : 2 tiers seraient donc ainsi alors limité à une seule : telle est le sens de cette amendement.

complèterait efficacement la simplification, moi je ne parlais du cadre réglementaire de ces projets, telle est la réforme Nash. Alors Monsieur l'emportera l'avis de la Commission sur ces 2 amendements identiques. Oui, merci Monsieur le Président, en fait, pour ces 2 articles, pour ces 2 amendements, pardon, c'est 2 à l'amendement 100 satisfait par le texte, donc il est demandé une demande de retrait ou un avis défavorable dans le texte, vous avez la réponse aux différentes questions que vous avez posée. Monsieur le ministre, êtes-vous du même avis. Merci Monsieur le Président, je je crains de ne pas tout à fait partager l'avis du rapporteur, mais ce qui ne m'empêchera pas pardonné d'être défavorable à l'amendement parce que je considère par contre que. le texte ne répond pas aux intentions, les 2 auteurs de l'amendement, mais le gouvernement considère aussi que les intentions qui sont poursuivis ne peuvent pas être soutenu à ce stade. Plusieurs arguments millilitres contre une fusion, une autorisation unique pour l'éolien en mer les autorisations sur le domaine public maritime et celle délivrée au-delà de la mer territoriale ne peuvent en aucun cas être fusionner les régimes de la loi sur l'eau, le code de l'environnement et la 2002 de la domanial était publics le code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas bien applicable en zone économique exclusive et sur le plateau continental ces zones situées au-delà, au-delà des 12000 marins sont régis par la convention des des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 par l'ordonnance du 8 décembre 2016 et par le décret d'application de la loi biodiversité 2 mai 2007, ainsi les droits des compétences des états ne sont pas les mêmes suivant l'espace maritime considéré et la rédaction proposée dans les amendements et contraire aux textes internationaux, la création d'une autorisation unique spécifique au projet de production d'énergie renouvelable en mer, incluant l'autorisation domaniales et l'autorisation environnementale est source de contentieux, la nature du titre domanial, s'agissant d'une concession d'utilisation du domaine public maritime dont un contrat sous sa forme actuelle permet une négociation portant sur les conditions et les limites de l'occupation du domaine public maritime entre les l'État est le lauréat de l'appel d'offres, si nous fusionnons ce titre avec l'autorisation environnementale en y associant notamment les mesures compensatoires y à l'évaluation environnementale la concession changerait de nature et aucune négociation ne pourrait être conduite, sans être contraire au droit européen 7 heures historique unique risque par ailleurs de rallonger le délai d'instruction alors que par ses articles, nous poursuivons un objectif inverse de simplification et donc pour ces raisons-là, c'est un une demande de retrait de ces 2 amendements qui dans leur application ne saurait être compatible avec les textes européens et internationaux. Merci Monsieur 800 j'aime retourner vers les hauteurs, les amendements puisque la commission propose le retrait en vous disant: vous devriez être satisfait Gelmini vous demande le retrait mais pour des raisons manifestement assez différentes, que faites-vous, chers collègues. Monsieur le président, on peut pas dire que nous soyons satisfaits dans la mesure où, notre le bon sens veut que nous puissions simplifier justement un certain nombre de réglementations et que les règles de la communautaire puisse évoluer, ceci étant, puisque c'est repris, comme le dit le rapporteur dans le texte, bien sûr, j'accède à condition de du retour de retrait, à condition qu'il soit bien précisé la précision qui est faite dans le texte. Alors monsieur rapporteur. Oui. Oui, merci Monsieur le Président pour rassurer mon collègue s'il en était besoin, dans le projet de loi document que nous avons, page 46 3ème alinéa, je vous laisse regarder mon cher collègue. 3ème il y a, il est bien montée. Quasiment 2, 3, 4 lignes avant la fin. La zone économique exclusive ou le plateau continental d'une ou de plusieurs autorisations. donc. Pour la. Donc je maintienne l'avis défavorable, avec des raisons différentes, vous l'avez rappelé monsieur le président, différente que que monsieur le ministre, mais mais mais je maintiens mon avis défavorable Camus. Bon alors, j'ai cru comprendre que le 16 rectifier s'était retiré il est retiré, je me tourne vers de coller Courteau : que faites-vous pour le 60. Non, moi je n'ai pas été convaincu ni pas monsieur le ministre, ni par monsieur le rapporteur, je le maintiens. Très bien, donc je vais me mettre au bois pas demande d'explication de votre supplément. Donc 2 avis défavorables qui votent pour le 62. Merci qui vote contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adoptée, nous avons ensuite 4 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune monsieur Courteau s'est de nouveau à vous pour le numéro 100. Merci Monsieur le Président, oui, la réforme que l'article 34 habilite le gouvernement à mettre et comme Plex Édouard reposé sur une analyse juridique robuste dans l'État structurante pour l'ensemble de la filière française des énergies marines qui est déterminé à être au rendez-vous des objectifs fixés par la loi de transition énergétique et la programmation pluriannuelle de l'énergie, il est donc nécessaire de donner, vous ne ment le temps suffisant pour élaborer une ordonnance qui répondent aux principes fixés par l'article 34 sur la base d'une concertation approfondie avec l'ensemble des services et en particulier des services instructeurs des les thèmes, la Dreal qui ont instruit les demandes d'autorisation des projets sélectionnés dans le d'premiers appels d'offres d'éoliennes en mer afin de faire évoluer les procédures de Total en compte du retour d'expérience, à qui il peut être un autre être particulièrement utile d'établir une comparaison détaillée des régimes d'autorisation aux énergies marines renouvelables dans les pays européens où de terre des installations d'été mise en service pour tirer le meilleur des règles et pratiques en vigueur au Royaume-Uni Anna Magne au Danemark ou encore en Belgique.

de 12 à 18 mois le délai de publication des ordonnances, vous l'avez compris comme cela vous a été expliqué, compte tenu de l'importance de ces ordonnances pour l'avenir de cette filière énergétique, il nous semble opportun que ce texte écrit en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière.

et doit reposer sur une analyse juridique robuste tout en étant structurante pour l'ensemble de la filière française des énergies marines renouvelables qui est déterminé à être au rendez-vous des objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et la programmation pluriannuelle de l'énergie, il est donc fondamental de donner au gouvernement le temps suffisant pour élaborer une ordonnance qui répondent aux principes fixés par l'article 34 sur la base d'une concertation approfondie avec l'ensemble des des services et en particulier les services instructeurs que sont la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du logement, des 4 départements qui sont concernés, qui sont, qui les demandes d'autorisation des projets sélectionnés dans le cadre des premiers appels d'offres éolien en mer, le but étant de faire évoluer les préoccupations, les procédures, tout en tenant compte du retour d'expérience acquis cet amendement, s'inscrit dans la suite logique de celui que nous avons déposée tout à l'heure, l'article 34. Oui, merci Monsieur le Président, donc là ça ne de ces amendements qui ont pour objet de rétablir à 18 mois le délai d'habilitation accordée au gouvernement pour réformer les règles applicables aux énergies marines renouvelables au motif comme tels délais seraient nécessaire pour mener une concertation approfondie tant avec l'ensemble des services instructeurs qu'avec des acteurs de la filière, je voudrais vous rappeler que cette concertation avec la filière et ses représentants et non seulement déjà bien engagée, mais elle a surtout déjà abouti à une réécriture complète du Champ de l'habilitation par un amendement du gouvernement adopté à l'Assemblée nationale, quant à la consultation des services instructeurs je n'imagine pas que le gouvernement est envisagé cette réforme sans les avoir préalablement consultés, j'ajoute que la France a déjà pris beaucoup de retard à la matière, je rappelle que les premiers parcs d'éoliennes posées attribué en 2012 et 2014 n'entreront pas un service avant 2020 et au Moyen, mais je suis persuadé qu'on y reviendra tout à l'heure, mais que cette réforme a précisément pour but d'y remédier et que la contrainte des 12 mois qui au passage ne débuteront qu'à compter de la mais bien sûr, de la loi incitera une mise en oeuvre rapide indispensable à l'atteinte de nos objectifs de développement des énergies marines renouvelables

a fortiori sur de tels sujets structurants pour l'avenir de notre pays est très consommateur de ressources publiques, c'est ainsi que la commission n'a donné un avis défavorable. Merci Monsieur le Président, j'ai j'ai sollicité en vain à 2 ou 3 reprises la mansuétude de la Commission pour obtenir quelques délais afin de rédiger et de concerter correctement et différents acteurs sur d'autres ordonnances les les amendements que vous nous proposez vise à laisser un peu plus de temps, en terme de temps maximal d'ailleurs, c'est un temps plafond pour rédiger des ordonnances sur un sujet complexe que le gouvernement ne peut être que favorable aux amendements qui ont été présents. Alors voilà, nous avons sont ces 3 amendements, un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement, Monsieur Richard, demande la parole, explications de vote. Oui, Monsieur le Président, sur ces questions d'habilitation et de durée d'adoption des ordonnances les expériences sont variés Plutôt que d'évoquer disons des suspicions ou des jugements de principe, cité des des expériences, nous avons les parlements dans les législatures successives habilité les gouvernements successifs, a procédé à beaucoup de législation par ordonnances et le débat sur la brièveté de l'élaboration de l'ordonnance revient à chaque fois, je voudrais simplement signaler aux collègues qui se produit très fréquemment que les délais d'habilitation expire alors que l'ordonnance n'est pas terminée que donc une partie importante du travail et simplement perdu que fréquemment aussi les gouvernements sont amenés à demander au Parlement qui généralement y consent une prolongation des durées d'habilitation, donc comme le disait à juste titre le ministre à l'instant, ce dont nous parlons est simplement un délai maximum, c'est-à-dire c'est le délai au terme duquel, si l'ordonnance n'est pas publié tout le travail est à recommencer, donc je ne vois pas quel est l'inconvénient de prolonger le délai d'habitation alors que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intérêt, de représentants de l'intérêt général, sont favorables à ce que le texte Vienne plus vite mais je voudrais simplement souligner que les services. De production juridiques des ministères, à qui on demande de préparer ses textes avec beaucoup de concertations avec beaucoup de précautions pour éviter les malfaçons ne sont pas extensibles qui sont même en général en effectifs, en cours de réduction et je voudrais même livré un petit secret qui est que certains ministères n'ont même pas du tout ses services, j'en ai rencontré donc il me semble qu'il n'y a pas d'inconvénient sérieux sauf on ne vote pas une résolution canton de défini le le le la durée d'une d'une habilitation on donne simplement un délai maximum, tenant compte des aléas de production de ce texte, en revanche, je pense qu'on peut insister auprès du gouvernement pour aller un peu plus vite, et ça n'a pas d'inconvénient.

qui vote contre

écoutez, il y a doute le Faire-part ainsi lever parce qu'on est vraiment une voie donc ceux qui sont favorables à l'adoption de ces amendements veuillent bien se lever.

Oui, le présent projet de loi prévoit la remise d'un rapport dans les 4 ans suivant la promulgation des ordonnances mettant en application le nouveau cadre réglementaire prévue par les premiers paragraphes de l'article 34 or au regard de l'expérience actuelle, il semble peu probable qu'un nouveau parc éolien en mer, soit en fonctionnement d'ici 5 ans, soit un an de préparation des ordonnances, plus 4 ans pour produire ce rapport, or le rapport vise à mesurer et évaluer les effets induits par le nouveau cadre réglementaire sur les délais de réalisation et les nouveaux éléments, donc il me semble plus judicieux de propos afin de demander que ce rapport soit remis 12 mois après l'entrée en service d'un parc éolien en mer produits suivant le nouveau cadre réglementaire, telle est l'objet de l'amendement.

mais je je vous proposerais, mes chers collègues, d'en rester à la rédaction actuelle et ceci pour plusieurs raisons : la première dame très c'est la réforme est même envisagée et c'est bien son principal objectif doit permettre de réduire les délais à 4 ans sans recours et à 6 ans en cas de recours premières observations, deuxièmement, 4 ans après la publication de l'ordonnance, nous devrions donc disposer d'au moins un projet pour lequel le débat public en amont de l'appel d'offres aura eu lieu, l'État aura réalisé les études techniques préalables le lauréat aura déposé une demande de permis enveloppe, même si le parc ne sera pas encore construit les aspects essentiels de la réforme donc je rappelle qu'elle ne porte sur la construction, le même pourront être analysés 3ème point un repos sans davantage les chiens s'en éloigneraient d'autant la possibilité d'adapter les règles, si cela s'avérait nécessaire, au vu de ce 1er bilan et enfin j'ajoute qu'il est déjà assez ambitieux d'espérer du gouvernement qui n'oublie pas de me remettre un rapport de 24 ans 24 ans, pour ne pas le reporter comme cet amendement, le propose à 7 ans au moins, alors n'en parlons pas donc demain de retrait ou avis défavorable. J'ai Ministre pour le gouvernement. Merci monsieur le président, le gouvernement vous l'imaginez, fait confiance à la nouvelle procédure pour permettre la mise en oeuvre d'un parc éolien Offshore aussi rapidement que possible cependant la la proposition portée par Madame la sénatrice, la barre nous paraît de bon aloi et opportune effectivement dès lors qu'un parc sera créé, quel que soit le délai d'ailleurs, mais dès lors qu'un parc sera créé, il est bien évident que nous procéderons à une évaluation pour en tirer les conséquences et pour en tirer les leçons, les plus profitables possible de disposer d'une évaluation dans un délai de un an après la la création du 1er parc nous paraît tout à fait opportune, c'est la raison pour laquelle c'est un avis favorable à l'amendement qui est présente. Alors, un cas de figure, un petit peu. Monsieur le Président, je voudrais simplement vous dire que je soutiendrai cet amendement non pas j'entends tous les arguments propose hanté par notre rapporteur, mais vraiment que lorsqu'on est amené à travailler sur le sujet, on voit bien qu'aujourd'hui, le délai de 4 ans pour la nation n'a pas et que pratiquement impossible, le texte qu'il est prévu qu'ne fera que nous n'aurons pas toutes les données avec une véritable capacité à analyser, à la fois gérer les procédures et surtout les coups et surtout les coups en sachant que nous sommes dans un environnement qui est extrêmement mouvant, le code de la réglementation de l'énergie notamment du raccordement des ce Bush sans arrêt, donc si on n'a pas de regard là-dessus, c'est pour ça que, même si j'entends le l'inquiétude du retard faut globalement ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte que les parcs sont le plus rapidement possible qu'arranger tout le monde, mais aujourd'hui je pense que si on veut réellement à 20 capoeira des données qui puisse être utilisable sur l'avenir, je pense que cet amendement est plutôt logique dans la démarche. Aux demandes d'explications de vote Monsieur Durand. Je crois que les arguments développés par par nos collègues sont assez convaincants, va suivre leur position et l'avis du gouvernement. Les demandes d'explications de vote, je vais mettre aux voix, c'est un moment 15 rectifier retrait ou défavorables de la commission favorable du gouvernement qui vote pour. Eh bien écoutez, ça ne fait pas l'ombre d'un doute qui vote contre qui s'abstient l'amendement adopté nous en venons à l'amendement 53 rectifier du gouvernement Monsieur Ministre. Merci monsieur le président, le présent amendement a pour objet de donnèrent une base légale à 2 options : d'abord une éventuelle future renégociation des appels d'offres en matière de développement des capacités d'énergie renouvelable avec les lauréats, le but : parvenir à la réduction du tarif d'achat avec leur accord, afin d'améliorer l'offre jacente alors que le cadre actuel impose de signer le contrat d'achat aux tarifs initialement proposé une seconde option permettant de retirer les autorisations administratives, donner aux candidats retenus lors d'une procédure mise en concurrence, le cadre juridique actuel ne prévoit en effet aucune possibilité pour l'autorité administrative de revenir sur les résultats de l'appel d'offres et cette décision évidemment le cas échéant, emporterait une indemnisation du lauréat dans le cas des appels d'offres pour les énergies renouvelables, les et caractéristiques techniques et tarifaires sont prévus par un cahier des charges qui ne peut être révisé après l'attribution de l'appel d'offres, le constat fait aujourd'hui avec ce dispositif est trop rigide, notamment pour ce qui concerne les appels d'offres éolien en mer, par exemple, on ne peut pas améliorer la compétitivité d'un projet attribué, même si des technologies plus efficaces et de meilleures conditions de financement permettrait d'en diminuer le coût pour la collectivité publique et les échanges que nous avons eu tout à l'heure sur le fait qu'il puisse se passer 10 ans entre la sélection d'un lauréat et la mise en oeuvre du programme montrent que dans cette période, les conditions peuvent changer, il convient de rappeler par exemple que les seuls appels d'offres attribués entre une en 2012 et 2014 représente un coût pour les finances publiques de 41 milliards d'euros sur 20 ans pour une puissance installée de 3 gigawatts seulement dans certains cas, notamment lorsqu'elle promet le progrès technique permet d'envisager des baisses de coûts substantiels, l'État pourrait ainsi renégocier les conditions de l'offre retenue à l'issue de la procédure mise en concurrence, afin d'améliorer et en particulier d'en diminuer le montant du tarif retenu cet amendement est destiné à donner une base légale au résultat de cette négociation qui serait réalisé avec l'accord du lauréat, aujourd'hui, je le disais, certains projets mettent très longtemps à aboutir les projets éoliens en mer mettent actuellement entre 10 et 15 ans à sortir, entre-temps, les paramètres évoluent les coûts diminuent les éoliennes deviennent plus puissantes, les techniques s'améliorent et savoir-faire progresser et la filière se structure, le gouvernement propose donc au Parlement de se doter de la possibilité de tenir compte dans les tarifs de l'amélioration des projets et de renégocier les contrats, cet amendement ouvre également la voie à un retrait de la décision d'attribution des 6 projets éoliens Offshore attribué en 2012 et 2014, aucun contrat d'obligation d'achat mais signé suite à ces appels d'offres et aucune des installations prévues n'est construite le tarif qui a été accordé à ces installations est très élevé et ne correspond absolument plus aux prises actuel de l'éolien en mer, entraînant des rémunérations excessives pour les candidats retenus pour mémoire le tarif unitaire d'achat du kW/h prévue dans ces appels d'offres et plus de 5 fois supérieur au prix actuel du marché dans l'hypothèse d'un abandon complet des 6 champs couplé abandon couplé pardon une compensation intégrale des capacités perdues l'économie très significatif pour les finances publiques qui pourraient être dégagées à moyen terme, justifie que le gouvernement propose au Parlement de valider la base légale permettant sa mise en oeuvre.

pour nous donner la vie, les commissions. Très bien, merci, merci Monsieur le Président. Par cet amendement mais Monsieur le ministre vient de le rappeler, le gouvernement entend traiter de difficultés en permettant d'une part. Pour toutes les énergies renouvelables, d'améliorer, avec l'accord du lauréat une offre après l'attribution de marchés afin que cette nouvelle offre s'impose à l'acheteur obligé d'autre part, et uniquement pour les 2 premiers appels d'offres d'éoliennes en mer, de pouvoir retirer unilatéralement la décision d'attribution et donc le droit à subvention que le ou les lauréats concernés avaient pourtant obtenu si d'aventure il n'acceptait pas d'améliorer leurs enfants, c'est évidemment une seconde série de dispositions qui appelle l'examen le plus attentif. D'abord sur le plan juridique. Revenir sur ces droits, qui suppose une Hemdani station à hauteur du préjudice subi et un motif d'intérêt général, j'observe qu'une indemnisation est certes prévue mais qu'elle serait à l'État limité aux seules dépenses à engager et non à la perte du droit qui le motif d'intérêt général, lui, ne ferait guère de doute, compte tenu des sommes en cause pour la collectivité, ça c'était le 1er point, deuxièmement, sur le plan pratique. On comprend qu'il s'agirait pour le gouvernement de disposer de leviers pour inciter le lauréat à renégocier. Enfin, depuis 2011, il est certain que l'évolution des conditions de financement, la meilleure reconnaissance des risques et la maîtrise des technologies, permettraient de réaliser des gains significatifs, même s'il ne faut pas comparer les coûts des parcs attribués en 2012 ou 2014 avec ceux qui le sont aujourd'hui, je précise car il règne une faire une forme de confusion sur ce point qu'il ne s'agirait pas nécessairement de modifier les technologies utilisées, sauf à devoir Alain relancer tout à la procédure, mais bien de rogner sur certaines marges apparu depuis par exemple l'amateur de financement de provisions pour risques. La méthode retenue par le gouvernement et par ailleurs, excusez-moi, monsieur le ministre, assez brutal sur la forme comme sur le fond. Voir pourrait même s'avérer contre-productive pour les futurs appels d'offres. Les investisseurs potentiels pourraient en effet craindre. Sort identique leur être réservé et douter de la parole de l'État, ce qui est paradoxal zone texte qui prône dans le même temps, le retour de la confiance, vous l'admettrez. a fait une telle disposition pourrait remettre en cause l'émergence d'une filière industrielle française et je pense tout particulièrement aux usines et un certain nombre d'entre vous connaissez véritablement ces projets-là, les usines de sel Nazaire de Cherbourg ou du Havre, voilà, mes chers collègues, et c'est important ce que je vais dire autant de risques qui ont conduit notre commission a donné un avis défavorable à cet amendement. Mais j'ajoute, à titre personnel. Que s'il est parfaitement légitime hier et examiner l'équilibre économique de ces projets, cela ne peut se faire qu'au travers de négociations avec le lauréat, donc j'espère qu'à l'aboutira dans les meilleurs délais, notamment pour purger ce dossier à Bâle la semaine du 3ème appel donc. En clair, laissons l'Intelligence. Réagir Des porteurs de projets pour qu'il revoie par la suite avec l'État, dans quelles conditions ils peuvent renégocier mais ne remettant pas rappela la salle des projets qui sont avancés jusqu'à aujourd'hui, donc il vous est proposé, vous l'imaginez, un avis défavorable. Je rapporteur alors vous êtes nombreux à avoir demandé la parole, on commence par monsieur Oui, merci Monsieur le Président et hier, le gouvernement a été par les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire par courrier le 1er ministre donc le gouvernement que vous représentez, Monsieur le Ministre, font part de leur étonnement quant à l'absence de concertation tant avec les acteurs de la filière qu'avec les collectivités territoriales concernées qui apprécie présidé au dépôt de cet amendement dans le caractère rétroactif est en outre de nature à amoindrir la confiance des investisseurs comme des industriels de la filière, mais aussi à fragiliser l'engagement de la parole de l'État, nous tenons également vous exprimer nos plus vives craintes quant aux conséquences de l'adoption d'une disposition qui pourrait conduire l'État à reporter de plusieurs années, le lancement de ce parc éolien Offshore alors que notre pays accusant déjà un retard significatif, encouragé par le gouvernement, nos régions ont par ailleurs investi dans les infrastructures portuaires afin de maximiser les retombées économiques des projets en France, plus de 600 millions d'euros ont été mobilisés, notamment par rapport aux appels d'offres de 2012 et 2014, alors nous sommes d'accord que pour l'éolien, il y a un tarif public Monsieur le Ministre, nous avons connu à peu près la la même chose il y a une dizaine d'années sur le photovoltaïque également puisque il y a eu un changement de politique sur le financement de du photovoltaïque devant l'engouement des investisseurs, grands ou petits d'ailleurs à l'époque pour cette filière, beaucoup plus dur d'ailleurs un effet d'aubaine que par une conversion intellectuelle et on peut le regretter d'ailleurs philosophique aux énergies renouvelables et la lutte contre le réchauffement climatique, ce soir, je m'en avait été acté à partir d'une date qui n'était pas rétroactive postérieurs à la décision par rapport à ce qui nous est proposé aujourd'hui, je rappellerai également que le grand Ouest, c'est vraiment le pays de la Loire ont été pénalisés économiquement par l'annonce de l'abandon de renoncement de l'aéroport du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes il y avait d'ailleurs l'État s'était engagé à produire un contrat d'avenir qui me semble plutôt sombre, puisque nous n'avons rien pour l'instant pas une ligne décrites et que nous avons des inquiétudes pour l'avenir de la centrale thermique de Cordemais, la raffinerie longe le grand port de Nantes-Saint-Nazaire les dysfonctionnements réguliers de TGV et TER, elle annonce également d'Airbus d'une réduction des effectifs, voilà je voulais rappeler le gouvernement à ses engagements précédents merci. Merci, vous êtes encore 8 à vous êtes inscrit, donc nous serons obligés de suspendre avant d'avoir terminé de la à toutes et à tous, mais nous reprendrons ensuite monsieur Courteau. Monsieur le Président, oui, c'est un engagement est pour le moins surprenant mais surtout inquiétant quant à ses conséquences s'il était adopté, en proposant notamment de mettre unilatéralement de manière rétroactive à tout projet lauréats de l'appel d'offres d'ailleurs pas encore sécurisé son contrat d'achat, l'État va créer une instabilité sans précédent qui, effectivement, comme cela a été dit a instantanément la confiance des investisseurs ainsi que la comme dès industrielle et de l'État qui place dans l'État, si cet amendement comme cible dans les faits, essentiellement la filière Offshore, il constitue un précédent désastreux, avec la possibilité de remettre en cause tout projet renouvelable sélectionnés par appel d'offres, un mandat été inquiétant au regard des enjeux et des impératifs de la transition énergétique et il est préoccupant pour l'image de la France, porteuse de l'accord de Paris et pour son attractivité sur la scène internationale, je rappelle que les objets qui l'homme vicieux la France ainsi que son engagement dans la lutte contre le dérèglement climatique impose une diversification du mix énergétique, notamment grâce au développement des filières renouvelables innovantes éoliennes en mer, en fait partie. Et justement, l'éolienne en mer fait partie de ces filières d'avenir dans laquelle les acteurs et les territoires français ont considérablement investi et dont ils attendent beaucoup en terme d'emploi comme de retombées locales je rappelle également que l'État s'est aussi donné pour objectif d'installer 3000 mégawatts de capacité éolienne en mer à l'horizon 2023, une remise en cause de certains de ses projets conduirait l'État à renoncer à cet objectif, puisqu'il ne sera pas possible au regard des délais de développement des projets éoliens en mer 8 9 10 ans compte 2, 3 ou 4 ans chez nos voisins européens, de construire et de mettre en exploitation de nouveaux projets, à cette date, c'est un demandant retarderait les échéances, nous empêchant d'atteindre nos objectifs et ruinerait la confiance que l'on porte à l'État français, donc merci de de rejeter cet amendement. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, comme mes 2 prédécesseurs, je suis également contre cet amendement du gouvernement je ne reviens pas sur la forme, notre rapporteur, Monsieur Lüscher a parlé de brutalité, c'est vrai, c'est arrivé comme ça, de cette manière-là, c'est vraiment un drôle de texte compte observe qu'on analyse aujourd'hui au Sénat, donc, cet amendement, mais c'est un mauvais coup, ça a été dit, c'est un mauvais coup pour la filière, en général, notre collègue tout à l'heure, parlait de choix de société, c'est vrai que si on veut faire le choix d'énergie des carboniser dénucléarisé énergie en éolien et Offshore en est un exemple et donc là on peut que regretter vivement ce coup d'arrêt que vous faites sur les 6 projets qui sont déjà partis et pour parler plus précisément de celui que je connais un peu plus en Loire-Atlantique, qui est mon territoire c'était vraiment un mauvais signal qui est donné là à la fois au département, mais aussi sur la région, ça a été dit par mon collègue Priou, donc je voterai contre cet amendement en redisant encore une fois que pour recréer, redonner confiance aux territoires aux collectivités, quelles qu'elles soient les villes de métropole, le département, la région, ce n'est pas du tout une bonne manière de s'y prendre sur ce domaine-là. Merci, la parole est à madame Agnès Canayer. Offshore polarise depuis de nombreuses années l'énergie des défenseurs, dont je fais partie et des opposants en Seine-Maritime, les 2 chansons prévu Fécamp et Dieppe, Le Tréport subissent depuis près de 10 ans, les aléas d'une procédure complexe, mal ficelé et donc tous les sauts et soubresauts des autorisations des recours successifs qui repousse encore et encore leur réalisation conséquence aujourd'hui évidemment les conditions ne sont plus les mêmes, tant en ce qui concerne les solutions techniques que l'économie, l'équilibre économique de ces projets, la renégociation des conditions et donc justifié pour recourir aux avancées technologiques, notamment les nouvelles turbines et limiter l'impact sur les finances de l'État 2 c'est la construction de ces champs, des renégociations ne peuvent se faire sous la contrainte, avec effet rétroactif, comme le propose l'amendement du gouvernement qui crée un véritable risque pour la filière de l'éolien maritime, au Havre, donc je suis élue, l'enjeu est fort, plus de 60 millions d'euros ont déjà été investis par les collectivités territoriales, sur le terrain du Grand port maritime pour permettre la création de 750 emplois prévus par Siemens, je voterai donc contre l'amendement pour des raisons plus de forme que de fond car la méthode n'est pas la bonne, elle n'associe pas les acteurs économiques et les élus locaux, elle impose de manière unilatérale la nécessaire révision des conditions financières négocié conjointement. Merci, la parole est à Hollande Françoise Gatel. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre vous solliciter notre indulgence tout à l'heure, elle vous est acquise, mais pour ma part, je ne vous ai quitteraient pas de l'amendement que vous proposez, vous posez une enfin, vous faites un constat qui est excellent, c'est-à-dire que le retard que la France a prise dans la structuration d'une filière génère des coûts considérables, mais la réponse que vous apportez me semble pardonnez-moi à courte vue et contre-productive, et je me permettrai de citer un exemple que Jean-Yves Le Drian connaît bien parce qu'il a signé un pacte électrique breton avec la région je voudrais donc à partir de cet exemple montrer à mon avis, le côté contre-productive de la solution que vous proposez, vous savez que, en Bretagne, nous avons un déficit de production électrique assez considérable et un pacte électrique a été signé entre l'État, la région Bretagne en 2010 Les énergies marines renouvelables, soit une partie importante de cet objectif de la diversification de production puisque la région et l'État conjointement envisage une production d'énergie renouvelable, à partir de ces EMR à hauteur de 32 pourcent de la consommation électrique bretonne, les retombées économiques sont très fortes et en lien avec l'État, le projet de la baie de Saint-Brieuc a été accompagné par la région, en contrepartie d'un schéma industriel propice au développement d'une filière française consacré aux énergies marines renouvelables, ce qui n'existe pas aujourd'hui les retombées économiques constitue un point central, je parlerai de la localisation du lot fondation à Brest et en France de 1860 emplois, dont 500 emplois à temps plein à Brest et il s'agit là, en plus, monsieur le ministre d'une opportunité de reconversion de filières industrielles en des prises comme celle de la construction et de la réparation navale à ses employes s'ajouteront inévitablement des recours important en sous-traitance locale donc, pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, mais votre amendement me paraît très nocive à l'instauration d'une filière française et votre proposition d'amendement contrevient aussi à des accords de partenariat engagé entre l'État et la région, sans parler de l'émotion que va à nouveau susciter la renégociation de l'accord sur lesquels vous savez que nous rencontrons régulièrement des oppositions de l'opinion publique, difficile à gérer, je vous remercie. nous n'avons plus le temps de les écouter avant la suspension, je vais donc suspendre la séance sera reprise. à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte.